La séance est reprise, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue que James Marson, qui fut sénateur de la Seine-Saint-Denis de 1975 à 1986. Lors du jour Lors du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances adoptées par l'Assemblée nationale pour 2018 : nous poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions le Sénat va examiner les crédits de la mission sécurité au pluriel et article 62, terre et 62 quater du éduquons spécial, contrôle de la circulation et du stationnement, routiers et article 67. La parole est à monsieur Philippe Dominati, rapporteur spécial de la commission des finances pour les programmes, police nationale et gendarmes ne rit nationale pour 7 minutes. Monsieur le président, Monsieur le ministre, chaque allègue avant d'aborder l'examen de cette mission je souhaite saluer l'efficacité et le courage de nos forces de l'ordre, dont la mobilisation est particulièrement forte, leur activité opérationnelle s'effectue dans un contexte de grande tension. Comme en témoigne par exemple le les plus de 900 perquisitions administratives menées en 2016 au titre de l'état d'urgence où les millions de contrôles aux frontières mené au titre du rétablissement temporaire de ces dernières, je veux également rappeler ici avec gravité les nombreuses suicides qui ont eu lieu ces dernières semaines. Pourtant, malgré le caractère prioritaire de cette mission, le présent projet de budget ne semble pas être à la hauteur des enjeux. Premièrement, l'évolution des crédits est en baisse dans la loi de programmation triennale. Si en 2018, les moyens de la police et de la gendarmerie nationale sont en légère hausse mais évolution prévisionnelle des crédits de la mission sécurité sur le triennal

En prenant en compte les prévisions d'inflation du gouvernement mais évolution des crédits sera négative et diminuera de 0,4 Cette évolution est surprenante alors que la sécurité nationale est toujours présentée comme une priorité par ailleurs la mise en place une politique de sécurité quotidienne ne s'accompagne d'aucun volet budgétaire et devrait donc ça puis et sur les moyens existants. Les annonces faites ne dissipent donc pas à ce stade, la crainte de voir émerger un nouveau dispositif créant une charge de travail supplémentaire pour les forces de l'ordre, deuxièmement la hausse des effectifs s'effectue au détriment des moyens de fonctionnement et de l'investissement. Perpétuant ainsi la principale faiblesse des Budgets de la fin du quinquennat précédent s'il est vrai que le total des créations d'emploi était de 8837 postes au cours de ces 5 dernières années, le rythme de recrutement devrait sensiblement s'accroître sur le quinquennat actuel puisque le président de la République s'est engagé à créer 10000 emplois sur la période 2018, 2022 pour renforcer les forces de sécurité intérieure, dans ce cadre, la police nationale, bénéficiera de 7500 ETP, la gendarmerie nationale de 2500 unités ainsi le nombre de policiers, de gendarmes devraient augmenter en 2018, 2835 ETP, 459 pour les gendarmes et 1376 pour les policiers. Mais la conséquence de cette constante augmentation des effectifs depuis 2014 et que la part des dépenses de personnel sur l'ensemble des crédits au sein des 2 programmes atteindra 86,78 pourcent en 2018, ce ratio ne permettra pas de garantir la capacité opérationnelle des policiers et gendarmes. Depuis 2006 en 10 ans, les dépenses de personnel ont augmenté de plus de 31 pourcent, tandis que les autres dépenses ont connu une baisse de 4,98 je rappelle par ailleurs que les comparaisons internationales ne témoigne pas d'une sous-dotation des forces de sécurité intérieure de notre pays, bien au contraire parmi nos principaux voisins européens, seule l'Italie a des effectifs supérieurs aux nôtres. Troisièmement, le maintien de ce ratio à un niveau aussi élevé induit désormais une paupérisation de nos forces, la faiblesse des dépenses d'investissement et de fonctionnement, a des conséquences directes sur le vieillissement du parc immobilier, on peut prendre un exemple, les loyers de la gendarmerie pour 114 millions d'autorisations d'engagement et 92 millions de crédits de paiement et le plan nécessaire sur 5 ans pour résorber la dette de ses loyers le budget présenté ne permettra pas d'assurer un abaissement de l'âge de la flotte de véhicules également en constante augmentation, 4 ans et 10 mois en 2006 qui atteint 6 ans et 9 mois en 2016 alors même qu'il y a de moins en moins de véhicules depuis 2006 un véhicule de police est supprimé lorsque 3 postes sont créés. L'équipement des agents va également pâtir d'un important sous-financement plusieurs centres de tirs ont dû fermer depuis septembre, d'où un fort mécontentement des forces de police et de gendarmerie qui ne peuvent s'entraîner que 12 heures annuellement et ne tirer que 92 cartouches par an quatrièmement une meilleure organisation des forces auraient permis de gagner en capacité opérationnelle, l'application de la directive européenne de 2003 relative au temps de travail, de la gendarmerie pour la première fois à partir de 2017 a ainsi engendré une baisse de la capacité opérationnelle des forces de 5 pourcent des ETP, comme je l'avais prévu l'an dernier les recrutements prévus ne compenseront donc pas l'application de cette directive pour la police nationale, l'entrée en vigueur de la vacation forte devrait entraîner en 2018 une perte opérationnelle celle vend à 433 ETP, mais il est possible que davantage d'effectifs soit à terme concerner par ce si par exemple il n'est pas appliquée à la préfecture de police de Paris, la perte opérationnelle pourrait s'accroître dans les années à venir, et cette réforme peut donc toujours être qualifié de bombe à retardement, le principal levier permettant de dégager des effectifs et le recentrage des forces de l'ordre sur leur coeur de métier par la suppression progressive des tâches indues qui mobilise l'équivalent d'environ 6000 ETP, je pense notamment au transfèrement judiciaires à la gestion des procurations et aux tâches administratives qui détourne et forces de l'ordre de leurs missions premières je vous présenterai donc un amendement visant à substituer des crédits du titre de par des crédits d'investissement et de fonctionnement afin de donner les moyens aux hommes de copieur leur mission, cet amendement doit être interprété comme une volonté d'aboutir à une vision constructive dans le cadre de ce budget sur un sujet aussi important pour notre pays, si le gouvernement veut pour ce 1er budget du quinquennat maintenir sa version initiale, si peu conforme aux exigences de la situation, votre rapporteur vous proposera le rejet des crédits de la mission sécurité je vous remets. La parole. Et maintenant à monsieur Jean-Marc Gabon qui, rapporteur spécial de la commission des finances pour le programme, sécurité, éducation routière. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais maintenant évoquer un autre fléau particulièrement meurtrier l'accidentalité routière cercle : augmentation du nombre de morts tend à décélérer en 2016, 2017 mais la courbe de la mortalité routière, mais toujours pas inverser la France vient de connaître 3 années consécutives de légère augmentation du nombre de victimes de la route, l'objectif que s'était assigné le gouvernement de Manuel Valls descendre sous le seuil des 2000 morts en 2020 paraît de plus en plus hors de portée. En effet, sur les 10 premiers mois de l'année 2017 on dénombre encore 2878 personnes tuées en France métropolitaine, soit plus de 9 par jour, tandis que le nombre d'accidents 160 par jour et 2 blessés, plus de 200 par jour continue d'augmenter. Ce bilan doit cependant être restitués dans l'espace et dans le temps évidemment la mortalité routière est bien moins élevé que dans les années 70 où le nombre de décès de mort, dépasser les 18000 réduire encore la mortalité et donc de plus en plus ardu. Néanmoins, sur le plan européen, la France ne se situe qu'au 14ème rang de plus lorsqu'on tient compte de la distance parcourue sur les réseaux routiers, la mesure se fait en en milliards de kilomètres parcourus plusieurs de nos voisins comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse font mieux que nous, donc une marge de progression existe encore. La politique et la politique de sécurité routière telle qu'a été infléchie en 2015, n'a pas encore produit de résultats sensibles et ne saurait être centrée que sur les seuls radars, elle doit s'accompagner d'une lutte intensive contre les causes, les autres causes d'accidentalité tels que l'alcool, les stupéfiants ou l'inattention et d'une politique de progrès de prévention renforcée dans l'efficacité doit être encore mieux évaluer. On arrive maintenant au programme, sécurité, éducation routière de la mission sécurité Jean viendra ensuite au compte spécial sur le programme, sécurité, éducation routière, je note que les dépenses inscrites augmente légèrement, de près de 3 pourcent de 38,8 millions d'euros en 2017 à 39,9 millions d'euros en 2018 je salue également l'effort de sincérité des dépenses de communication régulièrement sous budgété ces dernières années, elles ont été nettement relevé pour 2018 j'observe également que le ralentissement de l'opération, permis à un Euro par jour semble se confirmer, malgré la création d'un prêt complémentaire de 300 euros, pourriez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, si vous envisagez de relancer ce dispositif de permis à un Euro par jour sur le qu'on affectations spéciales contrôlent la circulation et du stationnement routier dit-on dit-on d'affectation spéciale radar mes observations sont les suivantes : le produit total des amendes de la circulation et du stationnement devrait atteindre en 2018, 1 milliard 830 millions d'euros et sur cette somme, 73 pourcent sont inscrits en dépenses du compte d'affectation spéciale radar, ce qui représente un milliard 340000 euros, soit un montant en légère baisse de 3,6 pourcent par rapport à 2017, la politique du nouveau gouvernement s'inscrit pour le moment dans celles arrêtées par le comité interministériel du d'octobre 2015, cette stratégie qui s'appuie sur le déploiement de nouveaux radars, moins prévisible et dotée de nouvelles fonctionnalités et le remplacement du point de contrôle par le parcours sécurisé devrait commencer à porter ses fruits, toutefois l'implantation et le parcours de ces équipements, je pense notamment aux voitures radars doivent être mieux liés à la carte de l'accidentalité l'objectif demeure bien entendu, la diminution du nombre d'accidents et de morts, et non l'augmentation du produit des amendes et départements d'outre-mer et les réseaux routiers secondaires ou l'accidentalité particulièrement élevé doivent notamment être privilégiée, je vous renvoie sur ce sujet au rapport d'information notre collègue Vincent Delahaye, dans le cas de sa mission de contrôle budgétaire. Le développement des radars tronçon vitesse moyenne mieux accepter des usagers doit être encouragée, tandis que l'alternance des limitations de vitesse doit être rationalisée et encore mieux signaler trop de conducteurs en effet dépasse la vitesse maximale autorisée parce qu'ils n'ont pas perçu un changement de limitation vitesse, la réglementation, pardon, sur les limitations de vitesse doit être défini en considération de l'état d'une roue de sa dangerosité et de l'accidentalité et non pas en fonction de son statut qu'on entend parler actuellement pour les routes nationales. Afin d'améliorer les résultats de la sécurité routière, ces acteurs et notamment les collectivités territoriales, les usagers, les employeurs, sans oublier les concessionnaires d'autoroutes doivent être encore mieux associés à la définition de cette politique à cet égard je propose 2 amendements qui réduisent l'ampleur de la baisse des versements Servent collectivités locales pour améliorer leurs infrastructures routières, l'impact de la décentralisation du stationnement payant est en effet à ce stade encore difficiles à apprécier, y compris au niveau de son impact financier à court terme, il semblerait donc imprudent de trop anticiper sur les effets de cette réforme par ailleurs la dimension interministérielle de la politique de sécurité routière doit impérativement être renforcés, le comité interministériel de sécurité routière ne s'est réuni que 2 fois depuis 2 1000 ans, pourriez-vous nous confirmer, monsieur le ministre, un prochain comité va bientôt être réunis et nous annoncer quelles inflexions vont être apportés à la stratégie arrêtée en 2015 afin d'améliorer ses résultats. S'agissant de la gestion du permis à points, il est prévu en 2018 plus de 22 millions de lei de notification ou de retrait de points soit adressée au conducteur pour une dépense estimée de 17,5 millions d'euros, je note pour la première fois l'effort de dématérialisation d'une partie de ces courriers cependant cet effort, qui ne couvre en 2018 que 10 pourcent des crédits de ce poste doit être poursuivie dans la mesure où il permet d'engendrer des économies de traitement des documents, enfin, je constate une fois encore que le fonds de roulement de l'entaille au 1er janvier 2017 s'avérait plus de 2 fois supérieur au niveau préconisé à hauteur de pratiquement 37 millions d'euros, je proposerai donc un amendement qui vise à diminuer les crédits qui lui sont destinées, en effet, les justifications apportées par les documents budgétaires et les réponses au questionnaire me semble à ce jour peu probante sur l'évolution de ce besoin notamment le besoin en fonds de roulement, mais peut-être que le gouvernement pourra nous apporter des précisions sur ce point, en conclusion, la commission des finances propose donc d'adopter les crédits de la mission dans sa partie sécurité routière sans modification et ceux du compte spécial ainsi modifiées, je vous en mer. Merci, monsieur, la parole est maintenant à Jean-Pierre Vogel, rapporteur spécial de la commission des finances pour le programme sécurité civile. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, les crédits du programme Sécurité civile qui ne représente que 54 pourcent de dépenses de l'État en crédits de paiement consacré à la sécurité civile, au sens large, connaissent cette année une hausse importante, les crédits de paiement et les autorisations d'engagements demandés sont ainsi en augmentation de respectivement 5,36 pourcent et 80 2,34 pourcent par rapport aux crédits votés en loi de finances initiale pour 2017 cette hausse importante s'explique toutefois par les autorisations d'engagement affectés au renouvellement de la flotte d'avions traqueur, qui représente en 2018 404,1 millions d'euros en en autorisation d'engagement et 60 et 1,4 millions d'euros en crédit de paiement si on neutralise l'impact de l'acquisition des avions dans le budget 2017 et 2018 le budget or titre 2 du programme sécurité civile et stable en AE, plus 0,3 pourcent est en baisse en crédits de paiement, moins 5 le renouvellement de la flotte de traqueur était devenu indispensable en raison de son vieillissement, qui avait atteint 60 ans, et de l'atteinte prochaine du potentiel de vol maximale fixée à 25000 euros à cet effet, le marché d'acquisition d'un avion multirôle s'inscrivant dans le contexte du retrait des services de service d'avions traqueur avait été lancé dès 2016, le ministre de l'Intérieur a confirmé en juillet 2017, que ces derniers seraient remplacés par 6 bombardiers d'eau d'eau multirôle de type Dash 8 sans que ce choix ne soit formalisé juridiquement si ces avions présente l'inconvénient d'être particulièrement coûteux leur caractère multirôle plaidaient en leur faveur les Daschle 8 ont en effet pour principal Avantage de pouvoir être convertis en avion de transport, ce qui n'était pas le cas des traqueurs, on ne peut donc que se féliciter de ce renouvellement, il ne doit toutefois pas masquer le vieillissement du reste de la flotte qui entraîne de nombreuses indisponibilités. Nous l'avons en effet vu cette année, les pilotes d'avions bombardiers d'eau se sont plaints de l'indisponibilité de la flotte qui s'est parfois élevé à 25 pourcent, et ce en pleine saison des feux c'était égard je plaide pour qu'une rénovation des Canadair sont envisagés le plus tôt possible par la DGAC essaie pour pallier ces indisponibilités éviter les surcoûts liés à une prise en compte, trop tardive des problèmes. Le budget 2018 est aussi marquée par la poursuite du déploiement du essayent P, le système d'alerte et d'information des populations dont les choix stratégiques fortement contestable ne sont toujours pas remis en cause, je vous avais alerté monsieur le ministre, par le biais de mon rapport d'informations du fait que ce projet concentré près de 80 pourcent des crédits prévus au volet sirène alors même que leur impact apparaît beaucoup plus faible que celui de la téléphonie mobile, qui ne bénéficie pourtant que de 3 pourcent des crédits consommés ou prévues pour ce budget après un an de fonctionnement et à la suite des recommandations formulées dans mon rapport, l'application smartphone, donc j'avais relevé les insuffisances, fait l'objet actuellement d'une évaluation par l'inspection générale de l'administration qui doit se prononcer sur les améliorations possibles et les technologies Gisèle terre natif pose pouvant être mises en oeuvre à ce type Monsieur le Ministre, je vous serais reconnaissant de nous faire connaître, si vous avez eu les conclusions de l'inspection générale parce que, naturellement, cette évaluation est la bienvenue mais il me semble nécessaire de procéder à une réorientation stratégique plus large de ce projet avant que l'affectation des crédits de la phase 2 qui débute en 2020 ne soit effectué, enfin il me semble important d'évoquer la situation financière des SDIS services départementaux d'incendie et de secours, dont les Budgets ont diminué de 1,27 pourcent en valeur brute de 1,47 pourcent en volume en 2016 alors même que le nombre d'interventions qu'il réalisa poursuivi ça : hausse de 2 pourcent pour atteindre près de 4 millions et demi d'intervention, cette baisse des Budgets doit être compensée par la multiplication des mesures visant à parvenir à une meilleure maîtrise des dépenses des SDIS, qui passe notamment par une meilleure mutualisation à cet égard la réduction du nombre de numéros d'appel d'urgence et la recherche d'une plus grande mutualisation avec le SAMU, ainsi qu'entre les SDIS doit être impérativement poursuivies cependant le point le plus alarmant, me semble être l'évolution des dépenses d'investissement des SDIS, moins 4,58 pourcent en 2015 et moins 6,49 pourcent ces baisses ne peuvent se poursuivent sans entraîner une perte de leurs capacités opérationnelles le gouvernement ne me semble pas avoir pris la mesure du problème puisque la dotation aux investissements structurels en 2018 est en baisse de 62 cette dotation sera très majoritairement consacré au financement du projet de système d'information unifié desdits c'est de la sécurité, le SGA SG au projet considéré comme stratégique par le ministère de l'Intérieur et me semble-t-il, à juste titre, de l'avis général, cependant, son montant, 10 millions d'euros en AEC paient pour 2018 et très sensu très insuffisant, il me paraît donc indispensable que cette dotation soit réévaluée dans les années à venir, je vous remercie. Maintenant, la parole est à monsieur Philippe Paul, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour le programme de gendarmerie nationale et maintenant c'est 3 minutes par orateur. Monsieur le président, Monsieur le Ministre d'État, mes chers collègues, je souhaite d'abord rendre hommage aux personnels de la gendarmerie nationale qui ont montré la force de l'engagement tout au long de l'année 2017 en particulier outre-mer après le passage de l'ouragan Irma. Si les crédits du programme 152 prévue pour 2018 ne paraissent clos Balmont satisfaisant, je souhaiterais néanmoins attirer l'attention sur le problème posé par l'obsolescence de certains matériels. Il s'agit des capacités prix pivot décrite par le livre blanc de 2013 que je cite la gendarmerie mettra en oeuvre des capacités pivot, hélicoptères, véhicules blindés de maintien de l'Ordre réseau national durcit de transmission qui s'inscrivent en complémentarité des moyens des armées. S'agissant d'abord véhicules blindés, la capacité de la gendarmerie est prévue à la hauteur de 90 véhicules actuellement, il reste 71 véhicules blindés à roues datant de 1974 complété par 20 véhicules de la avons lundi racheté à l'armée de terre lors d'engagement en Afghanistan ces matériels sont actuellement. Très sollicité outre-mer et des renforts devraient être déployés en Nouvelle-Calédonie pour le référendum de 2018. Le remplacement de ces véhicules très usés par 99 nouveaux véhicules tout-terrain représenterait un coût d'environ 45 millions d'euros, en second lieu, la gendarmerie nationale emploie 26 hélicoptères de type Écureuil affichant un âge moyen de 32 ans, il serait nécessaire de remplacer les 10 modèles les plus obsolète par DEC 145, le montant total serait d'environ 140 millions d'euros, plus 6 millions et demi annuel pour le maintien en condition opérationnelle, j'ajoute, pour être complet sur les capacités pivot, le système de transmission durci, il faut également renouvelé pour un coût d'environ 10 millions d'euros. Par ailleurs, la vétusté de cet hélicoptère du groupe inter-d'hélicoptères qui constituent un outil essentiel puisqu'il permet au GIGN et aurait de se projeter pour la défense des centrales nucléaires est également préoccupante, il s'agit en effet de vue plus mode des armées de l'air et de terre, il est indispensable d'envisager l'remplacement par des hélicoptères de transport moyen de type Caracal, soit une dépense d'environ 125 millions d'euros dans le cadre du budget des armées si nous voulons préserver la capacité de projection de nos corps d'élite au total en ce qui concerne le budget de la gendarmerie, il s'agirait d'une dépense d'environ 200 millions d'euros, monsieur le Ministre, candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron a clairement exprimé sa vont et de mettre en place, je reprends là son programme une véritable programmation sur 4 à 5 ans pour la modernisation des moyens de la sécurité intérieure. Certes, le renseignement une compense Jean majeur de la sécurité intérieure, mais ce n'est pas la seule cet effort de modernisation doit aussi porter sur les équipements que je viens d'évoquer de manière à assurer l'avenir de cette capacité essentielle : l'intervention de la gendarmerie pendant plusieurs décennies, compte tenu de la durée de vie de ces matériels, bien entendu, il faudra y ajouter parallèlement le remplacement de ces Pumas du jeu, ce qui relève de la ministre des armées, de la loi de programmation militaire sur ses réserves commission donner un lit à l'adoption des crédits prendre 152 je vous. Merci. Merci. Monsieur Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères et de la Défense et des forces armées pour le programme, gendarmerie nationale. C'est le président, Monsieur le Ministre d'État Michard. Avec une hausse modérée des crédits une progression d'environ 500 emplois le budget de la gendarmerie nationale pour 2018 devrait permettre aux gendarmes de continuer à exercer leur mission de manière correcte premières aspects positifs, l'augmentation des personnels bénéficiera en priorité à la gendarmerie départementale, et je pense que les élus, ils seront particulièrement sensible, l'élargissement en 2018 de l'expérimentation des brigades territoriales de contact qui sont déchargés de tâches s'administrative et se consacrent au contact avec la population et les élus me paraît également aller dans le bon sens nous pouvons aussi saluer l'achèvement du déploiement des 75 les 65000 pardon équipements mobiles du plan néo-jaune au profit des gendarmes, les unités opérationnelles, c'est évolution devrait améliorer la productivité des gendarmes valoriser leur travail quotidien et simplifier l'accomplissement de leur tâche, à côté de ses aspects positifs, je souhaiterais évoquer 2 sujets de préoccupation. S'agissant d'abord de l'application de la directive temps de travail dans la gendarmerie nationale, il a déjà été dit que l'application depuis septembre 2016, des règles relatives au repos quotidien de 11 heures à globalement conduit à une perte d'activité équivalant à 6000 emplois temps plein d'un côté le fait que les gendarmes bénéficient d'un temps de repos convenable est un conseiller simplement une bonne chose et nous savons que cette nouvelle pratique hé bien perçu de l'autre, il y a l'exigence de disponibilité propres à l'état militaire et la nécessité de préserver le niveau d'activité de la gendarmerie face à tous les défis qui se présentent aujourd'hui, c'est une question particulièrement délicate, une remise en cause totale de cette réforme pourrait être difficile alors que des aménagements peuvent être acceptées, à défaut de nouveaux recrutements pour compenser l'effet de la directive, mais peu probable, nous en avons conscience en cette période de rigueur budgétaire, nous suivons donc ce sujet avec une vigilance tout à fait particulière, un 2ème, point de préoccupations et la question de la dette des loyers, je rappelle que la dette des loyers de la gendarmerie s'élève actuellement à 110 millions d'euros en autorisation de de programmes 89 millions en crédits de paiement, ce qui grève d'emblée l'exercice 2018 vous avez toutefois indiqué, Monsieur le Ministre, que l'apurement de ses dettes de loyer, fera l'objet d'un plan pluriannuel financé à hauteur de 13 millions d'euros dès l'an prochain, permettant ainsi à la gendarmerie de ne pas trop rogner sur ses dépenses d'investissement 2018 pour rembourser la dette, pourriez-vous nous dire si vous envisagez dès à présent un financement supplémentaire pour ce plan ou s'il s'agit seulement à crédit constant de lisser la dépense au total sauveur de ces quelques préoccupations et compte tenu de l'augmentation prévue des crédits et des personnels de commissions en conséquence, a donné un avis favorable au crédit qui sont dédiés à la gendarmerie nationale pour 2018, je vous remercie.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État mais, chers collègues, la commission des lois partage pleinement et totalement le constat présenté par notre collègue rapporteur spécial de la commission des finances cette consolidation budgétaire que nul ne peut nier demeure très largement insuffisante au regard de la dégradation très avancée de la situation de nos forces de sécurité intérieure et du contexte sécuritaire. Monsieur le ministre d'État, votre gouvernement a fait le choix, comme le précédent de mettent l'accent sur l'augmentation des effectifs, on annonce 10000 créations d'emplois de policiers et de gendarmes sur la durée du quinquennat exactement 7500 pour la police et 2500 pour la gendarmerie, mais en 2000 18376 emplois seront créés dans la police et 459 dans la gendarmerie ne nous limitons toutefois pas aux seules annonces nous connaissons l'impact dramatique sur les capacités opérationnelles de nos forces de la directive européenne du 4 novembre 2003 sur le temps de travail, selon les informations qui m'ont été communiquées les créations de postes annoncées permettront tout juste, tout juste de combler cette réduction des capacités opérationnelles, il y a là un véritable sujet de préoccupation, que le gouvernement paraît avoir écarté de ses calculs je souhaiterais, monsieur le ministre d'État, que vous puissiez nous apporter des réponses sur ce point, la principale difficulté de ce budget réside toutefois dans l'insuffisance des dotations de fonctionnement et d'investissement alloués à la police comme à la gendarmerie nationale ce que relève à l'unanimité, à l'unanimité, les forces de sécurité sans distinction de corps de grades, de niveaux d'exécution ou d'affectation, Monsieur le Ministre, ce n'est pas tant le manque d'effectifs, mais plutôt les conditions matérielles dans lesquelles il travaille désormais difficilement acceptable et soutenable, les sujets de préoccupation sont multiples, je ne citerai faute de temps, que quelques exemples, les équipements tout d'abord une mise à niveau des armements ils équipements de protection a été engagée au cours des dernières années, en revanche, l'état des parcs automobiles est aujourd'hui très préoccupant l'état moyen, des véhicules de la police et de 6 ans et 9 mois, il dépasse 8 ans dans la gendarmerie et plus de Centre 30000 kilomètres de moyenne au compteur, l'effort budgétaire consenti en 2018 est loin d'être à la hauteur des besoins de renouvellement. Autre sujet majeur de préoccupation, l'immobilier, les commissariats et les casernes ont atteint un état très avancé délabrement face à ce constat, on ne peut que regretter que les crédits d'investissements prévus demeure en deçà, non seulement de l'ampleur des besoins de rénovation, mais aussi de leur urgence, prenons l'exemple de la gendarmerie, l'investissement qui est prévu, de 100 millions va permettre de rénover 5900 logements qui s'ajoutent aux 13000 mais cet investissement est toutefois en deçà de l'effort nécessaire pour les 76300 logements de la gendarmerie. On ne peut que déplorer à cet égard l'impact dramatique des mesures de régulation budgétaire qui conduit chaque année à reporter d'importants chantiers leur rénovation, je terminerai en évoquant le problème de l'importante dette imposée sur les loyers accumulées par l'agent mais au cours des derniers exercices et qui relève à plus de 100 millions vous-même l'avez dit dans votre ministère trop crédit n'est prévue par le projet de finance pour permettent de résorber cette dette, ce qui contraindra nécessairement la gendarmerie à réduire les autres dépenses de fonctionnement. Enfin, c'est un défi, le budget que vous proposez, Monsieur le Ministre, j'en ai pour 2 minutes

La parole maintenant à Madame Catherine 3 les rapporteur pour avis de la commission des lois pour le programme Sécurité civile Monsieur le président, Monsieur le ministre des sapeurs-pompiers sont décédés dans l'exercice de leur mission en 2016 et 2017 je leur rends hommage et saluer à travers l'engagement, le courage, ainsi que le civisme de l'ensemble des sapeurs pompiers au service de leur population, par ailleurs, Monsieur le Ministre, je suis particulièrement préoccupé par les conclusions d'un récent rapport de l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales qui souligne une augmentation de près de 18 pourcent du nombre de sapeurs-pompiers agressés lors d'interventions en 2016 je tiens donc à condamner avec la plus grande fermeté ces agressions inacceptables les personnels de la Sécurité civile ont connu en 2017 une année d'épreuves et de réformes, il était donc légitime de fonder certains espoirs dans le budget 2018 de la sécurité civile, si certaines attentes ont pas été vaines, je pense à l'augmentation globale des crédits alloués au renouvellement nécessaire d'une partie de la flotte d'aéronefs de la sécurité civile, ainsi qu'à la création de 31 postes de démineurs ce budget comporte néanmoins une déception si grande qu'elle a conduit la commission des lois, sur ma proposition à émettre un avis défavorable à son adoption, il s'agit de la baisse de 60 pourcent de la dotation de soutien aux investissements structurants des indices qui passe de 25 millions d'euros en 2017 à seulement 10 millions en 2018, cette somme de 25 millions d'euros ne constituait pas une nouvelle, Monsieur le Ministre, pour les acteurs de la sécurité civile mais bien simple réguliers âge d'une partie des économies réalisées par l'État, à l'occasion de la réforme de la paix à faire verser aux sapeurs-pompiers volontaires, c'est l'enveloppe versée par l'État au département au titre de la paix à faire qui est ainsi passée de 32 millions d'euros en 2015 à 3,4 millions d'euros en 2017 sur les 25 millions d'euros alloués à la dotation de soutien aux investissements structurants des indices en 2017 20 millions d'euros étaient destinées à financer d'une part des projets locaux, d'intérêt national et, d'autre part des projets nationaux au 1er rang desquels la préfiguration du système au SGA à destination des SDIS dans un contexte de baisse continue des dépenses d'investissement des indices, les conséquences de cette perte sèche injustifiée et préjudiciable sont particulièrement inquiétantes la viabilité du projet SGA SG pourrait tout d'abord, être mis en cause, le ministère de l'Intérieur, m'a répondu que les crédits restons lui demeurerait principalement insectes affectés mais alors c'est l'avenir des différents projets locaux des qui seront directement compromis, telles sont les raisons pour lesquelles la commission des lois a donné un avis défavorable aux crédits alloués au programme de la sécurité civile, mais néanmoins, chers collègues, je voudrais féliciter Monsieur Bazin et lui apporter tout Mossoul tout mon soutien à son amendement qui tente de restituer ces 10 millions d'euros à la sécurité civile et j'ai la faiblesse de croire que le Sénat votera massivement cet amendement, monsieur le Ministre est-ce que l'Assemblée nationale, saura-t-elle faire preuve de la même sagesse que le Sénat. Et tout cela dit, en 3 minutes très précises dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque unité de discussion prend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote, tout est compris, par ailleurs, le gouvernement dispose au total de 20 minutes pour intervenir et je donne tout de suite la parole donc à Monsieur Frédéric Marchand pour le groupe, la République en marche, il y a 6 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre d'État, mes chers collègues, vous savez, il a beaucoup fait référence en cette fin d'année à Georges Clémenceau et je ne résiste pas commencer mon intervention en usant de cette formule chère à celui qui aimait se présenter comme le 1er flic de France, il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut ensuite et enfin l'énergie de le faire, voilà bien le fil conducteur, que l'on retrouve dans la proposition budgétaire qui nous est soumis ce jour, les crédits de la mission sécurité représente 13,3 milliards d'euros, et nous avons pour 2018, un budget qui correspond aux ambitions portées en matière de sécurité qui je le rappelle, est la première des libertés de nos concitoyens, ce budget, il reflète la conscience qu'on, président de la République, l'ensemble du gouvernement, vous Monsieur le Ministre d'État de l'importance des missions exercées par le personnel du ministère de l'Intérieur, en particulier en matière de sécurité et la volonté dans les années qui viennent, d'aller vers une France apaisée, ce sera là tout l'objet de la police de sécurité du quotidien, dont nous attendons beaucoup les crédits de la mission sécurité augmente donc de 1,5 pourcent en 2018, ce qui représente un effort conséquent lorsqu'on connaît les difficultés de l'exercice budgétaire ce budget il est offensif, en effet, par rapport à 2015 on constate que les crédits personnels qui atteignent 710 millions d'euros sont en hausse de 7,3 pourcent plus encore le budget de fonctionnement et d'investissement, des services de 440 millions d'euros, est en hausse de près de 18 pourcent par rapport à 2015 la volonté claire rompant avec des pratiques anciennes de baisse continue des Budgets de sécurité non seulement les efforts faits ces dernières années sont consolidées mais ils sont accentués cette évolution à la hausse est très importante, elle signifie que les moyens supplémentaires exceptionnels obtenus depuis 2015 pour les forces de sécurité dans le cadre de différents plans de court terme sont désormais devenus la norme l'effort du gouvernement dans le domaine de la sécurité marque donc une orientation puissante pour ce quinquennat ce qui était hier exceptionnel est aujourd'hui est désormais inscrit dans la durée, conformément aux engagements du président de la République, le gouvernement procédera donc sur l'ensemble du quinquennat à la création de 10000 emplois de manière à restaurer les capacités de nos forces de sécurité dès 2018 seront recrutés, environ 1000 policiers 500 gendarmes et 400 membres du personnel de la DGSI et du renseignement territorial, cette montée en puissance en matière de personnel sera aussi accompagnée d'un effort important pour l'équipement, ce sont en effet 230 millions d'euros de crédits qui sont consacrés aux de force, police et gendarmerie, c'est-à-dire un niveau équivalent à celui qui a été atteint les 2 dernières années et qui était le fruit de plan exceptionnel ce budget permettra, dès lors, d'investir dans de nouveaux équipements technologiques tablettes smarphones mais aussi caméras piétons qui apparaissent essentiels aujourd'hui pour réussir la réforme de la police de sécurité du quotidien, ils permettront à la fois d'atteindre une efficacité technique supérieure et de procéder à des contrôles dans des conditions plus sereine, enfin, le gouvernement a décidé de faire un effort exceptionnel en matière d'immobilier pour que nos forces de sécurité soient pleinement opérationnel, il faut en effet que leur quotidien s'améliore, nous en sommes toutes et tous conscients, nous allons donc rénover les commissariats, les casernes aujourd'hui parfois très dégradés faute d'entretien régulier suffisant par le passé, c'est une préoccupation très forte des policiers et des gendarmes, et ils ont raison. Pour les 2 forces de sécurité, les Budgets immobiliers sont donc en forte augmentation 196 millions d'euros pour la police nationale, soit une hausse de 5,4 pourcent et 100 millions d'euros pour la gendarmerie nationale, soit une hausse de 9 En outre, les décisions relatives aux petits travaux seront déconcentrés pour rendre les services plus réactif et plus à l'écoute des besoins, c'est bien là du pragmatisme et du bon sens, les crédits de la mission sécurité pour 2018 apporte aux policiers, aux gendarmes des moyens matériels et humains à la hauteur de leur mission et de leur niveau de sollicitation, ce budget est en résonance avec l'arsenal législatif mis en place à travers la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, face auxquelles nous ne baisserons pas la garde, ni dans la volonté, ni dans les moyens alloués ce budget met également en oeuvre les ambitions nouvelles du gouvernement, la lutte contre les inégalités face à la délinquance et aux incivilités qui nourrissent les sentiments d'injustice et d'abandon par la République avec la police de sécurité du quotidien de service de la sécurité publique seront dotés d'outils qui leur permettront de mieux identifier les besoins de sécurité pour à la fois prévenir et réprimer les délits en s'adaptant aux réalités des territoires, la sincérité, mes chers collègues, est aussi la marque de ce budget, contrairement à celui de 2017 qui affiche aussi non soutenable et qui avait entre autres pour conséquence des annulations de crédits en cours d'exercice et des reports de loyer de la gendarmerie nationale, le budget 2018 permettra d'amorcer l'apurement de sa cette dette liée loyer, je l'ai dit, dès 2018 et tout au long de la législature en matière d'effectifs, les 2 forces de sécurité seront dotés de 10000 emplois supplémentaires, conformément aux engagements du président de la République et je me permets de rappeler à mes collègues, que les suppressions d'effectifs, sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012 avaient profondément désorganisé les services particulièrement les forces mobiles et le renseignement intérieur en 2012 un rattrapage timide a été initié puis accélérer à la suite des attentats 2015, grâce à ce budget, les effectifs de la police nationale dépasseront, enfin le niveau de 2007, avec plus de 150000 policiers et ceux de la gendarmerie nationale retrouveront le niveau de 2009 avec plus de 100000 gendarmes et 30000 réservistes ce budget porte un coup d'arrêt à la tendance de paupérisation opérationnelle des forces de sécurité, l'effet sur le quotidien des agents et des services sera rapidement visibles, notamment grâce à l'acquisition de véhicules légers en nombre suffisant, ou encore grâce au crédit pour les petits travaux d'aménagement et d'entretien des commissariats qui augmenteront de 10 millions d'euros et pourront être utilisés directement au plus près des besoins ce budget et la volonté politique qu'il traduit cherchent à créer une relation de qualité entre la population et les forces de sécurité, il permettra de mieux identifier les besoins de sécurité de nos concitoyens au plus près des territoires et de garantir leur sécurité de manière déterminée et efficace la sécurité intérieure, nous le savons, est une grande priorité du quinquennat à ce titre, ce budget traduit un engagement fort pour la sécurité des Français engagements que le groupe la République en marche portent avec conviction et détermination, c'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous appelons à voter ces crédits. Merci. Merci, la parole est à Madame Éliane Assassi pour le groupe républicain communistes, citoyens écologistes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous avez officiellement lancé le mois dernier à La Rochelle, la police du sécu de sécurité du quotidien, l'objectif serait de construire avec les élus de terrain avec la population et avec l'ensemble des acteurs de la sécurité et la prévention des solutions pour répondre plus efficacement aux préoccupations de nos concitoyens, déclarait ainsi le président de la République en octobre dernier en présentant sa principale annonce en matière de stratégie de sécurité, la grande concertation lancée le 28 octobre s'achèvera donc dans 15 jours, et les premières expérimentations débuteront dès janvier 2018 allo monsieur malgré une étude attentive du budget, je n'ai trouvé aucune dotation allouée à ce nouveau dispositif, pas un bureau, autrement dit, cette police de sécurité du quotidien ne s'accompagne d'aucun volet budgétaire et devra donc s'appuyer sur les moyens existants et créer une charge de travail supplémentaire pour les forces de l'ordre sans aucune compensation compensation à moyens constants, c'est également ce que révèle le rapport de monsieur Dominati, vous vous défendez de vouloir remettre en chantier la police de proximité, pour notre part, nous souhaitons véritablement la réhabiliter, vous n'êtes pas sans savoir que nous défendrons en ce sens, notre proposition de loi dans l'ordre du jour réservé à d'autres groupes le 13 décembre prochain mais dans ces déjà pour que votre proposition prennent corps, nous vous proposerons dans le cadre de ce budget par voie d'amendement de réparer entre guillemets, bien évidemment, un oubli en budget de 6 ans, la police de proximité pour que cette police voit réellement le jour, il faut déployer de véritables moyens ce dont elle n'a jamais bénéficié la réalisation d'une police de proximité suppose une gestion des effectifs adapté, d'abord en la dotant des moyens nécessaires, mais aussi en créant, sur le mode de la direction générale de la sécurité intérieure créée le 14 avril 2014 une direction générale de la police de proximité, celle-ci disposerait comme toute entité de cette importance de services administratifs et de soutien nécessaires à son fonctionnement et à sa gestion, je crois qu'il est vraiment temps de s'attaquer une idée de, de, de cesser aux conséquences, sans songer aux causes et de donner la priorité à la prévention et à la dissuasion plutôt qu'à la répression, en outre, les fonctionnaires de police et de gendarmerie souffrent souffrent directement de la dégradation de leurs relations avec la population, leurs conditions de travail se trouve extrêmement détériorées, notamment en raison du renouvellement incessant de l'état d'urgence ces 2 dernières années et du stress permanent qu'engendre des relations trop souvent conflictuelles, or, si le régime d'état d'urgence a pris fin le 1er novembre dernier le gouvernement reconnaît que la menace revêt désormais un caractère durable et a souhaité doter l'État de nouveaux moyens juridiques permanent de droit commun, la loi du 30 octobre 2017 faisant entrer l'état d'urgence dans notre droit commun, poursuit donc cet objectif, le surcroît opérationnel, neveu de devrait donc aucunement se trouvait diminué par la fin de l'état d'urgence et pourrait même s'accentuer à ce sujet, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour saluer la sage décision du de du Conseil constitutionnel qui situe suite à une saisine de la Ligue des droits de l'homme vient de censurer un article de la loi sur l'état d'urgence permettant aux préfets des contrôles d'identité et des fouilles de bagages et des visites de véhicules circulant arrêtées arrêtées ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, comme nous l'avons dénoncé avec les autres membres de mon groupe lors des multiples provocations de l'état d'urgence le Conseil constitutionnel a reconnu que le législateur n'avait pas assurer une conciliation équilibrée entre d'une part, la chose la sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée, garanti par la Constitution. Pour en revenir précisément au budget dans le total des crédits qui doivent augmenter de 1,34 pourcent pour cette mission, nous notons que les recrutements se font au détriment des dépenses d'investissement et de fonctionnement comme le rapporteur spécial de la commission des finances, nous n'avons de cesse de dénoncer l'insuffisance de la formation de nos forces de l'ordre, cela est absolument déraisonnable et dangereuse pour nos concitoyens et pour les fonctionnaires de police et de gendarmerie même je ne peux pas faire ici de parallèle avec les suicides qui qui continuera à s'aggraver, s'agissant des policiers, pas en faire, il fait référence ici dans mon propos quant à l'augmentation continue de l'âge moyen des véhicules, cela devient une constance des insuffisances constatées, mais tout le monde connaît également la situation dramatique de la vétusté de nos commissariats qui en font, à la fois des lieux de travail désagréable mais aussi des lieux peu accueillant pour nos concitoyens et justiciable à l'heure où les victimes sont encouragés à parler à déposer leur plainte, la question des lieux de recueil de la parole des victimes et des formations de ceux qui la reçoivent la retranscrivent doit être prise très au sérieux, je vous le demande solennellement, Monsieur le Ministre finalement nos polices et gendarmeries sont hélas depuis trop longtemps en voie de paupérisation et les Budgets proposés ne sont en aucun cas à la hauteur de l'enjeu et de la crainte que cela représente pour l'avenir de notre pays, le budget préparé pour nos soldats du feu n'est guère plus reluisant et nous suivrons l'avis défavorable de notre collègue Catherine sur le sujet, je vous remercie. La parole est à monsieur Philippe Bohn Carrère pour le groupe Union centriste. Oui, Monsieur le président Monsieur Ministre d'État n'espère collègue en matière de défense, le maître mot est la remontée en puissance, il veut aussi pour la sécurité intérieure, au-delà des missions classiques de sécurité civile ou de lutte contre la délinquance, la lutte contre le terrorisme est une priorité durable de notre société, la mission sécurité du projet de loi de finances améliore les moyens mis à disposition de notre police et notre gendarmerie pour exercer leurs responsabilités. Outre le remplacement de tous les départs à la retraite 1376 emplois de policiers pourront être crées et 450 employes de gendarmerie dans le contexte d'extrême contrainte financière de notre pays, l'effort est substantiel, soyons cohérents avec nous-mêmes, ce budget marque un infléchissement positif à ceux qui estimerait que ce budget est insuffisant, chacun doit mesurer ses critiques au regard des actions du passé et des perspectives budgétaires soumise à nos concitoyens lors de l'élection présidentielle sans brandir, chers collègues, comme vous le faites régulièrement monsieur ministre la courbe d'évolution des effectifs, reconnaissant que les engagements pris par le gouvernement sont tenus en termes de priorité. Il vous a été fait observer Monsieur minus que les créations que j'ai compenser une réduction du temps de travail, nous parlons de quoi, de la directive 2003 sur 88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de la transposition qui en a été faite par 2 instructions ministérielles Honda des 19 septembre 2016 et 4 mai 2017, ainsi que par un décret du 30 janvier 2017, la question de la qualité de vie des agents doit être traitée avec efficacité et humanité, il n'est pas cependant interdit de regarder le choix des nouveaux cycles de travail et notamment celui dit de la vacation forte, lequel aurait des conséquences importantes sur la disponibilité opérationnelle, je souhaiterais également que soit vérifié, les conditions de transposition fin 2016 et 2017 de la directive de 2003 à laquelle je faisais référence il y a quelques secondes et que puisse être en particulier explorer les possibilités d'évolution de cette directive, il est un effet classique que les directives portent exception en matière de défense et pour ma part la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure sont un même sujet pour notre pays, j'entends la critique de mes collègues sur le manque de formation et le manque d'équipement, j'ose espérer Monsieur minus que dans la durée du quinquennat il sera possible d'améliorer les moyens de fonctionnement, les équipements comme je compte également sur les évolutions procédurales de nature à elle ai la charge de travail des enquêteurs, sujet que nous espérons pouvoir être à l'ordre du jour du prochain semestre enfin autorisé, moi, insister sur le respect de la parole de l'État lors de votre audition devant la commission des lois, vous nous avez indiqué qu'à fin 2017, le ministère de l'Intérieur avait accumulé depuis plusieurs emmener des retards de loyer qui s'élève à 114 millions d'euros s'il n'est pas possible de tout rattrapé en une, on est, et si en regard sévère peut-être porté sur l'absence de sincérité des dispositions budgétaires antérieure, je me permets d'insister pour que la parole de l'État soit respectée, même de manière pluriannuelle pluriannuelle avec en perspective les enjeux de meilleure maintenance des commissariats comme des brigades de gendarmerie plusieurs de mes collègues sont intervenus sur ce thème et nous partageons effectivement les enjeux de maintenance au au quotidien des commissariats comme aidez brigades de gendarmerie, vous l'avez compris le groupe centriste partagera son vote l'avis favorable de la commission des finances.

Monsieur le président Monsieur mise état mes chers collègues. La prégnance de la menace terroriste, l'importance de la pression migratoire à laquelle notre pays fait face depuis désormais plus de 2 ans. Et le maintien d'un niveau élevé de la délinquance impliqué au cours des derniers mois, une mobilisation sans précédent des forces de la sécurité intérieure, sur le territoire. Mais gare au niveau élevé et la défense et des menaces des gouvernants, je suis successifs ont engagé au cours des années les efforts budgétaires certains élaborer des plans de lutte contre le terrorisme et contre l'immigration clandestine. Ainsi, les effectifs des forces de police de gens meurent, ils ont été renforcés au cours des exercices budgétaires et un effort de mise à niveau sur l'intérieur été initié, sans toutefois atteindre le niveau exigé par l'aggravation de la situation.

Ces 2 temps budgétaire demeure toutefois bien en deçà des attentes et des besoins des forces de sécurité intérieure. Dans les conditions matérielles, je rappelle quand il ne se dégrader. Contribuant au mal-être généralisé au sein de la pêche national comme de l'agent avait national. Cette mission budgétaire, mes chers collègues, suscite donc de nombreuses interrogations, tout d'abord, en dépit des roches de crédit parfois faibles de baisses significatives apparaissent au sein du programme 176, police nationale et nous semblent difficilement compréhensible, en effet, les crédits d'action ordre public et production de sa souveraineté démis de 59 millions d'euros quant au crédit de l'action sécurité et public sont eux amputé de de 62,6 millions d'euros, ensuite, toujours au sein du programme française alors que la France a des décidé de maintenir les contrôles frontière jusqu'au 30 avril 2018 l'action police étrangers et sécurité des transports internationaux, qui en assure notamment le contrôle des personnes aux frontières, la lutte contre l'immigration clandestine et le démantèlement des filières, qui organisent ne représentent que 8,3 du programme enfin le programme 152 relatifs au crédit de la gendarmerie nationale s'élève, quant à lui à 8,9 milliards d'euros en autorisation d'engagement et à 8 degrés question : de 6 milliards d'euros en crédit en soit soit une quasi-stagnation par rapport aux crédits accordés par la loi de finances initiale pour 2017 en euros constants, ce budget dans l'armée nationale connaîtra donc une baisse de 0 44 pourcent de paiements cette évolution qui pèse sur le budget de fonctionnement et d'investissement et d'autant plus rude le regrettable que la gendarmerie a vu le panel de 6 missions aussi élargir considérablement au cours des dernières années avec un rôle accru. En matière de lutte contre le terrorisme et contre l'immigration irrégulière concernant les 2 programmes 176 et 150 2 police nationale, j'en avais national les formes circonspect petit sur les moyens humains, masque une sous-dotation manifestent en crédits de fonctionnement et d'investissement et ne permettra pas de remédier au vieillissement des parcs automobiles de la police Jean-Marie de permettre la région à la rénovation du parc immobilier qui se trouve dans l'État de la de la délabrement avancé et de poursuivre la mise à niveau des équipements des forces de sécurité, enfin, que dire de l'important : dégradation de la situation matérielle de nos forces de sécurité qui contribue au mal-être croissant au sein de la puce national et la journée nationale aujourd'hui, la colère est légitime, le policier s'ajoute à celles de leurs compagnes, elle doit être entendue, avant de conclure : je vous souhaite rendre hommage à cette tribune aux hommes et aux femmes qui tous les jours, souvent au péril de leur vie, assure notre sécurité, je veux aussi saluer leur engagement au service des citoyens monsieur à mes chers collègues, ce projet de budget de budget n'apporte pas à la police et à l'infirmerie national des moyens financiers matériaux l'humain à la hauteur de leur mission et leur niveau de sollicitation, il ne prend pas également en compte la pleine mesure de la dégradation du contexte sécuritaire dans notre pays groupe, les impôts, les indépendants ne votre aura pas les crédits de la mission sécurité du projet de loi de finances 2018, je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Mesdames et messieurs, Madame et messieurs les rapporteurs spéciaux et pour avis. Mes chers collègues, débattre et voter le budget de la nation, c'est bien plus qu'autorisé les recettes et les dépenses, c'est d'abord assurer le soutien de la France à tout ce qui garantit sa sécurité quotidiennement, s'est donné les moyens concrets, à ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie pour assurer la protection de nos concitoyens, avant d'aborder des considérations d'ordre strictement budgétaires, je veux rendre un hommage solennel aux membres des forces de sécurité blessés ou disparus en services policiers, gendarmes et pompiers sont héros discret mais ils sont indispensables à la vie des Français, je crois utile de le rappeler. Monsieur le Ministre. Nous aurons à coeur d'entendre les réponses aux préoccupations des rapporteurs, le travail qu'ils ont réalisé, mérite d'être salué 2 points retiendront l'attention : le 1er concerne la directive européenne relative au temps de repos car le temps de récupération est indispensable néanmoins l'équation devient très difficile puisque les recrutements sont à peine suffisants pour assurer la rotation. Le 2ème point concerne l'organisation de travail et la répartition des tâches au sein de la gendarmerie, il est temps que la gendarmerie cessent d'effectuer des tâches indues à la place d'autres administrations, la réalité des menaces nous impose de créer les conditions pour qu'elle retrouve des activités au coeur de son métier, son travail d'enquête est très important à l'heure où la société se judiciariser de plus en plus et où l'opinion ne supporte plus les vices de procédure bénéficiant taux criminel à cet instant du débat, je voudrais revenir sur des points spécifiques concernant la gendarmerie qui avait tiennent à coeur, la joint, il a une image largement positive auprès de nos concitoyens alors présents, l'ordre et la proximité auprès des Français pour les sénateurs représentant des territoires que nous sommes, les gendarmes ont un rôle primordial dans le maillage social et territorial, la gendarmerie incarne la souveraineté de notre État et l'unité de notre nation, non seulement les gendarmes contribue à la sécurité de nos citoyens, mais de par leur statut militaire, ils sont les garants de la résilience, alors que notre pays fait face au terrorisme depuis plusieurs années la résilience est une notion des plus précieuses de fait. Ce corps historique de protection de l'État et de la nation, la cible de ceux qui ont la haine de la France, de ceux qui méprisent nos institutions tragiquement la haine de nos forces de l'Ordre s'accompagne de violences inacceptables et intolérables, le sang-froid dont elles font preuve, force le respect et démontrent leur niveau de professionnalisme, il convient de saluer, récemment encore, une brigade territoriale de la gendarmerie a fait l'objet à Meylan, d'un incendie, ses conséquences auraient pu être encore pire même criminel, 5 véhicules ont été détruits, mais l'intention était de tuer des gendarmes, la multiplication de ce genre d'initiative démontre que certains ne vivent pas dans la peur du gendarme médian, celle de la haine, ces différents événements doivent de notre part et de la part de la justice, entraîné un appui sans faille, rappelons la complexité des défis auxquels sont confrontés les gendarmes notamment dans les secteurs relatif à la lutte contre le terrorisme dans ce domaine, je me réjouis de voir le rôle de la gendarmerie renforcés : je veux saluer l'apparition de nouvelles unités qui protégeront certains sites sensibles, en outre, la gendarmerie a en effet une expérience historique comme peut en témoigner le GIGN j'espère que la mutualisation d'ailleurs ne nuira pas à son moral tout ce qui contribue à préserver et améliorer ce savoir-faire, de la gendarmerie doit être encouragé la lutte contre le terrorisme constitue aussi un travail global qui ne se limite pas aux seules interventions ou omission de protection ce combat se tient également en amont dans la surveillance et dans la détection de certains comportements, par ailleurs, il faut souligner le rôle que joue la gendarmerie dans la prévention contre la radicalisation dans ce domaine, l'apport de la gendarmerie est particulièrement précieux en effet par son ancrage territorial historique par sa connaissance du terrain, la gendarmerie jouent un rôle indispensable dans le renseignement de proximité qui est l'échelon de base de notre renseignement par sur l'implantation, la gendarmerie peut détecter les moindres signes de radicalisation c'est un appui précieux dans la lutte contre le radicalisme islamiste antichambre du terrorisme, nos 3611 brigades et chacun de l'eau gendarmes sont autant de postes de d'observation dans ce combat qui doit être mené sans faiblesse, nous devons utiliser au maximum la connaissance du terrain que possède la gendarmerie car cela contribue à une défense efficace de notre ordre public mais la reconnaissance de ce savoir-faire en matière de renseignement territorial réside aussi dans la création de ces antennes de renseignement territorial dont je me réjouis de voir qu'elles sont animées par nos gendarmes Jaïpur et donc tout ce qui va dans la perspective du renforcement de ses capacités de renseignement, représentante de l'État auprès de la population, il faut à ce titre-salué le rôle de la gendarmerie dans les territoires ultramarins c'est actuellement le cas auprès de façon puis pourcent de la population des territoires ultramarins, c'est bien l'unité de la République et de la nation qui est assurément qui est assuré, concrètement, pardon de compatriotes d'Outre-mer le savent et sont en demande de gendarmerie en particulier au moment où le facteur d'insularité rencontrent de plein fouet la mondialisation de trafic et de criminalité dans la protection de leur public et de la sécurité du quotidien, le bilan de l'action de la gendarmerie est positif, on constate ainsi une diminution de violences physiques et de cambriolages ces signes encourageants ne évidemment pas été possible sans son travail. Outre les territoires ultramarins, nous devons impérativement prendre en compte la dimension européenne de la gendarmerie. Sur ce point, on peut regretter parfois le manque de volonté des Européens eux-mêmes aussi Monsieur le Ministre, il serait bienvenu que la France appelle ses partenaires à maintenir, il y a augmenté effort et politique de coopération. Je pense par exemple à certains réseaux et mafia dont le commerce d'armes, de drogue, d'être humain leurs ramifications et implantations sont pleinement européenne, c'est-à-dire sans frontières et libres de leurs mouvements, n'oublions pas que la France par sa géographie est au coeur de trafic à l'Est mais aussi au sud, pour preuve le nombre d'interpellations des go-fast entre l'Espagne et la Belgique, nos concitoyens exigent de l'Europe des frontières sûres et bien gardé, dont la porosité ne peut qu'alimenter le terrorisme et tous les trafics, pour cela, il faut soutenir la gendarmerie dans la lutte contre les filières d'immigration irrégulière 100 gendarmes ont été engagés dans le cadre de Frontex, c'est un début encourageant mais je crois qu'il faut absolument que les dotations suivent la gendarmerie doit être appuyée dans la défense de ses frontières, que l'Europe a trop tardé à protéger. La gendarmerie peut ainsi contribuer à rendre l'Europe plus efficace, plus proche des Français, le mot protection doit pas être un tabou, mais devenir une réalité. Avant de conclure, permettez-moi d'attirer votre attention sur un nouveau terrain de jeu du grand banditisme, le Crime et la commence peuvent être virtuel mais les conséquences et dommages sont bien réels, avec hélas de nouvelles victimes, la question de la cybersécurité est aussi l'un des nouveaux terrains de la gendarmerie s'allonge, vital pour l'ensemble de la société et de ses acteurs tant gouvernementaux qu'économique sur Internet, se livrent une véritable guerre des délinquants. Ils ont des capacités de sans échelle leurs cibles sont aussi bien les particuliers, les multinationales et les institutions gouvernementales, en réalité, la criminalité numérique ne nécessite non pas une politique de défense, mais une politique offensive et cela passe par une politique de recherche d'investissements et de formation de grande ampleur. Contrôle de l'action du gouvernement afin que les crédits de fonctionnement cesse d'être engagée au détriment des crédits d'investissement et soutien permanent aux forces de sécurité sont les 2 valeurs de mon groupe, je vous remercie. Merci Monsieur Charon. La parole est à monsieur Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste et républicain. 5 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voulais partager les propos de Pierre Charon, quand il a rendu hommage. Aux forces de la police de la gendarmerie, de la sécurité civile et à ces hommes et ces femmes qui donne tant. Jour et nuit 365 jours par an, pour notre sécurité. Malheureusement, je ne serai pas d'accord avec lui sur d'autres propos, cela arrive, mon cher collègue, et notamment s'agissant des effectifs parce qu'enfin, Monsieur le Ministre, j'ai remarqué que vous alliez créer 1629 postes de policiers, et 459 postes de gendarmes et à mes collègues R monsieur Karoutchi je sais que ça vous fait de la peine que c'est difficile pour vous, mais je veux quand même rappeler au moment où ils nous donnent des leçons leçons et son rôle de faire mais que, entre 2007, 2012, monsieur le ministre, vous en souvenez bien. Il y a quand même plus de 10000 emplois supprimés, plus de 10000 emplois supprimés dans la police et dans la chambre et c'est une réalité, et aujourd'hui, je sais, c'est terminé, mais enfin

il faut laisser les orateurs intervenir dans le calme. On est tout à fait, donc, mais non, mais je on on est, on est là pour parler, c'est un parlement, mes chers collègues, on a le droit de parler et vous avez le droit de parler alors je rappelle aussi pour mémoire que dans la même période, les crédits d'investissement pour la police, ont baissé de 16 pourcent et ceux de la gendarmerie de 18 pourcent donc on ne peut pas ne pas dire qu'il y a eu depuis un redressement et que d'ailleurs monsieur le ministre, vous êtes dans le droit fil de vos prédécesseurs à cet égard bien et comme mes chers collègues, nous détestons les uns les autres le simplisme après avoir donné acte. le ministre, de ces augmentations d'effectifs, qui doivent être noté, je dirais, comme vous l'avez dit les uns les autres que s'agissant des crédits d'équipement, hé bien, nous ne sommes pas au niveau que nous pourrions espérer pourquoi parce que, alors qu'un effort exceptionnel a été fait dans la loi de finances pour 2017 de 37 millions d'euros. Cette fois-ci, monsieur le Ministre des crédits d'équipement, c'est-à-dire ce qui concerne l'armement, l'habillement, les moyens de protection d'intervention des forces de police et de gendarmerie. Il y a là un vrai problème, comme il y a un vrai problème. Qui risque de se poser et je reprends le rapport de monsieur le roi qui explique que dans la pratique,

qui peuvent donner lieu à des ajustements c'est pourquoi monsieur le ce serait très heureux si vous prenez l'engagement que ces crédits seront complètement sanctuarisé, qu'il n'y aura pas de régulation parce qu'alors qu'ils ne sont pas suffisants, il serait extrêmement dommageable qu'il y avait une régulation pour finir puisque le temps nous est compté, je voulais saluer l'effort pour la sécurité du quotidien tout en reprenant les questions qui ont été posées par Madame Assassi notamment sur le financement, monsieur le ministre, de ce programme et enfin je voulais souligner l'action des actions que vous menez dans la continuité totale avec vos prédécesseurs pour lutter contre le terrorisme qui nous préoccupent tous et notamment je n'assisterai que sur un point : vous savez que quand la DGSI a été mise en place et avant qu'elle fut mise en place, il y avait un grand souci dans la connexion entre le renseignement de terrain et le renseignement au niveau central, je sais que vous vous êtes attaché, vous l'avez dit, à ce qu'il n'y a plus cette distance dans un souci d'efficacité et je salue cela et peut-être pour ne vous nous en parler davantage, parce que c'est nécessaire pour l'efficacité de cette priorité absolue que dans notre pays, la lutte contre le terrorisme, Monsieur le Ministre nous ne suivrons pas nos collègues qui ont décidé de voter contre le budget, nous ne suivrons pas non plus nos homologues de l'Assemblée nationale du groupe homologue de l'Assemblée nationale, nous nous, ça fait tiendront ce qui signifie que nous voyons à la fois le positif des effectifs et les insuffisances, en espérant que cela sera un encouragement pour poursuivre votre action à cet égard, La parole est à monsieur Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE.

en faveur du renforcement des moyens dévolus aux forces de sécurité intérieure qui ont été accompagnés par une augmentation parallèle des crédits de la mission sécurité au sein des forces de la police de la rendant lui ensuite national des programmes de modernisation des initiés par ailleurs

Comores après le président de la République de nom, adresse aux forces de sécurité intérieure du 18 octobre dernier, vous nous avez demandé, monsieur le ministre, que Toulouse à notre ministère sont associés à la redéfinition de notre stratégie de sécurité intérieure, par voie de consultation, c'est une excellente méthode de travail destiné à valoriser le travail d'agent

les risques encourus sont devenus plus aussi grand, il va tente donc concitoyens, c'est pourquoi nous soutenons notre initiative il nécessaire de redonner à vos effectifs tous les hommes âgés qui leur reviennent par leur action en faveur de l'ordre et de la paix civile et la la valorisation des forces de l'ordre et la sécurité publique est également eu conditionné CCR pour le succès des réformes que vous proposez, qu'il s'agisse du renforcement du code du mur de sécurité ou dans le cas de la poésie national de la création de la politique de sécurité du quotidien l'incomparable durant attaque terroriste ne doit pas nous faire oublier les effets de la délinquance des cambriolages et il y a visité quotidiennes sur la propagation du samedi, moins d'insécurité dans l'ensemble de la population sur les 3800 postes créés dans la police nationale 12 femmes ont été affectés à la DGSI et aux services de renseignement territorial, cependant, le développement des moyens techniques et humains doivent servir enseignements et de lutte contre le terrorisme, non pas compromettre la mise en oeuvre d'autres réformes aujourd'hui à l'expérimentation, je pense notamment à l'accès à l'intention des caméras piétons et au sein de la grande Amaury au développement des brigades territoriales de contact, il faut remettre le gendarme au plus près de la population, c'est comme ça que vous avez l'information qu'il y aura également également des outils numériques Néo-Zed qui devrait faciliter les agences terrain toutes ses applications utiles dans les démarches quotidiennes des forces de l'Ordre devrait être maintenus à propos de la maman ils national il est par ailleurs de savoir que l'évolution des crédits de son programme, monsieur, pas le profil que celui de la police nationale est arbitrages intervient alors même cru attendent sécuritaire ont grandi sur l'ensemble du territoire, pas simplement dans les zones protégées par la police nationale dans nombre de communes

l'Association des élus à la définition des stratégies locales sécurité afin de maintenir l'expression de notre vie culturelle et associative c'est ma vision de ce que pourrait être le code d'union territoriale de sécurité et il semble que sur ce point-là, nous visions pourraient converger, Monsieur le Ministre, sans remettre en cause la politique menée à ce domaine je voudrais également vous faire quelques remarques sur les moyens affectés à la lutte, le contre le terrorisme, près de 3 ans après, du déclenchement de l'opération samedi Neil et plusieurs décennies sous le régime Vigipirate il faudrait il faut à présent celle sur l'efficacité de telles opérations préventives mobilisant par ailleurs le moment important d'effectifs mais dernière observation. Concernant la sécurité routière alors moins des crédits et justifiée par l'augmentation du nombre de personnes accidentées et du ralentissement de la baisse de nombre de personnes tuées depuis les années 60 le nombre de personnes tuées dans les accidents de la route a baissé sensiblement, passant pas ça, ne plus le 16ème et le parrain à un peu moins 16 hommes parce qu'on ne puisse cette année mais la cible fixée à 2000 morts par an n'est toujours pas atteinte et parmi ces victimes, beaucoup sont des cyclistes et des piétons en conclusion sur les terminer par un petit billet d'humeur, j'ai pris connaissance. D'une éventuelle proposition de réduire la vitesse autorisée sur les routes à 80 kilomètres à l'heure.

et la voiture reste le seul moyen de se déplacer sur coup au coeur des territoires enclavés de forts l'oblige urbaine que je respecte, pousse à cette mesure, mais il a toujours préféré la prévention à la répression,

La parole est à monsieur Marc Laménie pour le groupe, les républicains. Pour 5 minutes. merci. messieurs les présidents des commissions, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, je voudrais saluer le travail de nos reporteurs partager avec l'ensemble des personnels de notre institution. Et il est vrai que depuis que j'interviens modestement depuis 2007 sur cette mission sécurité j'ai pu mesurer son importance et son évolution de plus en plus complexes, certes les sécurités constitue un gouvernement après gouvernement une priorité, la sécurité des personnes et des biens, cela été beaucoup rappelées porno collègue est en effet l'affaire de tous, c'est pourquoi je tiens à rendre hommage à l'ensemble des personnels qui travaillent avec professionnalisme, gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers on associant également nos militaires dans le cadre des opérations sentinelle dans le cas de la lutte contre le terrorisme, ainsi que celles et ceux qui oeuvrent au sein de 3 fonctions publiques, les dangers sont présents partout en secteur urbain comme on secteur rural, d'où l'importance aussi pour notre secteur rural des brigades de gendarmerie de proximité qu'il convient aussi de soutenir, élu d'un département frontalier les Ardennes je peux remarquer et mesurer le surcroît d'activités opérationnelles liées aux contrôles aux frontières, dans le cadre de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la loi de finances pour 2018, les crédits de peu manque progresse très légèrement, c'était, rappelez plus un virgule 34 pourcent pour atteindre 19,2 milliards d'euros répartis comme suit des yeux 5 milliards d'euros pour le programme, police nationale et 8,6 milliards d'euros pour le programme, gendarmerie nationale. Les moyens financiers sont ceux qu'ils sont sur l'été rappelé mais je tiens surtout à mettre en valeur les moyens humains, même si une progression des effectifs et temps. L'émission de nos policiers, gendarmes, sont de plus en plus éprouvantes métier très difficile, dangereuse, nous, nous, on nous en prenons conscience très régulièrement, notamment lors des cérémonies annuelles, dommage pour les gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers décédés en service, c'est pourquoi le respect et la reconnaissance, l'écoute et le dialogue doivent être également des priorités en direction de l'ensemble des personnels, à ce titre également la tâche reste immense, je prendrai un instant pour relater de témoignages, mais que aussi l'ensemble de nos collègues dans nos département respectif dans le cas de notre mission de parlementaire. Il y a quelques jours, j'ai participé à Charleville-Mézières où 73ème anniversaire des compagnies républicaines de sécurité puisqu'on en compagnie CRS 23 et j'ai pu réellement et sincèrement mesurer le rôle important de ces compagnies, dont les missions sont malheureusement souvent méconnu. Autre modeste témoignage j'ai participé plusieurs de nos collègues, on avait parlé à une réunion organisée par Monsieur le préfet des Ardennes, monsieur le procureur de la République, dans le cas de la mise en place de la peu police de sécurité au quotidien, c'est vrai que cette réunion fort intéressante, mais qui mobilise aussi beaucoup de partenaires mais il faut espérer aussi que les moyens soient à la hauteur des objectifs en terme d'efficacité, il convient de soutenir le dialogue, la concertation s'était rappelé s'était rappelé avec les élus locaux, les policiers municipaux, le secteur la sécurité privée également mais aussi les acteurs économiques et en particulier aussi, naturellement, l'éducation nationale, les travailleurs sociaux, protéger nos concitoyens partout : tels sont les objectifs lutter contre l'insécurité routière, là aussi, même s'il a des choses à fait qu'il en reste aussi beaucoup à faire, je dirais aussi également la lutte également les violences conjugales, le harcèlement fait malheureusement des sujets d'actualité, et je le dis également en liaison avec les collègues qui font partie de la délégation du droit des femmes présidée par notre collègue Annie que Guillon et je crois que là, là aussi il y a, il reste beaucoup à faire et je crois que c'est la mobilisation de toutes et tous et pour conclure, j'aimerais, nous, nous nous devons de renforts ont forcé cette mobilisation pour la sécurité, donc je suivrai bien entendu la vie de notre commission des finances puis je dirais vive les policiers vivent les sapeurs-pompiers de vive les gendarmes jour merci. La parole est à monsieur Jean-Luc Fichet pour le groupe socialiste, pour 5 minutes. Monsieur le président, monsieur ministre, mes chers collègues, mon intervention s'intéressera spécifiquement aux crédits alloués à la sécurité civile au sein de la mission sécurité. Nous le savons, les intervenants dans le domaine de la sécurité civile sont nombreuses : outre l'action essentielle des sapeurs-pompiers et en particulier des sapeurs-pompiers volontaires sur laquelle je reviendrai plus particulièrement on y compte également les services de déminage des formations militaires ou encore des actions, les aspirations et les actions citoyennes l'ensemble de leurs actions s'inscrivent dans un contexte composé de défi d'ampleur à relever, on pense aux traditionnelles mais spectaculaires feux de forêt, survenu ce début 2 dernières années, mais également aux attaques et aux menaces terroristes auxquels notre pays doit faire face, ainsi qu'aux catastrophes naturelles telles que celles qui ont tout récemment ravagé les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, ainsi que les départements de Martinique et de Guadeloupe, rappelons en outre que si la politique publique de sécurité civile et défini à l'échelon national et conduite par le ministère de l'Intérieur en vue d'assurer la protection des populations et la gestion des crises, elle était également largement financé et appliqué au niveau local les collectivités territoriales ainsi près de 5 milliards d'euros par an aux actions, émission de sécurité civile au sein du budget de l'État, il ne faut par ailleurs veiller à ce que la sécurité civile ne soit pas le parent pauvre des moyens globaux accordés à la sécurité. en examinant à première vue les chiffres contenus dans le projet de budget du gouvernement pour 2018 on pourrait spontanément, je veux dire que ce n'est pas le coeur. Les moyens de ce programme, passant de 469 virgule 109 millions d'euros à 855,39 millions d'euros en autorisation d'engagement sont 14 millions d'euros à 533 millions d'euros en crédit de paiement. Mais cela a été dit, cette hausse de près de 400 millions d'euros s'explique par la commande par l'État en 2018, 2 6 appareil multirôle dont la livraison s'échelonnera entre 2000 19 et 2022 afin de renouveler la flotte d'avions bombardiers d'eau du fait de l'usure des matériels en fonction depuis de très nombreuses années. Surtout, cette hausse de crédits dissimule un Net recul de soutien aux acteurs de la sécurité civile, notamment une diminution de 60 pourcent de la dotation de soutien aux investissements structurants DC10 alors que doit s'amorcer la mise en oeuvre du système unifié de gestion des alertes et des opérations des services. Cette dotation de soutien créé par la loi du 27 décembre 2016 relatives aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires et qui s'élèverait en 2017 à 25 millions d'euros ne sera plus que de 10 millions d'euros on dit cela est d'autant plus préoccupant que parmi les acteurs agissant en matière de sécurité civile et relevant de la sphère publique et 10 et les sapeurs-pompiers occupe une place particulière qu'il convient de préserver notre pays comptait 97 services départementaux d'incendie et de secours et les statistiques témoignent de leur activité soutenue, plus de 4 millions et demi d'interventions en 2016, 122 interventions par jour et, dans certains virus jusqu'à 254 interventions par jour, en outre, je voudrais insister sur l'importance de poursuivre l'action initiée sous la précédente mandature, en matière de valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers qui est au coeur du dispositif de protection de la population au quotidien à cet égard nous nous félicitons Monsieur le Ministre, que vous il y a annoncé hier le lancement d'une mission gouvernementale destinée à augmenter le nombre de sapeurs-pompiers volontaires, cela est nécessaire car les difficultés à pouvoir concilier ce statut et sa vie professionnelle et familiale sont nombreuses, même s'il faut rappeler que sous la présidence de François Hollande, nous sommes parvenus à enrayer la crise du volontariat qui a affecté les effectifs après être passé de 200000 en 2007 à 192000 en 2013 le nombre de sapeurs-pompiers volontaires est enfin reparti à la hausse à partir de 2014, on dénombrait ainsi 193800 sapeurs-pompiers volontaires au 31 décembre 2016. Les sapeurs-pompiers reçoivent une formation professionnelle une formation à la hauteur de ce des professionnels et donc il est nécessaire qu'ils aient les mêmes équipements voilà donc ce que je peux vous dire, pour l'essentiel, c'est que, malgré les effets d'apparence crédit accordé pour 2018 ne sont pas au rendez-vous et c'est pourquoi, avec mes collègues du groupe socialiste et républicain, nous nous abstiendrons sur ce programme budgétaire, nous avons versé. Merci monsieur et maintenant la parole est à monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur pour une durée de 20 minutes. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs spéciaux, Madame et messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames et messieurs les sénateurs, tout d'abord, permettez-moi de m'associer aux propos qui ont été ceux de Monsieur Sharon de monsieur sueur pour rendre hommage. Alain aux forces de l'ordre de sécurité publique de protection civile. J'avais eu le occasion de les connaître, dans des fonctions précédentes et aujourd'hui je les bois agir comme ministre de l'Intérieur. Et je veux dire que je suis extrêmement fier de l'action qu'ils peuvent mener les uns et les autres sur le terrain. Je suis allé voir comment nos policiers pouvaient travailler dans un certain nombre de quartiers difficiles, je suis allé dans un certain nombre de communes de la périphérie avec la BAC et j'ai pu voir combien était difficile, c'est missions, je suis allé voir des gendarmeries dans des zones rurales j'ai pu voir combien était grand le contact avec la population combien était grande aussi leur technicité, j'ai eu à gérer avec les forces de la protection civile, à la fois l'épisode des feux de forêt est plus important que nous ayons connue depuis 14 ans, et en même temps, les ouragans que nous avons connu dans les Antilles, j'ai pu voir l'engagement des uns et des autres, ils sont absolument formidables et je voudrais aujourd'hui leur dire merci souhaite polémiquer polémiquer avec personne, parce que chacun a ses difficultés et toutes les périodes peuvent connaître leurs problèmes. Je me tiens simplement aux chiffres et je pense que c'est sur ces chiffres, que la commission des finances, débattu et c'est pour cela qu'elle a rendu un avis favorable permettrait de lire l'avis de la commission des finances, en conclusion de mon intervention si on regarde et je le montre toujours quelques-uns d'entre vous y ont fait allusion le petit tableau qui montre l'évolution en base 100 depuis 2007, on s'aperçoit que sur les effectifs, nous avions connu une chute extrêmement importante jusqu'en 2012 et qu'ensuite ils sont remontés, on s'aperçoit que dans le même temps, nous avions connu sur les dépenses d'équipement une chute relativement progressive qui elle a duré jusqu'en 2015 et c'est à partir de 2015, que les chiffres ont remonté l'engagement que j'avais pris lorsque je suis arrivée au ministère de l'Intérieur était selon les engagements du président de la République de donner la priorité à la sécurité et c'est avec cette priorité que je suis venu devant vous présenter la loi si tôt, je sais ce qu'à l'époque, on a dit politique trop sécuritaire qui pouvait tuer les libertés, je suis allé la semaine dernière sur le marché de Noël de Strasbourg et j'ai vu que c'était peut-être grâce à cette loi que nous avions prises que nous pouvions organiser de belles manifestations où je sentais celles et ceux qui étaient présents sur le terrain, pouvoir jouir d'une liberté qu'il n'aurait pas eu si nous n'avions pas adopter cette toi alors les crédits que je vous présente aujourd'hui sont des crédits en augmentation de 1,5 pourcent en 2018 par rapport à 2017 on peut dire, ce n'est pas beaucoup, sauf que comme vous le savez, nous avons aujourd'hui 2200 milliards de dettes, une charge de la dette de 42 milliards par an, soit les Budgets cumulés de l'enseignement supérieur et de la recherche de la justice, du sport et de la culture avec demain, si les taux d'intérêt remontent de grandes difficultés pour le budget français, c'est pour cela que le gouvernement a décidé de réduire le déficit de 7 milliards d'euros et dans cette période où nous réduisions la dépense publique, parce que c'est absolument nécessaire, les crédits de la sécurité continue à augmenter, évidemment, c'est sur cela

donc s'ils augmentent de 1,5 pourcent et le 1,9 pourcent hors personnel, ça veut dire que les dépenses de fonctionnement et d'équipement, prise globalement sont évidemment plus importante encore que l'augmentation en personnel, comme vous le savez, les crédits de personnel sont en hausse de 7,3 pourcent si vous regardez globalement, le budget de fonctionnement et d'investissement, il est lui en hausse de près de 18 pourcent par rapport par exemple à 2015 eu 2 années exceptionnelles après évidemment les attentats. Et donc nous continuons sur cette ligne a parce que nous voulons faire de la sécurité une de nos priorités, le message est donc clair : non seulement nous consolidons les efforts passés mais nous Les Jacques sont tous mesdames et messieurs, que voulons-nous faire, nous voulons effectivement créé un certain nombre de postes 10000 créations d'emplois, de manière à restaurer les capacités des forces de sécurité en 2018, nous procéderons donc à ce titre-au recrutement d'environ 1000 policiers 500 gendarmes, 400 personnels de la DGSI et du renseignement territorial en 2000 19 et 2020, ce sera au total 2500 chaque année les 1500 2021 et en 2022, on peut toujours dire que ce n'est pas assez, mais c'est quand même vous l'avouerez, un effort conséquent mesdames et messieurs, on pourrait se dire, et quelques-uns d'entre vous l'ont dit, mais est-ce que par exemple ses créations, le personnel ne seront pas totalement prise par la vacation for je peux vous dire que nous avons décidé, parce que nous voyons bien quel est le problème : un moratoire pendant un an pour que, effectivement, l'ensemble des créations de postes ne soit pas totalement pris par la vacation forte là où il est possible d'avoir des cycles, ils ne font pas que progressivement nous ayons moins de monde sur le terrain après avoir créé des postes, nous ferons la vacation dans le cas contraire, nous ne la ferons pas en même temps, nous procédons à ce que vous dites, c'est-à-dire que les réformes de structures sont les réformes particulièrement important pour la sécurité et nous allons faire une grande réforme de la procédure pénale, les uns les autres vous connaissez les policiers et les gendarmes, que disent-ils aujourd'hui, ils disent la moitié de notre temps et pris par les tâches administratives, pour la première fois en même temps que nous ferons la police de sécurité du quotidien, nous pourrons l'affaire parce que nous allons avec madame la ministre de la justice, faire une réforme de la procédure pénale qui libérera nos policiers et nos gendarmes d'un certain nombre de tâches administratives, oui, moi j'ai entendu les policiers, les gendarmes je sais ce qu'aujourd'hui sont les tâches indues, je serai effectivement comment ils sont pris par des procédures qu'à la fois, policiers, gendarmes, déplore mais qu'en même temps, magistrats, déplore et pour la première fois, nous avons organisé à Amiens, une réunion conjointe à la fois de policiers, de gendarmes et de magistrats, de manière à pouvoir travailler ensemble sur la numérisation sur l'an Lisa Sion des procédures de manière à pouvoir libérer les uns et les autres et pouvoir créer une sécurité et une justice qui soit, celle du 21ème siècle, mesdames et messieurs, on peut dire que le budget sécurité que nous vous présentons les propositions que nous faisons ne sont pas satisfaisantes, mais il se trouve que nous avons lancé une grande consultation sur la police de sécurité du quotidien et mesdames et messieurs les sénateurs, allez voir les maires et vous verrez, vous verrez qu'ils réagissent de manière extrêmement positive à cette enquête que nous avons lancé et ils en attendent beaucoup, parce qu'ils veulent qu'aujourd'hui effectivement nous retrouvions un certain nombre de forces de l'ordre sur le terrain, alors, cette police de sécurité du quotidien que sera-t-elle d'abord, ce sera un continuum de sécurité et nous avons voulu consulter à la fois, évidemment, les forces de sécurité nationale, policiers et gendarmes, mais nous avons consulté les élus locaux, les élus locaux, avec leur police municipale parce qu'il nous semble qu'il y a effectivement des relations à pouvoir créer entre nous avons travaillé aussi avec les agences de sécurité privées, de manière à voir comment on peut pouvait renforcer leur professionnalisme et donc nous allons dans cette ligne, crée un vrai continuum une vraie chaîne de sécurité qui nous permettra, effectivement, dans les prochaines années, de mieux assurer la sécurité de nos concitoyens, vous avez parlé les uns et les autres, des conditions de travail de nos policiers, de nos gendarmes, je l'ai vu comme je regardais un certain nombre de commissariats de casernes de gendarmerie, j'ai vu dans quel état elle pouvait être, et donc nous avons décidé de faire un effort conséquent certes j'ai remarqué, il y avait une dette qui était de 114 millions d'euros pour les loyers qui n'étaient pas payées par la gendarmerie, mais nous avons commencé dès 2017 a commencé à payer cette dette et donc ces 13 millions par an, ils serviront à payer cette dette, ce qui ne nous empêche pas de consacrer des sommes extrêmement important pour pouvoir rénover, à la fois les postes de police et les gendarmeries dans la police, le budget immobilier de constructions et travaux lourds atteindra 196 millions d'euros, soit une hausse de 5,4 pourcent des opérations importantes seront lancés en 2018 et nous avons voulu que nous puissions déconcentrer un certain nombre de crédits, ce sera à 50 millions d'euros déconcentré, cette année, contre 19 millions d'euros l'an dernier dans la gendarmerie, de même, le plan d'urgence logement sera non seulement son clé mais aussi augmenter et les crédits de réhabilitation du parc domanial atteindront 100 millions d'euros en 2018 dans ces 2 forces, j'ai souhaité, là aussi pour la gendarmerie, il y a une déconcentration des décisions de manière à ce que, au niveau local, on puisse décider de ce qui va bien pour la mettre un coup de peinture la réparer telle ou telle chose plutôt que les décisions soient prises d'en haut, la déconcentration est quelque chose de nécessaire et qui sera efficace sur le terrain, enfin, le gouvernement, comme vous le savez, a souhaité prolonger le régime juridique qui permet aux collectivités locales d'être maître d'ouvrage, voire cofinanceurs de travaux intéressant la sécurité intérieure cela répond en effet à un souhait de nombreuses collectivités pour ce qui concerne l'équipement, j'ai entendu parler tout à l'heure, nous avons là aussi consolider les moyens de forces de sécurité, avec 230 millions de d'euros de crédits dans les 2 forces, c'est-à-dire un niveau équivalent à celui atteint ces 2 dernières années années mais à l'époque il s'agissait de plan qui avait été présenté comme exceptionnel parce qu'il correspondait à la période de l'attentat cela se traduira par renouvellement du parc automobile, l'objectif est de tendre vers 3000 acquisitions annuelles pour ne pas dégrader comme vous l'avez mentionné l'âge moyen de la flotte, pour le et de force le budget prévisionnel est de 136 millions d'euros, enfin vous le savez, nous pensons qu'il faut un saut technologique et c'est pour cela que dans la gendarmerie nationale, le projet Neo jambes sera achevé à la fin de cette année 2017 avec 67000 tablettes et smartphones qui ont déjà été déployés dans la police, à la fin de l'année 28500 terminaux néo- Paul seront effectivement en service et j'ai demandé que 22000 tablettes et smartphones supplémentaires soient déployés d'ici 3 ans, mesdames et messieurs, quand on dit il n'y a pas d'équipement, il y a pas d'investissement, il se trouve que ce matin j'étais devant le comité scientifique de la gendarmerie, là où ils essayent de réfléchir sur l'innovation, moi j'invite celles et ceux qui veulent aller voir à Pontoise ce que développe aujourd'hui notre gendarmerie en coopération avec notre police et vous verrez que nous sommes sans doute l'une des forces de sécurité européenne qui consacre le plus à l'avenir, pour essayer de penser ce que sera la délinquance, la criminalité de demain et vous verrez comment il travaille sur la cybersécurité comment ils prennent en compte les défis un nouveau alors je suis extrêmement heureuse d'être à la tête de ce ministère parce que, oui, c'est un ministère d'innovation c'est un ministère aux forces de sécurité, nos forces de protection civile sont sans cesse dans la construction du futur des équipements, je signale que pour la gendarmerie nous achèterons l'an prochain 20000 gilets pare-balles individuelles que pour les munitions parce que vous en avez parlé nous augmenteront de 2 millions d'euros que pour la police, ce sera 30000 gilets pare-balles que ce sera 12 millions d'euros de plus pour les munitions qui dit que l'équipement n'est pas à la hauteur pour parler du budget de la protection civile, je dirais que Madame prenez serait plus compatissante à notre égard, lorsque évidemment on achète 6 avions supplémentaires que l'on commande, cela me semble un investissement qui est relativement conséquent, même si évidemment il s'engage sur plusieurs années pour ce qui concerne le programme SGA SG au dont vous avez parlé les 10 millions d'euros seront engagés cette année pour pouvoir commencer à développer ce programme qui ensuite permettra os 10 de faire des économies considérables sur le long terme, ce sont 600 millions d'euros de d'investissement au moins ils auront à consacrer, que, par rapport au hausse 10 le gouvernement ne fait pas des efforts pour essayer de penser à leur avenir, voilà, Mesdames et messieurs, en contrepartie de ce que nous faisons, nous engagerons un certain nombre de réformes structurelles, parce que aujourd'hui il convient de le faire penser mieux les actions de mutualisation entre la police et la gendarmerie, faire que dans nos services informatiques, on n'est plus de compatibilité la réforme dont je parlais de la procédure pénale suppose qu'évidemment l'informatique de la police de la gendarmerie, de la justice soit compatible et sur ces points-là, il faudra faire des efforts tout à fait considérable oui c'est par l'innovation que nous transformerons l'appareil d'État, en matière de sécurité et de justice, mesdames et messieurs, il faudra aussi sans doute réfléchir à la façon dont nous pouvons faire en sorte que la police scientifique de la police, celle de la gendarmerie puissent mieux travailler ensemble, mieux porter leur innovation, alors cela nous allons le faire parce que nous pensons effectivement que nous le devons à nos concitoyens, mesdames et messieurs, moi je suis extrêmement heureuse de vous présenter aujourd'hui ce budget il est une réponse à l'engagement qu'avait pris de la République, de faire de la sécurité sa priorité absolue et c'est sans doute pour cela, monsieur le rapporteur de la commission des finances que je cite réunis à nouveau le jeudi 23 novembre 2017 sous la présidence de Monsieur Vincent et blé, président de la commission après avoir pris acte des modifications adoptées par Assemblée nationale, la commission des finances, a confirmé sa décision de proposer au Sénat d'adopter les crédits de la mission et ceux du compte spécial, telle que modifiée par ces amendements, elle lui a proposé de quitter sans modification des articles 62 terre 62 quater et 67 et d'adopter la additionnel après l'article 67, mesdames et messieurs, je vous demande, parce que je connais l'objectivité du Sénat de vous fiez au Chili et au réel et non pas simplement à une subjectivité qui pourrait apparaître comme seulement politiciennes merci. nous allons procéder à l'examen des amendements maintenant portant sur les crédits de la mission sécurité figurant à l'État B.. à l'article 29. A un amendement présenté par monsieur Philippe Dominati au nom de la commission des finances. Vous le présenter. Oui, monsieur le président, Monsieur le ministre, je crois que dans cet hémicycle, tout le monde partage votre enthousiasme sur la mission des des forces de l'ordre, par contre en ce qui concerne l'interprétation des chiffres effectivement, nous pouvons avoir une vision différente parce que vous disiez : qui peut contester le fait que les équipements ne soit pas au rendez-vous, bah elle vote rapporteur spécial, le rapporteur de la commission des finances, a présenté à la commission des finances, le fait qu'il y a une dizaine d'années à effectif égal, comme le soulignait d'ailleurs monsieur Sueur monsieur Sueur l'a dit tout à l'heure, effectivement, nous allons dans le budget 2018 retrouvé à peu près les effectifs de l'année 2008, sauf qu'en 2008, il y avait 33000 véhicules de police, et 5000 véhicules annuellement. Tandis que cette année on est en dessous de 3000 j'ai signalé tout à l'heure, selon vos chiffres, le vieillissement du parc automobile, le fait que des incidents ont eu lieu dans la formation des personnels, le sous-équipement qu'il y avait et il y a une grande dit Ferrand Centre ce budget, comme vous l'avez souligné qu'est le budget d'une nouvelle mandature d'un nouvel exécutif avec un engagement réaffirmé avec le budget de l'année précédente où finalement le président de la République avait dû faire face au milieu de son mandat à des attaques liées au terrorisme et avait dû décliner un certain nombre de moyens par des plans d'exception et vous-même, vous l'avez souligné, or cette année, malheureusement, nous retrouvons les mêmes ratios, c'est-à-dire que, à chaque fois qu'il y a des créations de postes et moi, je ne voudrais pas revenir sur les polémiques comme des 2 derniers quinquennats, c'est-à-dire qu'il a effectivement à cause de la crise du terrorisme à cause de la crise migratoire, cause de la crise migratoire, il a fallu renforcer nos forces de sécurité, pour autant, nous ce que nous voulons, c'est leur donner des moyens or tendance prise par le gouvernement consiste à faire que lorsqu'il y a création de postes, c'est au détriment des moyens et ce budget malheureusement et dans la continuité de celui de l'an dernier et le ratio frais de personnel par rapport aux investissements et au fonctionnement et malheureusement le même, il n'y a pas de rétablissement vous citez les chiffres de l'investissement, vous êtes obligé de faire référence au budget de 2015, parce qu'effectivement on ne peut pas faire référence au budget de l'année précédente, alors, tant que ce ratio sera aussi déséquilibré, nous aurons des crises dans nos forces de l'ordre, l'ancien président de la République avait dû réunir en urgence, syndicats et et les différents représentants des forces de l'ordre, un plan d'urgence de 200 millions avaient été infectés, finalement, il y en avait que 35 c'est l'objet de cet amendement et vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, c'est sous réserve de l'acceptation de cet amendement, que la commission des finances anémie favorable si cet amendement n'est pas accepté une parure hurlement, la commission des finances en prendre acte. Merci l'avis du gouvernement, monsieur le Ministre. Oui, l'amendement de monsieur Dominati vise donc à augmenter pour la police nationale de 40000 millions les crédits finançant les dépenses d'équipement et les dépenses immobilières et donc en disant que cet abonnement sera financée par une baisse des crédits du thé 2 salaires des dépenses de personnel alors il nous dit financé par l'abandon des tâches indues, monsieur Dominati, nous allons le faire les tâches indues, mais ça va nous prendre un peu de temps, voyez le temps que vous adoptez la peau, la réforme de la procédure pénale, que nous examinerons ensemble et je ne vous demandera à l'aller à cette époque-là, beaucoup de bienveillance au Sénat pour nous aider à pouvoir. Aller de l'avant, mais vous comprenez bien que je ne peux pas réduire aujourd'hui les dépenses de personnel et baisser les effectifs au moment où des centaines de maires des milliers de mères dans leur pays, me demande au contraire de les augmenter.

comme le rappelait le ministre tout à l'heure tout de suite la proposition de cet amendement consiste à diminuer en quelque sorte le parcours professionnel et carrières, les rémunérations, les mesures catégorielles salariale du du personnel de, de, de la gendarmerie, en particulier je je comprends pas comment on peut argumenter ceci, d'augmenter les investissements et matériel dont dispose l'ensemble de nos forces de de l'ordre, en sus, gérant de diminuer par exemple rémunération. J'avoue que je n'ai pas bien comprendre, c'est comme si vous vouliez repas, l'ensemble des bureaux de poste et pour financer cela en termes d'investissements ou diminuer la rémunération des postiers,

La parole est à monsieur Philippe Bas. Président, je dois dire que j'interprète cet amendement comme un amendement d'appel, il est destiné à souligner une incohérence dans le projet de budget qui nous est présentée, car les moyens en matériel et en équipements, en véhicules ne sont pas en rapport avec les moyens humains qui sont annoncées dans ce budget, monsieur le ministre, vous nous recommandez d'être objectif et de regarder les chiffres, hé bien les chiffres nous disent que votre budget augmente approximativement du montant de l'inflation, vous nous demandez de vous faire crédit, d'une certaine façon, en alléguant le bénéfice pour l'instant virtuelle d'une réforme de la procédure pénale, quant à la directive de 2003, dont chacun sait qu'elle va absorber des moyens en personnel, vous nous dites que vous avez unilatéralement décidées à moratoire et que, si vous estimez qu'elle n'est pas applicable, vous ne l'appliquerait pas j'aimerais bien savoir comment vous ferais pour que l'État français ne soit pas condamné sous astreinte à appliquer les engagements européens qu'il a pris, qui sont d'ailleurs des engagements qu'on applique dans tous les autres domaines, les directives européennes doivent être appliquées quand on examine la question du logement, des gendarmes, des moyens de raccompagnement des étrangers en situation irrégulière, quand on examine la situation de la police de l'air et et des frontières quand on him examine les investissements de la sécurité civile, or le renouvellement nécessaire est prévu depuis longtemps de la flotte des avions quand on examine les dépenses supplémentaires que la police de sécurité au quotidien, elle risque de prélever sur les moyens de la sécurité, on se dit qu'il n'y a décidément pas d'autre choix que de rejeter vos crédits comme étant insuffisant pour mettre en oeuvre la politique de sécurité, que le président de la République a voulu. Oui, simplement, effectivement, le président de la commission des lois a très bien répondu à l'interprétation à l'interprétation caricaturale qui va être donner à ce à cet amendement effectivement actuellement la police nationale, comme la gendarmerie nationale, manque de moyens humains, mais elle manque aussi de moyens matériels informatiques immobilier par rapport aux effectifs dont elle dispose déjà aujourd'hui, c'est sur ce point que nous voulions attirer l'attention du gouvernement l'équipement informatique laisse toujours à désirer, les véhicules sont obsolètes, les locaux sont insalubres, combien Monsieur ministre, avez-vous déjà équipés de policiers par rapport d'éveiller l'existant de caméras individuelles que tout le monde juge absolument indispensable même pour assainir les rapports entre la police et la population, et même souvent entre le la de la police et la justice, cet équipement est absolument prioritaire et l'effort budgétaire qui nous est proposé n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. La parole est à monsieur Marchand. Oui, monsieur le président, Monsieur le ministre, j'ai entendu parler sur ces bandes un appel, je pense que le seul appel qui vaille aujourd'hui en cette fin d'année 2017 et celui qui a lancé par nos concitoyens et par les élus locaux en matière de sécurité à savoir donner à nos services de police, les moyens humains de renforcer le lien Direct avec nos concitoyens par une proximité qui est garanti, il n'y a pas une seule minute où les uns et les autres dans les contacts que nous puissions avoir avec les élus locaux avec nos concitoyens, pour voir que la demande d'effectifs est prégnante, elle est réelle et que par conséquent donc il importe de faire en sorte que les effectifs puisse augmenter pour que nos concitoyens puissent voir encore et toujours davantage de services de police, voilà pourquoi donc nous voterons contre cet amendement. Bien la parole monsieur le ministre, demande la parole : non à la fin de toute la série d'amendements très bien. Non, non, c'est là, on va voter Monsieur ministre donc Alesi. Oui, je veux redire redonner les chiffres. En disant que. à la fin de l'année prochaine. L'ensemble de la gendarmerie. Seraient équipés de tablettes aux gens. Que 28500 terminaux néo-Paul seront donnés cette année. Que nous allons pour l'année prochaine, faire en sorte que nous ayons Vannes 2000 tablettes qui puisse être à nouveau distribué. Et enfin que nous aurons 10000 caméras piétons alors certes, on peut toujours dire que on peut faire plus mais, dire quand même qu'on ne fait pas d'effort sur l'équipement ça, ça me paraît quand même un peu osé, et je vous disais que j'étais ce matin devant le comité scientifique de la gendarmerie sur des problèmes très technologique, mais quelqu'un ajoutait avec raison. Disait on peut faire toujours de l'Intelligence augmenter, au fond, quand même, ce qui compte c'est l'Intelligence de l'homme, hé bien, nous pensons qu'effectivement, il faut l'Intelligence des hommes, et donc il faut plus de policiers et de gendarmes pour assurer la sécurité. Bien, monsieur le rapporteur spécial où vous avez demandé la parole monsieur Dominati, ensuite on va passer au vote. Comme le président leur a souligné cet amendement Monsieur le Ministre, était un amendement d'appel en début de mandature pour montrer, pour nous la priorité en ce qui concerne l'équipement, vous parlez des États bête mais il y a pas assez de voitures et le parc qui est vieillissant et vous le savez très bien, il a pris 2 années de plus, en l'espace de 6 ans, c'est la réalité, on ne renouvelle pas assez les voitures, on arrête l'entraînement de au stand de Tir au mois de septembre, il n'y a pas assez de cartouches, c'est la réalité quotidienne est-ce que l'amendement qu'a voulu soumettre la commission des finances, c'est de donner une chance au gouvernement d'inverser la tendance est de donner plus de moyens pour les hommes, lorsqu'il y a 3 postes créés on supprimé une voiture en matière d'équipement, nous voulons les 3 hommes et nous voulons la voiture c'était le sens de l'amendement, si le gouvernement ne donne pas un avis favorable à l'amendement pour la clarté des débats, je retire au nom de la commission des finances, cet amendement et la commission des finances, proposera le rejet de la mission sécurité. je crois que le ministre a répondu donc vous retirer cet amendement, donc on ne vote pas et on passe à l'amendement de Madame Assassi. merci, monsieur le président, général de la police nationale, déclaré, je le cite : le retour à la police de proximité est une bonne nouvelle, abandonnés depuis 15 ans alors que sa mise en place n'était pas achevé cette police est indispensable au moment où où on assiste dans certains quartiers à des phénomènes de radicalisation mais allez surtout indispensable pour renforcer le lien de confiance entre la police et la population parce qu'il s'est atténué, estompé et dans certains quartiers, il a disparu, je dois dire qu'il n'est pas le seul à s'en être réjouit puisque sur l'Euro, selon les résultats du baromètre réalisé par Fiducial Hourdeaux au même moment, pas moins de 84 pourcent des Français, considéré comme une mesure efficace de remettre en place sa police de proximité pour donc renforcer la sécurité dans les quartiers, alors qu'on l'appelle police de proximité ou police de sécurité du quotidien, j'oserais dire peu importe ce qui compte, ce sont bien évidemment les missions qu'on lui assigne et les moyens, ce dont elle n'a jamais pu bénéficier, or je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes au regret de constater que dans ce projet de loi de finances, aucune ligne budgétaire n'est dédié à cet objectif fort louable, reconnaissons-le, c'est la raison et tout le sens de l'amendement que nous avons déposée aujourd'hui. Bien l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Oui, Madame la sénatrice, vous soulignez à un sujet très évidemment très importante puisque c'est le président de la République qui a pris l'initiative au mois d'octobre, de réunir les principaux responsables de nos forces de sécurité pour changer cette orientation mais malheureusement nous ne trouvons pas comme vous l'avez souligné dans ce budget, une concrétisation, il y a pas un Euro prévu dans le budget pour la mise en place de la politique, la police de sécurité au quotidien, ce qui me gêne également, par contre, dans votre amendement c'est la c'est c'est la ne création d'une direction nouvelle et je pense que c'est le contenu de la faiblesse du montant symbolique que vous mettez sur cet amendement, moi je proposerais le retrait puisque vous avez exprimé votre préoccupation que je partage, puisque le chiffre n'est pas en cohérence et deuxièmement, je suis plutôt hostile à la création d'une nouvelle direction centrale spécifique pour cette police de sécurité au quotidien, donc avis retrait ou avis défavorable.

Oui, merci Monsieur Monsieur le Président, je partage une partie de la réponse que nous a fait monsieur le rapporteur, mais je, je vais le retirer mais pas parce que je partage la totalité de de vos propos, mais tout simplement parce que nous aurons l'occasion d'y revenir au moment du débat, de dos, de notre proposition de loi qui tend à réhabiliter la peau, la police de proximité et qui sera présenté au sénat, ici le 13 septembre donc nous aurons l'occasion de revenir sur cette proposition, comme sur d'autres d'ailleurs. Merci Madame Assassi donc cet amendement est retirée, donc il n'y a plus de discussions dessus, nous passons à l'amendement de Monsieur Ravier. Oui, merci Monsieur le président Monsieur, Président Monsieur Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je profite à mon tour de la Défense et demandant pour renouveler mon total soutien à nos policiers à nos pompiers à nos gendarmes qui, au quotidien, assure notre sécurité dans des conditions extrêmement difficiles au contact de certaines populations pas tout autant autochtones d'ailleurs trop souvent très hostiles aux forces de l'ordre et à tous ceux qui, au peut représenter l'État et la France. Dénoncer ses conditions de travail matérielle, financière et morale pour le moins critiquable, nombreux sont les policiers, j'en rencontre beaucoup à Marseille et qui me font part qu'ils sont obligés d'acheter eux-mêmes une partie de leur équipement indispensable à leur protection si les achats sur Internet n'existait pas, les policiers les auraient inventé tant il est vrai que ce gouvernement se soucie davantage des conditions de détention des délinquants et des criminels, plutôt que des conditions de travail au quotidien des forces de l'ordre pour vous en convaincre mes chers collègues, je vous invite à venir à Marseille, et de constater, dans quelles conditions de travail sont les policiers, les 13ème et 14ème arrondissements, dans quel état se trouve leur commissariat respectif, un seul mot : une honte et quand, le 24 novembre dernier un policier condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir administré une gifle à un migrant alors que la racaille qui a tenté de tuer un policier en mettant le feu à son véhicule est sorti libre du tribunal, comme les policiers comme les Français, je suis révolté par ce double scandale et ne peut dès lors que constater qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume républicain de France dans ces camps, disions, comment s'étonner que bon nombre de suicides que bon nombres de policiers et de gendarmes se suicide, cette année encore, alors que la menace est terroriste est toujours plus élevé, je propose par cet amendement de créer 25 en terme de renseignement territorial supplémentaires depuis le début de cette série infernale d'attentats qui frappent la France et l'accent a été mis sur l'exploitation du renseignement au sein des services de police et de gendarmerie services qui avait été démantelée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la police a créé la direction générale de la sécurité intérieure, les services central du renseignement territorial, la gendarmerie a lancé de son côté un plan pour créer des antennes de renseignement territorial 73 ont été créés depuis 2015, je propose de permettre le développement de ces antennes sur 12000 individus fichés pour radicalisation 1000 sont traités par la gendarmerie,

Monsieur Monsieur je m'en tiendrai une une réponse stricte sur ce qui figure sur votre amendement, c'est-à-dire la proposition : la création de 25 antennes supplémentaires de renseignement territorial qui en soit, effectivement, n'est pas n'est pas même si l'ampleur du transfert de de crédit opéré par cet amendement conduirait est moins important que d'autres qui vont venir ensuite cela conduirait son adoption conduirait à une diminution de, de 15 pourcent de l'action des interministérielle et communication, alors que le gouvernement fait de louables efforts de sincérité dans ce domaine puisque régulièrement je dirais ces crédits avaient été sous-évalué les années des la politique de sécurité routière doit trouver doit s'efforcer de trouver un équilibre délicat entre répression et prévention, et la réduction des crédits de la politique de communication ne serait pas un bon signe envoyé aux usagers de la route puisque ce que je pense que la sensibilisation et la prévention doivent être prioritaires en matière routière par rapport à la répression, donc avis défavorable. Merci monsieur le ministre, votre avis. Je veux d'abord redonner à nos collègues, un certain nombre d'informations aujourd'hui les moyens humains consacrés au renseignement sont considérables : nous avons en effet 4400 agents de la DGSI à ce jour, contre 3300 2014, nous avons 2630 agents affectés au renseignement territorial dont les effectifs de militaires de de la gendarmerie, des antennes de renseignement territorial, contre 1980 en 2014 et donc dans le cadre des 10000 créations de postes, dont je vous parlais tout à l'heure, 900 créations d'emplois seront faites au profit de la DGSI et du renseignement territorial. Parmi lesquels des gendarmes, donc oui, nous faisons un effort conséquent pour protéger nos concitoyens du terrorisme par ça nous semble quelque chose de tout à fait prioritaire donc les favoris. Merci 2 avis défavorables, il y a-t-il des explications de vote, je n'en vois pas, nous allons passer au vote qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient, cet amendement est rejeté, nous passons maintenant la discussion de 2 amendements identiques monsieur Baeza, c'est lui qui présente oui ah bon. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, j'associe à aux nombreux cosignataire de cet amendement notre vice-présidente Madame train de l'qui tout à l'heure, dont ce propos de discussion générale d'ailleurs à exposer tout l'intérêt de ce qui va vous être proposé après que notre collègue Vogel est quant à lui souligné la baisse continue des investissements des se dit ces 2 dernières années, ce qui n'est guère surprenant quand on sait qu'ils sont financés par les communes et les départements soumis à de très dures restrictions de dotation pendant le précédent quinquennat donc je vous propose, suite à la réforme de la prestation de filiation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, de revenir au à l'engagement qu'avait pris le gouvernement précédent d'abonder à minima, la dotation de soutien aux investissements structurants des SDIS à hauteur de 20 millions d'euros sur 10 ans la pérennité des montants financiers alloués devait permettent de concentrer buée directement à des projets nationaux tels que le déploiement d'un système unifié de gestion des appels des alertes et des opérations SDIS et de la sécurité civile à renforcer le maillage territorial DC10 à mieux coordonner l'action des acteurs à optimiser une réponse cohérente et équitable sur l'ensemble du territoire, or le projet de loi de finances de 2018 envisage de réduire de 10 millions les sommes promises pour l'investissement, 10 en conséquence c'est un amendement vise à respecter les engagements pris avec les élus départementaux à l'heure des aléas climatiques et des demandes d'interventions des sapeurs-pompiers de plus en plus nombreuses à urgente, nous vous proposons donc de rétablir les 10 millions d'euros de crédits pour arriver à un total de 20 millions d'aide à l'investissement dans les SDIS je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis : il y a un amendement identique, monsieur Capu. Oui, c'est à ce stade-là, l'amendement et défendu mais je j'interviens quand même, vous l'avez compris, il s'agit de porter à 20 millions d'euros, le montant total de la dotation de soutien aux investissements des SDIS on a et en CP pour tenir les engagements du précédent gouvernement, en 2017 et pour rendre possible la poursuite des dossiers de long terme structurant déjà engagé, même si effectivement on a bien noté que c'était un engagement du précédent gouvernement, ce sont 2 à 2 amendements rigoureusement identiques. Oui. à vous, monsieur le rapporteur.

Madame Catherine Tremblay tout à l'heure on on peut être tout à fait d'accord et je pense qu'une large majorité de la commission des finances aurait été d'accord avec je dirais l'objet de votre amendement la la difficulté si vous voulez, c'est que c'est une intention effectivement qui est louable, à laquelle on peut adhérer mais qui prive le programme 217 Éducation et sécurité routière du plus du quart de son budget, quant à l'action démarche interministériel de communication qui regroupe notamment toutes les campagnes de sécurité routière, elle trouvait à ses crédits diminuer de 16 millions 270 à 6 1000270, ce qui n'est pas sérieux disons dans un budget, le second, on va faire de la prévention en matière de sécurité routière, l'adoption de cet amendement, je dirais très une large partie du volet préventif de la politique de sécurité routière, c'est la raison pour laquelle tout en partageant je dirais votre souhait par ailleurs

Oui, comme je l'indiquais tout à l'heure donc, le gouvernement travaille donc en liaison étroite d'ailleurs avec l'Association française des départements sur un projet SGS GO qui vise à rendre compatible l'ensemble des systèmes et donc qui sera une grande avancée d'un point de vue technique je technologique et du point de vue de la sécurité pour ce qui concerne, vous me l'aviez demandé tout à l'heure monsieur le rapporteur, je n'ai pas répondu, nous aurons un comité de sécurité routière qui se atteindra début janvier sur lequel nous sommes en train de de travailler et nous aurons l'occasion de proposer un certain nombre d'orientation.

Merci beaucoup monsieur le président, Monsieur le Ministre, vous savez que ma démarche n'est nullement politicienne, mais c'est une démarche de conviction lorsque je parle de sécurité civile en ce qui concerne le budget de l'État consacré à la sécurité civile, c'est un budget moindre qui est totalement needed d'inadéquation avec les missions qui sont celles de de nos sapeurs-pompiers et les uns les enjeux qui sont les leurs, monsieur le ministre, pendant de nombreuses années, je me suis rendu compte que finalement, la baisse des dotations aux départements et aussi notamment le fonds d'aide à l'investissement, qui était un un fonds qui permettait justement hausse 10 d'investir dans des matériels de de de grande technicité bien ce fonds d'aide à l'investissement a été consacrée à Antarès entièrement et donc il avait, il est à 0 aujourd'hui, quand j'ai défendu également avec beaucoup de conviction, le texte de monsieur Baquet au mois de décembre dernier, sur la réforme de l'APF faire hé bien je l'ai fait également avec la conviction

avec cette idée qu'il y aurait un fléchage de ses deniers publics sur la sécurité civile, hé bien j'été particulièrement heurtée par le fait que cette ce budget soit amputée de ses 10 millions et aujourd'hui vous me dites, Monsieur le Ministre, que cette amputation se fait au détriment des projets structurels des outils sans merci, a eu un appel d'offres, ça sera honoré sur une année, mais pas sur les années à venir, je ne peux entendre cet argument et en ce qui concerne le le système j'au SGA, c'est un système qui se mettra en place sur du long terme, on ne peut pas aujourd'hui parler d'économie même des moindres économies sur le budget dix-dix alors je je soutient avec fermeté, j'appelle l'ensemble de mes collègues, comme ils ont pu le faire sur le texte de monsieur Baquet au mois de décembre dernier, de voter à l'unanimité, cet amendement, je vous remercie. de la Commission a demandé le retrait, vous répondez. Merci monsieur le président je ne retire pas la proposition d'amendement, je suis bien conscient des imperfections qui résulte de l'application des règles pour trouver les 10 millions mais je pense que pour d'autres propositions pourront être faites, le moment venu, en attendant, je voulais qu'on exprime notre volonté unanime de préserver ou synonyme que possible de préserver les capacités d'investissement des SDIS, avec une aide de l'État, qui soit un peu conséquente et non pas réduite à la portion congrue. Il y a donc, si je fais le point, la Commission avait demandé le retrait, il n'y a pas de retrait, donc un avis défavorable, donc avis défavorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour. Excusez-moi, monsieur, pu se manifeste pour son amendement identique. oui, parce qu'il y a, si on vote sur les 2 amendements, il faut que je donne mon explication, vous avez compris que c'était un amendement d'appel d'ailleurs, ce sont plutôt 2 amendements d'appel

de la mission interministérielle, la démarche de la mission démarche interministériel et communication de telle sorte que je retire effectivement, pour ma part mon amendement, étant donné qu'il me semble que nous avons bien d'attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de respecter les engagements du précédent gouvernement. Bien, donc ça ne change pas grand chose au vote puisque vous le retirez mais comme l'autre identité maintenu, nous votons, qui est pour l'amendement. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission sécurité figurant à l'État B. je n'ai pas été jeudi était saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite du jeu mais au mois les crédits de la mission qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Eh bien, les crédits sont rejetées. J'appelle en discussion : les articles 62 62 quater et les amendements tendant transférer des articles additionnels qui sont rattachés pour leur examen aux crédits de la mission sécurité qui viennent d'être rejetés. Donc je me on voit ces articles article 62 terre qui est pour. Qui est contre. Je pense qu'il va falloir recompter, puisque personne pour personne, personne s'abstient, on aura un problème donc est-ce que la Commission veut donner son avis pour éclairer notre assemblée. avis, c'est un avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient l'article est adoptée après l'article 62 terre un amendement de Madame Nathalie Goulet, à vous la parole. monsieur le président Monsieur, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement qui avait déjà été adoptée précédemment dans un budget précédent concernant un rapport liée au dépenses sur le financement des activités de prévention de la lutte contre le terrorisme, il y a une coquille et non pas de prévention et de lutte contre le terrorisme, il s'agit des actions de prévention vous savez monsieur ménisque que ces actions de prévention sont dispersés, dont on ne sait pas combien de programmes que par ailleurs elles sont confiées à un tas d'associations, alors on a pu, dans un texte précédent améliorer les dispositifs de contrôle de ces associations, mais néanmoins les Budgets nécessaires à la prévention. Sont extrêmement disparates et absolument pas contrôler, donc l'objectif de cet amendement est de pouvoir contrôler les actions de prévention parce que vous pourrez dépenser autant d'argent que vous voulez dans des mesures répressives, si les dispositifs liés à la prévention ne suivent pas, ça ne fonctionnera pas, j'ajoute à ce sujet, Monsieur le Ministre, même si vous n'écoutez pas qu'qui serait quand même utile merci qu'il serait plutôt intéressant et j'en ai parlé dans le cas de l'abus de de la mission de pouvoir confier à des missions de lutte contre la radicalisation aux épisodes qui sont extrêmement bien structuré et qui pourrait tout à fait jouer ce rôle, puisqu'en ce moment, on est en train de chercher désespérément des structures capables de recevoir des jeunes en voie de radicalisation ou des ou des jeunes suivis, je crois qu'aujourd'hui toutes les actions de prévention sont extrêmement nécessaire donc, cet amendement vise à avoir un contrôle par le Parlement des dépenses qui sont effectuées de façon à mieux pouvoir les contrôler, je trouve que c'était quand même notre travail, la prévention est absolument essentiel, monsieur le Ministre quand on connaît le nombre de jeunes radicalisés aujourd'hui sur le territoire, sans compter ceux qui reviennent et qui poseront également des problèmes, c'est l'objet de cet amendement. monsieur Dominati pour la Commission va travailler. Madame Goulet a souligné que le Sénat s'est déjà posé cette question et a souhaité remédier à un certain nombre de précisions concernant le renseignement, notamment lors du débat budgétaire, je rappelle, monsieur le ministre, que notamment dans la lutte contre le terrorisme et concernant les services du renseignement intérieur, nous avions souligné que en matière dans la mission sécurité nous n'avions pas les mêmes éléments que le ministère de la défense nationale et que, par exemple dans le ministère de la Défense nationale, les services de renseignement extérieur était très clairement fléchées, je dirais, en terme de budget sur les moyens et sur les personnels et nous avions souhaité qu'effectivement cela apparaisse au budget de la mission sécurité puisque, si le ministère de la Défense nationale pouvait faire cela, il y avait pas de raison que le ministère de l'Intérieur ne puisse pas le faire sur la sécurité intérieure, ça n'a pas été fait par vos prédécesseurs, peut-être que je je dirais vous entendez pour la première fois l'appel de Madame Goulet ou du Sénat, pour laisser peut-être un temps à l'amélioration des documents budgétaires, la commission des finances avait émis un avis de sagesse, mais plutôt défavorable Madame Goulet pour laisser le temps à ce gouvernement de répondre à votre question. Bien, donc il y a une nouveauté dans l'hémicycle sagesse défavorable, c'est défavorable, ça veut dire oui donc défavorable, Monsieur le Ministre. Oui, j'ai bien entendu le 1er cri de Madame Goulet mais comme le dit monsieur le rapporteur, faut se donner un peu de temps pour la réflexion, et donc je vais peut-être attendent le 2ème cri pour pouvoir effectivement me faire un avis, je vous rappelle d'ailleurs que sur l'ensemble de ces actions, a dit dans la loi si on fera un rapport global sur tout ceci et ce sera dans 2 ans, donc nous aurons l'occasion de revoir tout cela, on sent. Merci, il y a-t-il, oui Madame Goulet, vous avez la parole. Oui, Monsieur le ministre, je je je voudrais pas mais gosier et attendent que de je préfère mes explications, j'ai pas l'intention de crier j'ai jamais vu dans cet hémicycle, je voudrais simplement vous dire que dans le cas de la loi antiterroriste, nous avons voté des mesures de contrôle des associations en charge de la dé-radicalisation j'entends tout à fait la voix de la commission des finances, qui en général et la voix de la sagesse et j'retirer cet amendement mais monsieur le ministre, il nous faut absolument un contrôle des Budgets parce que vous ne pouvez pas exclure les effets d'aubaine, vous ne pouvez pas bon, il y en a et donc, quand vous regardez le jaune budgétaire et quand vous regardez la dispersion des moyens, compte tenu de la disette budgétaire général aider aidés et des moyens qui sont à la disposition de la lutte contre la radicalisation je vous demanderai à tout le moins comme Laval avait laissé faire votre prédécesseur Bernard Cazeneuve, de pouvoir aller rencontrer les responsables et parler avec eux de leur budget, je crois que c'est quand même extrêmement nécessaire qu'on puisse contrôler ses Budgets, donc je retire cet amendement mais le PLFR et pas loin et le prochain PLF arrivera très vite, merci Monsieur le Ministre.

Merci monsieur le président, Monsieur le ministre d'État, cette assemblée avec vous rendu hommage comme il se doit, aux forces de l'ordre qui protège nos concitoyens depuis maintenant de nombreux mois pourtant, nous le savons et le président de la République l'a indiqué lui-même, il y a un problème de confiance entre les forces de l'ordre et les jeunes qui vivent dans ces quartiers, c'est ce qu'il l'a dit lui-même, en mars dernier, je sais que vous êtes très soucieuse de rétablir cette confiance et je pense que vous aurez l'occasion de revenir sur la vertu que vous attribuez à la future police de sécurité du tout quotidien et pourtant depuis plusieurs mois, nous voyons que des discriminations et des disparités ce constat dans les contrôles d'identité. Un jeune à 8 fois plus de risques d'être contrôlé que un autre, un jeune homme d'apparence noir ou maghrébins à 80 pourcent de chances d'être de plus que d'autres et nous savons très bien que cela cause ce sentiment de tension avec les forces de sécurité, il est proposé depuis assez longtemps et j'ai, je dois le confesser peu de désespoir, de vous convaincre, Monsieur le Ministre d'État, mais pour autant, certaines grandes villes et vous le savez, Paris en fait partie, propose que soient expérimentées, ce qui s'appelle l'attestation de contrôle d'identité qui permettrait compris de le tracé ces processus de de contrôle donc, cet amendement a pour objectif simplement de demander au gouvernement de présenter un rapport dans les 6 mois afin d'indiquer de quelle manière, pourrait être mis en place cette attestation vous le savez, l'État a été condamné le 9 novembre 2016. Pour faute lourde pour des contrôles d'identité discriminatoires, donc ce n'est pas une une vue de l'esprit, un fantasme de personnes qui ne serait pas totalement ancrées dans la réalité, c'est bien la réalité que vivent nos concitoyens et notablement les plus jeunes et notablement ceux qui vivent dans des quartiers plus plus difficiles et donc, je vous demande, monsieur le ministre d'état d'examiner de manière très sereine et je compte sur votre talent pour expliquer ensuite aux policiers et aux syndicats de police que tout le monde a intérêt à ce que cela progresse dans cette voie.

je suis défavorable à cet amendement, d'une part, parce que cela irait à contresens par rapport aux tâches indues que je dénonçais tout à l'heure dans le rapporteur spécial puisque ce serait la délivrance de cette était station serait un travail supplémentaire à mettre à l'oeuvre des forces de l'ordre, d'autant que le ministère de l'Intérieur, c'est le 2ème argument et qui me semble le plus pertinent, développe les caméras piétons sur les agents et que notamment dans les 21 zones de sécurité, à titre expérimental je crois savoir, et il y a une grande efficacité sur ses caméras piétons qui sont, comme vous le savez, veut directement porté par les agents de la sécurité publique, donc l'avis de la commission est défavorable pour ces 2 raisons. Monsieur le ministre d'État. Monsieur le rapporteur de la commission des finances, défend avec tellement de conviction les arguments du gouvernement que je me demande s'il n'a pas comme avant, regret de ne pas avoir voté les crédits de la mission, j'y vois comme un encouragement pour l'avenir, donc même avis que le rapporteur de la commission des finances. Monsieur Grosdidier, vous avez demandé la parole. Oui, effectivement, d'abord pour rappeler que, lorsque les policiers et gendarmes consacrent les 2 tiers de leur temps aux procédures et seulement un tiers du temps à l'opérationnel, il convient de ne pas rajouter de la paperasserie à la paperasserie, deuxièmement vous soulignez un vrai problème, celui des relations dire entre les les policiers des contrevenants ou des contrevenants potentiels ou simplement des citoyens, parfois dans des zones qui sont des quartiers où les où les relations sont tendues, effectivement, la réponse a été fait par monsieur le rapporteur et par monsieur le ministre, sur les caméras individuelles, on peut s'en satisfaire, je regretterais simplement comme le rapporteur, les, l'équipement, soit pas plus rapide je regretterai aussi que nous en soyons toujours comme toujours trop timidement qu'au stade de l'expérimentation, il a fallu d'ailleurs que le Sénat se battent pour que les caméras qui équipait déjà les policiers municipaux ne soient pas retirées hors zone de sécurité publique, dire qu'il faut avancer, dès lors qu'il y a des caméras, hé bien les les citoyens sont garantis contre d'éventuels débordements des forces de l'ordre, les forces de l'ordre sont garantis contre les remises en cause injustifiée la hiérarchie est garantie contre les débordements des subordonnés et les magistrats disposent des éléments tangibles en cas de doute rajout de rebelles Lyon donc il faut aller plus vite dans cette direction, mais de ne pas rajouter de la paperasserie à la paperasserie. Alors il y a plusieurs demandes de prise de parole Madame taillé Oui, quelques mots pour pour préciser, monsieur le président Monsieur mise d'État que moi je soutiens cet amendement parce qu'il ne semble extrêmement important qu'aujourd'hui, dans notre République, dessine soit donné pour pour dire que

avec intérêt pour tous pour les forces de l'ordre, comme pour les publiques qui se sentent discriminés merci. La parole est à monsieur Karoutchi. Oui, monsieur le président, Monsieur le ministre d'État. Moi, je, je, j'entends bien ce que vient de dire Madame de La Gontrie sur cet amendement, mais de 2 choses l'une : au-delà de du problème des caméras, au-delà du problème si je puis dire, de l'évolution de la société, il y a, il y a déjà eu dans cet hémicycle un débat lorsque le problème s'était posé du temps de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, le problème s'était posé et le ministre de l'intérieur de l'époque avait lui-même dit : non, nous ne mettrons pas en place ce contrôle avec attestation tout simplement parce qu'au-delà des mesures prises par le ministre, c'est-à-dire que le ministre d'État, après tout, aussi sur la police, un pouvoir de tutelle, il fait des circulaires, il demande à ce que les choses se fassent. Si vous dites aux policiers non non non non, au-delà de ça, au-delà de la maison. Il faut une attestation. Qu'est-ce qui va se passer : Première éléments ça donnera le sentiment de la défiance à l'égard des policiers, il faut quand même dire les choses dans une situation qui est la nôtre, où la tâche des policiers, ce que l'on a dit tout à l'air avec l'ensemble des mesures qui doivent être prises avec le terrorisme, si vous dites en plus aux policiers, on n'a pas totalement confiance parce que c'est ça que ça veut dire, il faudra donc des attestations. Le sentiment dans la police sur un sentiment extraordinairement négatif et c'était déjà le cas à l'époque, les syndicats de policiers et le 2ème élément et on le sait bien, monsieur le ministre d'État, c'est que si vous faites ça et si vous dites ça et je comprends l'argument de fond le principe, mais si vous dites ça va beaucoup de policiers diront, déjà on est débordé et tous mes collègues l'ont dit, par la paperasse franchement. On va faire beaucoup moins de contrôles d'identité parce qu'on ne veut pas en plus avoir à faire de la paperasse supplémentaire qui suit ça devient impossible en tout à l'heure, tout le monde dit c'est trop, on n'a pas assez d'effectifs, il faudrait décharger l'amendement bah non, on va vous en remettre un petit peu en n'ayant pas des effectifs correspondants, donc moi je pense qu'il faut faire confiance à la police, c'est la police de la République et faire confiance au ministre d'État pour faire les circulaires et donner les instructions nécessaires pour que l'ordre public ne soit pas contradictoire avec la tolérance et la générosité naturelle. merci Monsieur le Président, je ne voterai bien sûr pas cet amendement pour l'ensemble des raisons que nos collègues ont exposé et je fait crédit à monsieur le ministre d'État, de sa volonté déployer les caméras personnelle sur l'ensemble de nos forces de l'ordre, je voulais quand même cependant, lui dire que si les gendarmes de personnes sont équipés de ces caméras suite aux événements tragiques que nous avons connu à Beaumont à personne, les environs en juillet 2016, c'est parce que la commune de persan, les a payés car l'administration était incapable de le faire à l'époque, cela nous renvoie au débat que nous avons eu tout à l'heure sur les moyens et justifie d'autant plus que le vote que nous avons eu merci. Monsieur Leconte, vous avez la parole. parce que finalement s'il s'agit de discrimination entre les citoyens qui est perçu, et qui est malsaine pour la cohésion de la société, alors je ne comprends pas, on peut par principe considéré que, compte tenu de la situation, il est inutile de surcharger le travail de la police, par ce type de démarche mais refusé même. De voir le problème. De se poser une question que le défenseur des droits, nous invite à regarder depuis plus de 5 ans. C'est quand même dommage, il ne s'agit pas de les voter, il s'agit simplement de demander un rapport pour regarder comment est-ce qu'on peut répondre à ce problème et je vais vous dire. Si il savez que ce sont les mêmes. Qui sont contrôlés : 5, 6, 10 fois par mois. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est du travail utile, c'est du travail inutile, vous, vous-même et vous empêcher la police d'avoir les outils de maîtrise et d'orientation de ces contrôles d'identité, donc vous pensez qu'en mettant un espèce de voile pour ne rien regardez-vous régler le problème, au contraire, je pense qu'il faut se poser la question et et là, on ne demande pas de l'établir de pas le mais sur l'ensemble du territoire de la République lorsque on demande une expérimentation à certaines communes qui le souhaitent, ça a été fait il y a quelques mois, on nous dit non et lorsqu'on demande un rapport, on nous dit, par principe, c'est pas possible, hé bah désolé je crois que, aussi, pour savoir un peu comment la police fonctionne sur ce sujet et pour l'aider à être plus performante, ça mériterait peut-être qu'on adopte cet amendement. La parole à Madame Esther Ben Bassa. Merci monsieur. D'accord avec mes collègues concernant cet amendement, puisque dès 2011 nous avions déposé une PPL et ensuite le ciel CE avait

sur ce sujet, bien sûr, je voulais rappeler que 2000 dès 2012 à séminaire de contrôles d'identité relations police-public pratique de police dans d'autres pays avait été organisé par le défenseur des droits de l'époque, monsieur Baudis et aussi bien la police des Britanniques, la police américaine et le le chef de l'expérimentation dans une banlieue de Madrid avait tiré les mêmes conclusions que la police avait longtemps n'est-ce pas refuser d'appliquer le récépissé mais qu'à la fin, lorsque le récépissé avait été impliqué, il y a, il y a eu un ratissage des relations entre la population et la police, ce qui a été positive et d'ailleurs par la suite Monsieur Rebsamen avait parlé, si ma mémoire est bonne, d'une expérimentation près de Dijon, de du récépissé à défaut de récépissé, je tiens à rappeler n'est-ce pas que les caméras proposé ne ne sont pas, on va, on ne les voit pas beaucoup, surtout qu'elles sont éteintes, lorsqu'il y a a des policiers qui l'époque mais très peu de policiers et que le numéro de matricule et souvent cachés, ça pourrait n'-ce pas pendant une période se substituer je tiens à rappeler également qu'après le ce qui est arrivé au jeune Théo, le ministre de de l'Intérieur avait proposé quelques milliers de caméras et nous les attendons encore donc, s'il n'y a pas d'olympisme récépissé au moins pour rétablir une certaine égalité entre nos concitoyens, il serait opportun que ces moyens proposés soient mis en place, merci. Merci, nous allons donc passer au vote, avec avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour cet amendement. Qui est contre. Qui s'abstient. Cet amendement est rejeté, nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur le les crédits du compte spécial, contrôle de la circulation et du stationnement routier figurant à l'État Monsieur aboutit, vous avez la parole pour l'amendement. 310. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, donc le présent amendement vise à diminuer de 20 millions d'euros, la subvention versée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions l'entaille en vue d'opérer un prélèvement à due concurrence sur le fonds de roulement de cet opérateur, en effet, le fonds de roulement de l'entaille dépassait 38 millions d'euros au 1er janvier 2017 donc en augmentation constante au cours de ces dernières années, alors ce un niveau prudentiels de ce fonds de roulement avait été estimée à 14 millions et demi les années les années précédentes sur ce sujet, on n'a pas obtenu, je dirais, de, de précision, d'information ou d'explication probante parce que un fonds de roulement, c'est fait pour financer un décalage de trésorerie entre des recettes et des dépenses, donc c'est essentiellement de la de la de la trésorerie, or l'entaille n'a pas décalage de trésorerie sur sa propre action, dans la mesure où l'ensemble des opérations qu'elle sous-traite en matière d'Editis, qui sont des opérations, effectivement, qu'il casse ou traiter des opérateurs extérieurs et il n'y a aucune raison qu'il y a des décalages de dates et de trésorerie entre le paiement des opérateurs extérieurs et l'éventuel recours Mans auprès des collectivités, Malik, ça peut prendre plusieurs mois, décalage ça veut dire que c'est une gestion qui n'est pas performante en en la matière parce que le fonds de roulement telle qu'il est constaté au 1er janvier représente quand même un tiers du budget de l'entaille, donc là il y a de l'argent qui, je dirais qu'il n'est pas utilisé correctement, à notre avis et les explications que nous avons obtenus ne sont absolument pas probante sur le sujet, c'est la raison pour laquelle on a maintenu cette cette disposition. Merci, monsieur le rapporteur de l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre d'État. compte tenu de l'intervention : 2018, 2 de rêve. Formes majeures : d'abord la décentralisation du stationnement payant l'entaille sera en effet en charge à partir du 1er janvier 2018 de l'édition et de l'envoi des forfaits de postes Ascione ment au nom au nom et pour le compte des collectivités territoriales qui choisiront de recourir à ses services, et enfin l'externalisation de la conduite des véhicules radar qui est appelé à générer un surcroît d'activité en matière de procès-verbaux électroniques et tout à l'heure, on a parlé de sécurité routière, c'est une des mesures importantes que nous allons développer en la matière. monsieur le ministre, je mets donc cet amendement au mois avec avis défavorable du gouvernement, c'est un amendement de la commission des finances, qui est pour.

la dotation totale du programme 754 contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun de la sécurité de la circulation routière dans le projet de loi de finances 2018 est en nette diminution, moins 22,3 pourcent par rapport au crédit de qui figure dans la loi de finances initiale pour 2017, ce qui est destiné aux collectivités locales dans la répartition qui est qui est effectué entre l'État, l'entaille la Fifth etc, la part des collectivités locales, baisse de 148 millions et donc se trouve réduit à 516,6 millions d'euros, il faut indiquer que dans le passé, les collectivités, bénéficier de l'intégralité du prélèvement de 170 millions issus des amendes forfaitaires radar et que dans le projet de budget pour effectivement 2018 n'en percevrait plus que 75 millions, soit une réduction de 95 de cette, de cette mesure est une anticipation sur les conséquences que pourrait avoir la décentralisation de de du stationnement payant qui ne commencera qu'au 1er janvier 2018 et dont les conséquences financières, au moins dans un 1er temps sont relativement incertaines puisque ce qu'il peut y avoir plus de recettes pour les collectivités, mais la première année, les collectivités peuvent être aussi amenées à investir dans des changements de matériels, des changements de 2 systèmes, ce qui est proposé, je dirais par le l'opération envisagée, c'est de maintenir les les crédits de l'État au niveau du désendettement du budget au niveau de l'an dernier, donc il y a pas de ponctions de l'État sur le le le désendettement de l'État, par contre effectivement de réaffecter 47,8 millions sur le le sur le le programme 754 en faveur des des collectivités qui verraient ainsi leur dotation diminuer de 15 pourcent au lieu de diminuer de 22 donc c'est un amortissement du dispositif dont on on peut accepter le, le, je dirais le le le principe mais avec Amona vit une anticipation un petit peu rapide des conséquences que vont avoir les réformes envisagées en matière de décentralisation du du

L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, comme on vient de le dire, il s'agit donc de savoir quels seront les effets de la réforme, qui donc sera faite à partir du 1er janvier 2018 même si la diminution exacte des recettes liées aux amendes de police ne peut être déterminée en amont de la mise en oeuvre de la réforme, dans la mesure où elle dépend de facteurs par nature imprévisible comme le comportement des automobilistes, la perte globale de recettes pour l'État, a été estimé à 200 millions d'euros quelques d'après la répartition 2014 du produit des amendes de police dernière répartition disponible au moment des simulations, la clé de partage du produit des amendes de police sur le compte d'affectation spéciale circulation et sécurité routière, c'est-à-dire 53 pourcent pour les collectivités locales et 47 pourcent pour l'État, a été appliquée à ces 200 millions, ce qui aboutit à une perte de 106 millions pour le programme 754 et 94 millions pour le grand programme 755 afin de garantir la neutralité pour le budget de l'État, de la réforme de la décentralisation du stationnement payant ces 94 millions que je vous concède : nous avons arrondi à 95 financeront le désendettement de l'État. Donc c'est un avis défavorable. monsieur ministre c'est un avis défavorable, oui, donc, qui est pour. Peut-être que je dois indiquer que la commission a dit qu'elle était favorable à son propre amendement. y a, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Cet amendement est rejeté, nous allons procéder au vote des crédits du compte spécial contrôle adopté Nous allons procéder au vote des crédits du Congo spécial, contrôle de la circulation et du stationnement routier figurant à l'État aidé. Il aucune idée si question de vote qui est pour. qui est pour. Il s'abstient c'est adopté, je vous vois l'art. Que 67 qui est rattachée, pour son examen au crédit du compte spécial au contrôle de la circulation et du stationnement routier qui est pour.

S'appelle aux discussions maintenant l'amendement on on a inséré un article additionnel, qui est rattachée, pour son examen au crédit du compte spécial, contrôle de la circulation et du. Stationnement routier, monsieur le rapporteur, qui avoue. C'est le dernier amendement de cette. Cet amendement est une est une conséquence des couleurs exactement de l'amendement précédent, c'est un changement de modification du texte qui permet de rendre opérationnel l'amendement de virements de 47 millions 5 du désendettement de l'État en direction des collectivités locales Merci, et en conséquence, Monsieur le Ministre. Défavorable comme pour le précédent. Il y a, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il être adopté. Je vais suspendre quelques instants la séance on va dire qu'on va reprendre à 17

La science est reprise, j'ai été saisi. D'une demande de priorité de la commission sur l'article 52 afin qu'il soit examiné avant les crédits de la mission cohésion cohésion des territoires durant la séance de l'après-midi du mercredi 6 décembre selon l'article 44 alinéa 6 de notre règlement, la priorité est de droit quand allez demander par la commission, saisie au fond, sauf opposition du gouvernement. Il n'y a pas d'opposition du gouvernement donc la prière, la priorité étant ordonnée le gouvernement était contre, c'est le Sénat qui doit. Statuer

Oui, Monsieur le Président vous venez dire l'essentiel je voulais confirmer la sollicitation de la Commission sur cet examen par priorité de de cet article, nous avons considéré, sur proposition du rapporteur spécial Philippe Dallier qu'il serait plus pertinent pour la cohérence de nos débats de débuter par l'examen de cet article rattaché à l'émission avant de procéder au vote sur les crédits de la mission, donc je remercie le gouvernement de son avis favorable tout ceci étant pour demain après-midi. Très bien lors du jour appelle la suite donc de la discussion du projet de loi de finances adoptées par l'Assemblée nationale pour 2018 : nous poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions: le Sénat va donc examiner maintenant les crédits de la mission Immigration, asile et intégration et article 56 57 57 bis, la parole est à monsieur Sébastien Meurant, rapporteur spécial de la commission des finances pour 100 minutes. Monsieur le président, Monsieur le ministre mais, chers collègues, cette mission s'intitule Immigration, asile intégration. Nous non, je voudrais vous présenter quelques remarques préalables pour le PLF 2018 tout d'abord je voudrais dire que ce budget ne semble, la première chose qui saute aux yeux à la lecture de ce budget, ce qui n'est pas sérieux. Du plan de vue financier que le chiffre sont manifestement erronée, nous l'avons dit à maintes reprises en commission, cette mission est globalement sous-budgétisé très sous-budgétisé alors moins que l'année dernière mais toujours sous médiatisées, spécialement dans un contexte de crise migratoire que nous traversons depuis quelques années et que nous continuons à traverser ces Siffre non seulement sont fantaisistes mais incohérent ainsi apprend-on que les crédits pour la lutte contre l'immigration irrégulière vont baisser de plus de 7 pourcent alors même que le gouvernement nous annonce une hausse de plus de 10 pourcent pour l'accueil des primo-arrivants, peut-on m'expliquer par quel miracle, nous pourrions accueillir davantage d'étrangers et que, dans son contingent, il y a moins d'étrangers à reconduire à la frontière. Parmi les incohérences je relève aussi que les demandes d'asile au titre de la procédure Dublin ne sommes pas comptabilisés, alors même que ces demandant en augmenter de 114 pourcent en 2016 et s'cusez du peu, encore un dernier exemple, alors que le financement global de la mission est notoirement insuffisant, alors qu'on le diminue le budget de la lutte contre les médias sont clandestines, on augmente de 62 les crédits dédiés au financement des centres provisoires des berges ment le nom même de la mission et mensonger cette mission s'appelle Immigration, asile, intégration, la réalité c'est que bien peu de choses, ils sont faites pour l'intégration, à peine 14 pourcent du budget de la mission pratiquement rien non plus n'est fait pour bâtir une politique migratoire digne de ce nom, savez-vous quelle part du budget de cette mission est consacrée à la lutte contre immigration clandestine 6 pourcent seulement, le gros de la mission, c'est l'asile 71 ne faisons pas semblant de discuter d'une politique de l'immigration de l'asile et l'intégration, nous comptons de gérer assez mal d'ailleurs, la crise des demandeurs d'asile sans réfléchir à ce que nous souhaitons pour notre pays et pour son avenir, mais même la politique de la ville qui se taille la part du lion de cette mission est dans un état calamiteux en 2017, le délai moyen de traitement d'un dossier s'élevait à 449 jours 2 fois plus que l'objectif affiché de 202 jours et cela, en particulier parce que l'asile a été presque totalement détourné de son objet naturel pour devenir, nous le savons, une nouvelle filière d'immigration clandestine, nous n'avons malheureusement pas de politique d'immigration digne de ce nom et ce n'est pas nouveau monsieur, ministre, je vous le conseil. Aujourd'hui les l'immigration clandestine et non une façon de venir en aide aux persécutés, contraints de fuir leur pays. pour aurait dû suffire invalider totalement, totalement les chiffres du gouvernement, on estime en effet que le coût de reconduite à la frontière et de leur de 4200 euros par personne, même en estimant en fourchette basse que seulement 30000 personnes sont déboutés, chaque année, le droit d'asile, cela devrait entraîner un budget de reconduite à la frontière d'au moins 126 millions d'euros, or on nous propose un peu moins de 83 millions d'euros, cette politique est dangereuse, dangereuse pour la France, dangereuse pour les Français, dangereuse pour les étrangers, dangereuse pour la France, qui se voit ainsi privé de ce choix élémentaires des nations souveraines choisir qui nous voulons accueillir chez nous, notre collègue Georges Patient évoquait le 17 octobre dernier la question de l'immigration clandestine, particulièrement dramatique en Guyane et signalait même que certains là-bas parlait de génocide de de substitution, le terme est fort sans doute exagéré mais qui peut nier que 11000 demandes d'asile pour 250000 habitants constitue un chiffre difficilement supportable, c'est à ce sens de politique est aussi dangereuse pour les Français je n'ignore pas qu'il n'est pas très bien vu de lier immigration terrorisme et insécurité mais d'abord je note que ce lien a été fait par l'État islamique lui-même qui a invité les à se glisser parmi les réfugiés et surtout le coordinateur de l'Union européenne, de la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove embraya avec des mises en garde particulièrement clair et Net que naturellement les commentateurs bien-pensants ont traité par le mépris, moindre ce n'est pas le moins des paradoxes nobs, absence de politique migratoire doublé de toutes les pompes aspirantes de l'État-providence déploie pour attirer toute la misère du monde et dangereuse pour les candidats à l'immigration est le même : le drame qui se joue actuellement en Méditerranée l'esclavage qui se répand comme une traînée de poudre en Libye sont directement liées à notre laxisme en matière de politique migratoire qui a donné des ailes aux passeurs aux trafiquants de Chair humaine, si le gouvernement le souhaitait réellement l'armée pourra mettre fin aux flux migratoires en quelques jours, déclarait le numéro de l'ex-numéro 2 de l'Otan en Afghanistan, le général italien Santo, cette absence de politique est aussi profanant injuste

la parole est à monsieur Buffet. Pour avis. Monsieur le président. Rapporteur monsieur le ministre, ministre d'État, au titre de la commission des lois, 3 minutes pour vous dire que, certes, le budget de la mission asile, immigration, intégration est en hausse de 10 pourcent en autorisations d'engagement. Certes, le Sénat a été entendu ce qui n'est pas toujours vrai concernant la construction en 2018, 2, 3 nouvelles 3000 nouvelles places pour les réfugiés en centre provisoire des berges ment. Mais sur ce budget 3 grandes difficultés persistent, la première, c'est une politique d'intégration en grande souffrance, au-delà des mots, 2 exemples. La réduction de 76 pourcent du nombre de visites médicales de l'office entre 2016 et 2017 qui nous pose je crois incontestablement un grave problème de santé publique, notamment dans les universités. Et puis le fait que près de 40 pourcent des étrangers en situation régulière qui suivent les formations linguistiques du contrat d'accueil et d'intégration n'atteignent pas le niveau de français requis. Alors que le budget propose une augmentation de 12 pourcent des crédits consacrés à l'immigration régulière, il nous faut revoir, je le crois sincèrement toute cette politique d'intégration, parmi celles-ci, il conviendrait sans doute d'abroger rapidement les circulaires dites valse de novembre 2012, qui par ailleurs ont contribué à augmenter de 31 ans et demi pour 100 le nombre de régularisations d'étrangers en situation régulière, constituant par le fait, une voie d'appel d'air réel pour les passeurs 2ème difficulté les déboutés du droit d'asile année dernière c'est environ 53600 déboutés qui nous sont venus engorger si vous permettez, suppression, le système d'accueil des demandes d'asile au détriment des personnes persécutées dans leur pays ou des victimes de guerre. Ils alimentent bien sûr l'immigration irrégulière et c'est bien là la 3ème grande difficulté immigration immigrés et régulière en métropole, mais également sur le territoire ultramarin sur ce point, les crédits sont en baisse de 7 pourcent par rapport à 2017, monsieur le ministre d'État, la fin du démantèlement de la jungle de Calais expliquer pour partie ce chiffre, mais c'est un argument ne peut pas résister très longtemps à l'analyse pour 3 raisons : d'abord les 10 millions et demi d'euros du démantèlement de Calais aurait très bien pu être utilisé pour améliorer la politique d'éloignement, je rappelle que pour la seule année 2016, 75787 personnes se sont maintenus sur le territoire français, sans en avoir le droit, nous ne pouvons pas les uns les autres ignorer cette réalité enfin l'enveloppe budgétaire dédiée aux éloignements forcés de permettra, selon nos calculs, que 14500 éloignements en 2018, c'est-à-dire un peu moins mais revoir nettement moins que sous le mandat précédent, il faut s'il voulait tenir l'engagement pris par le président de la République véritablement forcé sur ce point, les moyens de notre police, les Budgets des centres de rétention ministre sera légèrement inférieures à l'exécution de 2016 alors que le taux d'occupation a augmenté de 40 pourcent notamment à la suite des événements de Marseille, il faut donc se redonner des moyens aussi pour cela, ce sont les raisons pour lesquelles à l'impatience de monsieur le président de séance, je réponds que le commission des lois a décidé, a émis un avis défavorable, merci.

sujet, de 10 minutes pour intervenir. Et la parole est à monsieur Antoine Karam pour le groupe, la République en marre. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs mais, chers collègues, ce budget est essentielle puisqu'il semble traduire la volonté du gouvernement de mieux maîtriser les flux migratoires optimiser le dispositif de la ville et renforcer les moyens dédiés à l'intégration, nous avons tous conscience de l'importance de ces enjeux sensibles et de notre responsabilité en débattent et je le dis sereinement la mission Immigration, asile et intégration a doté d'un milliard 300 millions d'euros de crédit et progresse ainsi de 285 millions je je tiens à saluer la décision du gouvernement d'augmenter les moyens alloués au dispositif pour répondre à la pression migratoire exceptionnelles que connaît la France compte tenu, il faut le reconnaître, du contexte budgétaire contraint, c'est évidemment une avancée en commission notre rapporteur a présenté de nombreux Schiff, certains d'entre eux se sont avérés incomplet, en effet, notre collègue de Mayotte le collecte Annie Mohammed dit lui-même à le souligner l'immigration clandestine a mesuré à travers les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, or cette aide n'est pas applicable à Mayotte, pourtant, vous en conviendrez, monsieur le Ministre, le recensement des clandestins est essentielle pour apporter une réponse adaptée si la pression migratoire auxquels font respectivement face la Guyane et Mayotte et ça a été souligné sont souvent évoqué dans nos débats la gravité de la situation reste largement sous-estimé,

en 2016, ce sont plus de 22600 retours qui ont été opérés à titre de comparaison, le ministère de l'Intérieur a lancé pour la même année, près de 13000 reconduites aux frontières de l'Hexagone, je rappelle que Mayotte détient par ailleurs le taux de natalité le plus élevé de France et que 70 pourcent des femmes qui accouchent en situation irrégulière, voici maintenant le second chiffre pour la Guyane. 11000 c'est le nombre de demandes d'asile enregistrées au cours des 3 dernières années, notons que ça demande concernerait au total plus de 20000 personnes en comptant les familles, là encore, c'est comme si la France comptabilisait chaque année près d'un 1000000 de demandeurs d'asile sur son seul territoire hexagonal, chers collègues, demander l'asile atteint droit.

en 2016, seuls 2,6 pourcent des dossiers ont été acceptés par l'Ofpra, les reconduites à la frontière sont importantes, mais elles sont coûteuses et souvent il nous faut aller plus loin, innover et développer des mesures structurelles Le président de la République a annoncé en Guyane, plusieurs mesures qui poursuivent cet objectif réduction à 2 mois du versement de la dame, accélération des délais de traitement conditionnement de l'accès au RSA à 15 ans de résidence sur le territoire, plutôt que de 5 ans ou encore des monétisation du revenu de solidarité récemment un nouvel élan vient également d'être donnée à la coopération avec le Suriname, notre voisin le voisin de La Guyane cela donne bon espoir que l'accord de réadmission signé en 2004 soit prochainement ratifier par notre voisin du Suriname. Par delà ce budget devant nous satisfaire, donc de voir le chef de l'État et le gouvernement ouvert un dialogue franc et responsable sur la manière de mieux lutter contre immigration irrégulière dans ces territoires au bord de l'asphyxie. Je souhaiterais maintenant appeler votre attention sur un autre point : la situation des mineurs non accompagnés ou isolées et l'accompagnement des départements le nombre croissant de sa jeune se déclarant mineurs isolés, passant de 4000 en 2010 à 13000 en 2016 pour Athènes, près de 25000 en 2017, cela entraîne la saturation des dispositifs de protection de l'enfance, les départements qui doivent accueillir et prendre en charge ces mineurs ne pourront faire face à cette évolution sans le soutien de l'État le 1er ministre la ministre la la santé ont confirmé un financement exceptionnel de l'État en 2018 cependant, l'enveloppe de 132 millions annoncés 132 millions d'euros semble en deçà de l'évaluation effectuée par l'Assemblée des départements de France, selon laquelle le coût final de la prise en charge des mineurs isolés ça lèverait un milliard d'euros, alors Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous éclairer sur cette situation d'urgence, comment évoquer tous ces sujets, sans penser au drame humain qui se joue en Méditerranée éligible ou non à la ville, nous devons assistance à ces victimes de trafiquants qui, lorsqu'elles ne sont pas poussés à la mort en mer sont vendus sur des marchés d'esclaves, ce qui est un véritable scandale mondial rappelant les heures les plus sombres de notre histoire, c'est cette même assistance que l'AME l'aide médicale d'État apporte quotidiennement aux personnes étrangères sur le territoire national, il faut le rappeler cette aide poursuit un double objectif humanitaire et sanitaire aussi, nous ne pouvons que regretter que la majorité sénatoriale a décidé de diminuer ses crédits de 300 millions d'euros, ces situations sont la preuve en Outre-Mer mer comme dans l'Hexagone, les défis migratoires d'asile et d'intégration ont profondément changé les réformes à venir ne peuvent donc se contenter d'être conjoncturel, monsieur le ministre d'État, notre groupe soutiendra ce projet de budget qui va dans le bon sens en prévoyant une eau significatif de crédits pour 2018, l'attention portée par le gouvernement sur ces sujets et les efforts consentis dans cette mission marque le point de vue par des réformes ambitieuses capables de répondre avec responsabilité dignité au défi migratoire de la France et de ses outre-mer, nous espérons que le gouvernement poursuivra ce travail avec le projet de loi relatif à l'asile et à l'immigration, je vous remercie. Merci. Madame Esther Benbassa pour le groupe communiste, républicain, citoyen écologiste pour 5 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre d'hectares, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le 14 novembre dernier la chaîne américaine CNN revelée au monde ce que nombre d'acteurs de la solidarité internationale dénonçait déjà la vente d'exilés noir sur des marchés aux esclaves en Libye ce trafic qualifié par le président maintenant lui-même de crimes contre humanité devrait nous ouvrir les yeux sur le sort de ceux qui sont jetés sur les routes ou à la mer par la misère, la guerre ou l'oppression devrait nous ouvrir les yeux, dirige et nous inciter à une certaine pudeur toute non son non-sens pas capable, hélas, je vous cite, monsieur le rapporteur spécial. vous l'ai dit, mais l'allocation pour demandeur d'asile Ada et de 360 euros pour une personne seule, non les bergers, sans aller chercher au bout du monde, le salaire minimal en Roumanie, et de 320 euros. Nous attirons l'immigration clandestine. Pouvons-nous un instant décemment imaginer que des gens acceptent d'être réduit à Minsk, en esclavage prennent le risque de se noyer dans la Méditerranée de mourir en traversant montagnes ou cette femme : 360 euros, cette mission est de fait biaisée d'avance mettre ensemble l'immigration asile intégration est un tour de passe-passe politique visant à mêler dans l'esprit de nos concitoyens 3 problèmes différents, permettant à certains d'évoquer à tout propos et hors de propos, comme le fait le rapporteur spécial Monsieur que je cite la menace qui pèserait sur une autre cohésion sociale habile n'est-ce pas notre pays a enregistré en 2016,17 demandes d'asile pour 1000 habitants, contre un taux moyen de 2,36 dans l'Union européenne un virgule 99 en Italie de 4,71 Grèce et de 8,83 en Allemagne. du Sud demande pour 1000 habitants en France, comment pourrions-nous dire que nous n'avons pas les moyens d'accueillir ces réfugiés décemment. La hausse prévue par le budget dont nous débattons aujourd'hui ne saurait suffire à garantir ni un accès effectif à leurs droits pour les demandeurs d'asile, ni des conditions dignes de subsistance, ce budget est finalement une illustration parfaite de ce qui caractérise le nouvel exécutif une distorsion permanente entre les mots et les actes, le président sauf lorsque indigne et assure que tout le monde sera logé dignement, d'ici à la fin de l'année. Et en même temps, les préfets prennent des décisions illégales, les forces de l'ordre attendent chaque jour dans le Calaisis dans la reliant à Briançon, à la à la sécurité et à la santé des exilés sans compter n'est-ce pas que Monsieur Collomb envoie une circulaire aux préfets pour augmenter la répression à l'endroit des réfugiés voilà bah, c'est une des contradictions supplémentaire et de ceux qui nous gouvernent et en même temps des mineurs ne sont pas protégés, ils dorment dans la rue, certains étant même l'employé depuis Menton vers d'Italie sans autre forme de procès et en même temps, les militants associatifs, les bénévoles, les simples citoyens font l'objet de poursuites et d'intimidation, de plus en plus nombreuses, quand ils font simplement preuve d'humanité et de solidarité, nous ne voterons pas ces crédits Himachal collègues tout à fait insuffisant à nos yeux, pour relever le défi de l'accueil de réfugiés, tandis que la majorité sénatoriale, elle votera contre aussi. Mais parce que le budget des reconduites à la frontière est en baisse. Même vote donc traduisant en l'occurrence 2 visions radicalement opposées de Nantes, société et des devoirs de solidarité humaine qui s'imposaient, hors de tout prétendu ironise : moi,

Oui monsieur, ministre d'État, Monsieur le Président mais chers collègues notre discussion et des points de vue assez différents, que nous venons d'écouter démontre le besoin de réformes en matière d'immigration en matière de droits de l'immigration à l'intégration, en passant par le droit des îles tout état interdépendants et la solidité de la chaîne ne tient qu'à celle du maillon le plus faible et les maillons faibles sont nombreux notre approche budgétaire concerne le volet franco-français, ce n'est pourtant qu'une partie du débat, tant ce qui se déroule sur le continent africain dans la zone sub-sahélienne, en particulier dans l'Afrique de l'Est en Libye ou encore au Moyen-Orient a de l'importance, je mets à part à cet égard les questions concernant la Guyane et Mayotte quand était évoqué par Monsieur Karam avec beaucoup plus pertinence, ce que je ne pourrais le faire, nous avons à gérer, chers collègues, des cercles concentriques, si l'on se rapproche du territoire européen, le fonctionnement des accords de Dublin est en cause avec l'exercice effectif des responsabilités par les pays d'arriver, nous savons que ces engagements ne sont pas aussi respecter que nous aurions pu le souhaiter, ce qui pose aussi le problème d'une équité entre les pays européens, avec en arrière-plan, le débat sur le programme de relocalisation, qui est un peu la contrepartie que nous devons envisager si nous tenons à ce que les accords de Dublin soit intégralement respectée, la lutte contre l'immigration irrégulière poste collègues des questions budgétaires, mais son efficacité dépend aussi d'accords dits de réadmission, si la question du nombre effectif de mesures d'éloignement dépendait uniquement du budget alloué la réponse aurait été trouvée depuis longtemps nous savons, mes chers collègues, que cette question est plus complexe que simplement l'importance de l'écriture budgétaire je crois profondément que si le programme dit 303 Immigration, asile doit faire l'objet d'une discussion budgétaire classique, c'est notre mission, les enjeux sont ailleurs, à la fois dans la vision internationale, des choses comme dans la refonte de la mise en oeuvre du droit de j'espère, Monsieur le Ministre, que vous pouvez nous en dire plus sur les projets du gouvernement en cette matière si je reviens à l'approche strictement budgétaires l'essentiel des crédits vont à la garantie du droit d'asile, avec une augmentation importante en autorisations d'engagement en crédits de paiement votre budget Monsieur le Ministre, doit au moins être crédité d'une recherche de réalisme et de sincérité en mettant fin à une sous-estimation systématique des dépenses dans ce domaine, l'inflexion me semble notable est favorable, même si j'ai bien entendu les propos de notre rapporteur pour avis monsieur Laurent qui, de manière peut-être légèrement paradoxale si des permis d'exprimer avec le plus grand respect mis en balance à la fois ce qu'il estime être une forme dans ces séries d'insincérité et en même temps une augmentation très forte aider et crédits sur cette fameuse garantie comme je vous l'indiquais précédemment, je crois que l'angle d'examen du budget par le seul volet nombre d'éloignement forcé budgétés en 2018, ce qui est bien sûr important en matière d'immigration irrégulière, soit 14500 suivant le chiffre qui nous a été communiquée par Pierre Noël Buffet et vraiment réducteur, tant l'efficacité de ce site dépend d'éléments plus jours que les seules données budgétaires, je partage l'importance pour la crédibilité de l'action gouvernementale d'une efficacité réelle et d'un traitement différencié entre les personnes qui peuvent bénéficier du droit d'asile et les migrants dits économiques, le délai de 15 mois en commission pour traiter les demandes du droit d'asile à l'heure actuelle n'est pas acceptable, il convient de comprendre comment nos voisins allemands ont pu réformer leur système tout en respectant les dispositions de leurs lois fondamentales de leur cour constitutionnelle qui n'est pas moins exigeante que la nôtre comme de la CEDEAO, enfin, je serais assez attentifs Monsieur Ministre à ce que vous puissiez nous éclairer par votre analyse sur la portée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 27 septembre 2017 qui porté interprétation du règlement de l'Union européenne numéro 604 2013, doit-on comprendre que cette question peut être traité par la voie législative française, comme le pensent nombre de nos collègues à l'Assemblée nationale, doit-on comprendre que ceci nécessite une réforme du règlement européen et du dispositif du tous ces points me paraissent répondre au moins partiellement aux 3 domaines pointer avec justesse par François-Noël Buffet, en résumé, en vous renouvelant personnel même si de manière majoritaire notre groupe suivra les rapporteurs pour avis, donc on vous renouvelant mon approbation monsieur ministre des efforts budgétaires marqué que vous nous proposez, je vous appelle à un dialogue avec le Parlement afin d'améliorer l'efficacité des mesures actuelles afin aussi nous permettent d'avancer sur une réforme du droit d'exil en appréciant ce qui relève du législateur français ou du droit de l'Union européenne, au-delà des enjeux négociations ou de renégociations de nombre d'accords bilatéraux.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, asile et immigration, ce sont 2 politiques distinctes qui ne devraient pas être discuté ensemble, car cela porte à confusion, bien entendu, il y a des intersections entre ces 2 politiques, l'usage du droit d'asile pour rester sur le territoire, dans certains cas, la politique de gestion des maintient en ces situations irrégulières des déboutés du droit d'asile, enfin, l'intégration des personnes protégées, mais la ville, c'est d'abord un droit pour chacun, c'est pour la France un engagement, une traduction de nos valeurs, un principe qui est à la fois constitutionnel et un engagement conventionnel de ce point de vue, je voudrais d'abord saluer les orientations de la politique d'asile qui du gouvernement mais aussi et d'abord de, de ce qu'il a plus fait entre 2012 et 2017 et qui ont profondément réduit les délais d'étude des demandes d'asile et rendre à cette, à ce stade, un hommage à l'Ofpra et à la CNDA pour leurs actions tout en soulignant qu'il convient aujourd'hui de faire aussi des efforts en amont, c'est-à-dire sur l'accueil des demandeurs d'asile, les délais pour enregistrer une demande d'asile sont aujourd'hui scandaleusement on ne respecte pas les directives européennes et en aval, c'est-à-dire une fois que vous êtes protégé pour avoir le maximum, la capacité d'être intégré le plus vite possible dans la société française, je voudrais aussi saluer le travail de l'Ofpra, du ministère de l'Intérieur et de nos consulats pour la délivrance de visas pour Aziz c'est petit par rapport à l'ensemble des demandeurs d'asile mais c'est essentiel et mérite d'être développé car il n'est pas acceptable d'être obligé de risquer sa vie de risquer la vie de sa famille pour avoir des droits et pour pouvoir être protégé et je salue, de ce point de vue-là les les orientations du du président de la République, mais Monsieur le Ministre, nous avons aussi quelques inquiétudes sur le paquet asile en cours de négociation, la notion de pays tiers sûr auquel certains pays de l'Union européenne tienne et qui consiste à poser qu'un autre pays peut remplir à notre place, nos engagements convives conventionnel, en ce qui nous concerne, ça serait un déni de nos engagements et à un déni de notre de nos principes constitutionnels, comment voyez-vous, Monsieur le ministre, les orientations du paquet asile et l'incapacité pour le moment des Européens de converger sur ce point, je suis aussi perturbé par le fait que, aujourd'hui, dans notre droit la France ne donne pas aux demandeurs d'asile qui sont en demande depuis plus de 9 mois un droit effectif au travail, je crois que ce sera utile à la fois pour l'intégration, mais aussi pour les coûts enfin nous pouvons discuter des moyens, nous pouvons aussi discuter d'un certain nombre d'utilisation des moyens, j'ai été très choqué personnellement de du témoignage reçu de certains journalistes sur les mineurs reconduits à la frontière franco- italienne par des températures négatives au milieu des Alpes et sans aucun accompagnement ou sans aucune accepte de l'autre côté de la frontière en en Italie, je maintiens est aussi sur les conséquences du message que vous avez transmis après l'attentat de Marseille le limogeage du préfet de l'Union, quand on voit maintenant Dekra surchargés, des véhicules de police et les fonctionnaires de police qui font parfois 800 kilomètres par jour pour déposer d'une queue de, d'une part de la France à l'autre, un étranger qui a été constatée en situation irrégulière sur la surcharge des l'incapacité personnels qui travaillaient constatera à continuer à travailler dans ces conditions et par conséquent la dignité des personnes qui sont retenus retenus le le non-respect aussi de la décision de la Cour de cassation, sur la nécessité d'éviter les placements en crabe pour les dublinés décision de septembre, le 2013, enfin l'usage des tests osseux qui sont des, des, des escroqueries scientifiques qui ne permettent en rien de régler le problème des mineurs non accompagnés, je m'inquiète aussi sur l'avenir de d'une zone Schengen où finalement on arrive à donner un nouveau mandat Frontex pour protéger les frontières mais les pays européens n'arrivent pas à se mettent d'accord pour une politique d'asile plus intégrer, on ne peut pas laisser les pays de première entrée seuls face à leur fixation géographique, nous risquons à la fois une explosion de la zone de la zone Schengen et de voir ces pays comme un peu l'Italie a essayé de le faire avec la Libye en dépit finalement en ne respectant pas un minimum de, de, de, de principes de, de, de dignité envers les personnes qui essaye d'arriver sur le sol européen, monsieur le Ministre, l'immigration n'est pas une clé, il est préférable d'être un pays qui fait envie, plutôt qu'un pays que l'on fuit la capacité d'innovation d'un pays, elle se mesure à sa capacité de maîtrise et de la diversité des Hachd échanger des savoirs, de s'adapter aux nouveaux besoins et les personnes,

ne voyant pas d'immigration comme quelque chose de misérabilisme, mais au contraire comme quelque chose de positif pour l'économie qui accompagne la croissance de l'économie, nous avons tous été choqués par les images de CNN le choc, le scandale mondial de cette indignité de l'esclavage moderne, au sud de la Méditerranée, mais finalement. Le colonel Kadhafi sous nous permettaient de ne pas voir ce qui existait déjà, il ne cachait à nos consciences et finalement, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui nous voyons tous alors si aujourd'hui et l'Europe et l'Afrique ne peuvent plus faire semblant de ne pas voir ce qui se passe au sud de la Méditerranée, trouvant les moyens pour essayer d'éviter que cela continue monsieur ministre le président République a pris des initiatives en la matière, pensez-vous qu'avec nos partenaires européens et africains, nous pourrons vraiment avancer dans ce domaine et détruire les mythes qui peuvent conduire les gens à prendre des risques. Dans des conditions innommables est absolument indigne notre ses responsabilités, mes chers collègues, à Lourdes, car ces politiques pour réussir, ne sont pas que des politiques françaises doivent être des politiques européennes, l'attitude européenne sur ces questions, c'est d'abord notre crédibilité par rapport aux voix aux valeurs que l'on proclame, c'est notre capacité à assumer notre trajectoire historique et nos responsabilités, c'est l'expression de notre confiance ou non dans l'avenir, et aussi dans nos voisins c'est pour toutes ces raisons que le groupe socialiste, même si il doit elle constate un effort de sincérité du budget, d'autres sur certaines des priorités marquée du gouvernement et s'abstiendra sur ce budget je vous remercie. Merci, Monsieur le comte, la parole est à Dany va troubler. Pour le groupe, les indépendants. monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Dans le projet de loi de finances pour 2018 la mission Immigration, asile et intégration représente avec 35 milliards d'euros en autorisant d'engagement et un 38 milliards d'euros en crise de paiement, soit une hausse de 10 44 ans, Jauzion bagages, moins de 26 pourcent en crédit de paiement. Par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. Mais ne nous trompons pas. Cette augmentation de crédit s'explique en réalité par les mesures d'ajustement de la politique d'asile à l'immigration qui ont été actés au gré de l'évolution de la crise migratoire en effet entre 2010 et 2007 16 le nombre de demandes d'asile en France a connu une hausse de plus de 102 la différence entre discours et les actes du gouvernement, je verrai si j'ai agi pour chaque composante. De cette mission budgétaire l'immigration régulière et l'intégration, l'exercice, droit d'asile et la lutte contre l'immigration irrégulière. En outre, le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit même une baisse des crédits de la mission, immigration, asile intégration d'ici 2020. Ce budget suscite de nombreuses remarques concernant 1er lieu l'immigration régulière et l'intégration des étrangers à la cité française.

Dans le projet loi de finances pour 2018, 240 millions d'euros son sont consacrés à l'immigration régulière et intégration, soit une augmentation de 12 et demi par rapport à la finance initiale produit 17, or il s'agit de financer les nouvelles missions de l'Office français de l'Immigration, de l'intégration dans la priorité n'est plus, intégration, la prise en charge des demandeurs d'asile. La fonction historique d'intégration, l'étranger plus moi, ils vont se trouve ainsi fragilisé l'asile étant devenue l'axe majeur de la politique le l'Office français de l'immigration, intégration. On constate également une réaction drastique du périmètre d'élite médicale d'étrangers, puis tous les étrangers souhaitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire devait passer une visite médicale, cette visite est inscrit de santé publique, aujourd'hui, c'est une minorité de de primo-arrivants qui passe cette visite, le nombre de ses vite a connu une baisse de plus de 100 de 16 pourcent entre 2016 et 2017. Nous déplorons également l'échec du contrat d'intégration républicaine près de 40 pourcent d'étrangers qui suivent les formations linguistiques n'atteignent pas le dire aux qui, en français, s'agissant, second lieu, droit d'asile, la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme, droit d'asile, a échoué dans son objectif de réduire le délai global des demandeurs d'asile qui s'établit actuellement à plus de 14 mois toute la procédure doit être revu depuis l'enrichissement de la demande, jusqu'aux voies de recours. Par ailleurs, le gouvernement ne semble pas réaliser aucun suivi précis des déboutés, droit d'asile, dont le nombre pour la seule année 2016 s'est levé à 53600 personnes. Ces déboutés en or l'engorgement, le système d'accueil au détriment des personnes percutées persécutés dans leur pays, fragilise la paix du droit d'asile. Concernant le dernier lieu, la lutte contre l'immigration régulière, on peut déplorer l'échec de la police de l'reconduite à la frontière les étrangers des étrangers en se sont irrégulières-t-il d'exemple pour la seule année 2016, c'est moins de 18 pourcent des mesures d'éloignement prononcées qui ont réellement été exécuté ainsi 75000 personnes sont maintenus en France en toute illégalité le 15 août dernier le prendre la République avait annoncé son intention d'expulser les étrangers en situation irrégulière ayant commis un délit, malheureusement, nous regrettons que on on ne constate pas les moins nécessaires afin de respecter ses présidentielle en effet dans le projet de loi de finances 2018, 14500 éloignements forcés sont budgétés, c'est moins que sous le prix, le mandat du président Hollande. qui reconnaît que connaît l'Europe, Union européenne, dans le contexte de programme de relocalisation européens qui verront la France attire des demandeurs d'asile supplémentaires, il est évident que ce budget demeure très insuffisant aussi le groupe des indépendants ne votera pas les crédits de la mission Immigration, asile et intégration du projet de loi finance Milicevic je vous remercie.

Monsieur le président Monsieur Miss mais, chers collègues, à 3 minutes, le Front national à 3 minutes pour porter la voix de la majorité de nos compatriotes qui, malgré une propagande tout azimut considère non seulement l'immigration. Que non seulement l'immigration n'est pas une chance pour la France, mais qu'elle constitue une menace pour sa sécurité, son identité, sa prospérité, monsieur le ministre, votre politique de reconduite à la frontière qui n'existe plus, est une mauvaise plaisanterie vous consacrer un milliard 100 millions d'euros à votre programme 303 Immigration et asile soit un budget en hausse de 28 sur ce budget une part dérisoire est alloués à la lutte contre l'immigration irrégulière 82 millions, soit une baisse de 7 pourcent par rapport à l'année dernière le budget concernant l'allocation pour les demandeurs d'asile, relève de la provocation, s'il s'établit désormais à 318 millions d'euros au 31 juillet 2010 à 80000 étrangers, bénéficier de cette aide nos agriculteurs, nos artisans, nos jeunes et beaucoup de nos retraités aimeraient en percevoir autant un chiffre seulement 18 pourcent des expulsions ordonnées sont exécutées en 2017 ce 178000 personnes expulsables, qui sont restés sur le territoire et vous en profitez pour diminuer de plus de 3 millions les crédits destinés aux expulsions, nous devons faire face à une explosion des demandes d'asile vous le soulignez vous-même plus 17 pourcent entre 2016 et 2017 et les prévisions pour les années qui viennent sont alarmantes : il y a aujourd'hui 90000 demandeurs d'asile, soit une augmentation de 62 pourcent pour 2010 et 2017, parmi eux, 45 pourcent des gens ont fait une demande dans un ou plusieurs États-membres de l'Union européenne, via la procédure de Dublin et qui veut que les 500000 déboutés du droit d'asile en Allemagne peuvent le demander à nouveau à la France, votre obsession masochiste de protéger le lointain, y compris quand il est clandestins au détriment de de son prochain prend ici toute son ampleur au cours des 5 dernières années, plus d'un 1000000 de titres de séjour ont été délivrés, 151000 clandestins ont été régularisés et 120000 étrangers sont devenus français, l'Imprimerie nationale tourne après Régine cette mission Immigration et asile démontre avec quelle détermination, Emmanuel Macron et son gouvernement s'emploie non seulement déconstruire la France mais également à déconstruire l'unité du peuple français, monsieur le ministre, en parfaite application des consignes reçues par l'Élysée, loin d'endiguer la déferlante migratoire vous l'amplifier alors en parfaite application du souhait de nos compatriotes, j'affirme ici, il est urgent de sortir des accords de Schengen de rétablir de contrôler nos frontières de restreindre considérablement le droit d'asile n'trop souvent que le cache-sexe d'une immigration économique, son ampleur est telle qu'elle développe un communautarisme qui sonne le glas de l'intégration que vous essayez de masqués par le voile de la sémantique du vivre-ensemble quant au coût sécuritaire, il faut en effet chaque jour sinon dans les jeux dans les dans la presse, du moins dans les commissariats et sur les écrans du monde entier, lorsque les réfugiés se révèlent être des terroristes islamistes, il faut regarder la vérité en face, elle vous rendra libre, mes chers collègues, si l'immigration est une chance pour le grand patronat pour les résiduel syndicats pour les idiots utiles des partis de gauche pour les couloirs des partis de droite immigration constituent un dirigeant Fordo et un danger pour conclure en national et pour conclure, Libérez-vous Monsieur le Ministre,

La parole est maintenant à monsieur Guillaume Arnell pour le groupe Les RDA RDSE pour 6 minutes.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État. Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le 12 juillet dernier, le gouvernement a rendu public son plan d'action destiné à garantir le droit d'asile et à me maîtriser les flux migratoires, il est indéniable que les priorités fixées au sein de la mission Immigration, asile et intégration correspondent à ces engagements, notamment le 2ème objectif visant à redonner sa pleine portée au droit d'asile. De fait, les efforts budgétaires en faveur de l'amélioration de l'exercice de ce droit sont importants, l'action de garanties du droit d'asile qui concentre déjà dans l'exercice précédent, 67 pourcent des crédits de la mission. En trouve désormais 71 pourcent à ceci s'ajoute également les crédits de l'action Accompagnement des réfugiés au sein du second programme intégration et accès à la nationalité française, qui double presque cette année, il faut en autre ajouter les crédits ventilés dans tout le budget qui ou indirectement à la réalisation de cette mission, je pense notamment au moyen des préfectures, mais surtout à ceux attribués à la Cour nationale du droit d'asile rattaché au Conseil d'État et aux juridictions administratives au sein de la mission, conseil et contrôle de l'État, ces efforts budgétaires devraient permettent de réduire les délais d'examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié ou de protection devant l'Oprah aider recoupent Horter devant la CNDA, il s'agit d'une première étape dont nul ne peut contester la nécessité la priorité actuelle hé bien agir face à une situation d'urgence découlant de la déstabilisation de pays de la rive sud de la Méditerranée qui agissait jusqu'alors comme B régulateurs et la mise en oeuvre du règlement Dublin III, adopté en 2013 ce règlement pose le principe suivant le pays dans lequel a été formulé la demande d'asile et celui qui est chargé de son instruction et de la décision finale, il faudra ensuite poser se poser la question d'un rééquilibrage entre la force reconnue au droit d'asile et celle du titre de séjour un parcours d'intégration dans la perspective d'acquérir la nationalité française pour des raisons aisément compréhensibles, de nombreuses personnes en situation d'immigration illégale sont tentés de solliciter le droit d'asile ou la protection subsidiaire auprès de l'Ofpra afin de régulariser leur présence sur le sol français et inversement, les parcours juridique tend donc à s'entremêler une confusion entre immigration et asile se manifeste également de façon de plus en plus récurrent dans les médias sur le plan administratif, ce phénomène a pour conséquence le développement d'une administration et d'une juridiction propre à l'asile et animée principalement par 2 jeunes diplômés recrutés comme agents contractuels, la détresse des demandeurs, ce double donc parfois de l'inexpérience de ses agents qui leur font face à terme un rapprochement des services examinant les demandes de types de séjours, d'asile et de protection subsidiaire pourraient donc être envisagées, permettant ainsi à mieux orienter de mieux orienter les personnes vers les procédures correspondant à leur situation réelle tout en réduisant les coûts d'examens et le recours juridictionnel, il faut redonner à la ville son sens 1er, telle que définie par l'article 120 de la Constitution de 1793 qui disposait, le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour cause de la liberté et il le refuse aux tyrans, une meilleure distinction entre la ville et l'immigration passe également par la revalorisation du parcours d'intégration proposé aux personnes immigrés arrivant en France de ce point de vue, le lancement d'une mission parlementaire sur la refonte de la politique d'intégration par le ministère de l'Intérieur est une bonne nouvelle, comme les États à l'échelle européenne les territoire français ne sont pas exposées de la même manière au phénomène migratoire les zones frontalières et particulièrement les îles françaises les plus éloignés, ce sont les premières impactées mon territoire Saint-Martin Martin est un cas d'école mais n'est pas le seul, je pense aussi à mal à Guyane et à Mayotte, mais est le seul qui cumule à la fois les 2 facteurs cela justifierait que le député, or il y attacher nous rendre visite dans le cas de familles mission sur la refonte de la politique d'intégration, selon une récente une récente évaluation de la direction générale de l'outre-mer, pourcent des habitants de l'île sont nés à l'étranger, principalement des ressortissants de l'île d'Hispaniola lundi les mains existence d'une frontière étatique physique sur l'île, tente également à favoriser l'installation de populations immigrée dont la précarité c'est coup avec les désastres causés par l'ouragan Irma, une révision des modalités de contrôle s'impose, dont il devient l'autre extrêmement urgent de repenser les différents parcours d'intégration républicaine aussi, il faut adapter à chaque âge de vie afin de donner les moyens à chacun à chacun la faculté de s'insérer dans la société française, non seulement comme des agents économiques, mais également comme d'authentiques citoyens, cette question n'est pas abordé avec la même manière, genre termine Monsieur le Président, dans les territoires français qui lutte conte le dépeuplement et la désertification administrative en définitive et en conclusion, l'immigration n'apparaît plus comme un phénomène épisodique mais durable qui se renforcera probablement avec l'immigration climatiques, la France, bien que n'ayant plus la capacité d'agir d'accueillir toute la détresse du monde doit continuer à en prendre sa part, en veillant à ne pas mettre en péril les équilibres, sociaux, sociétaux et territoriaux, le groupe RDSE conscient des efforts budgétaires consentis en cette période portera un regard bienveillant et apportera son soutien au gouvernement. Monsieur Bernard Fournier pour le groupe, les républicains pour 4 minutes. Monsieur Alain Dufaut d'abord 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre d'État m'messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ne disposant que les 4 millions d'interventions, je souhaiterais focaliser mon propos sur un seul axe de la mission, la maîtrise des Fumiya migratoire et plus spécialement la lutte contre l'immigration irrégulière. Notre politique migratoire notre droit d'asile et nos efforts pour favoriser une bonne intégration des personnes immigrées en situation régulière, ne pas voter à être pleinement efficace que si en même temps, passez-moi l'instruction nous luttons sans ambiguïté contre l'immigration irrégulière que la baisse notoire des crédits destinés à ce poste, ça a été dit, moins 7,1 pourcent en crédits de paiement est en totale contradiction avec la volonté affichée du gouvernement oui cette liste Lutte est incontestablement le parent pauvre de cette émission, Monsieur le Ministre, avec seulement 6 pourcent des crédits total de la mission alors en entendant dans le détail de ces crédits qui atteindront 82,82 millions d'euros en 2018 41 millions virgule 4 euros permettront le financement ça a été dit aussi des 27 centres la rétention administrative 23 en métropole et 4 en outre-mer, pour un total de 1000 700 80 places, plus les 4 locaux de rétention administrative de la zone d'attente des personnes en instance de départ à l'aéroport de Roissy, enfin 32 millions seront consacrés aux frais d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, hé bien tous ces montants je répète sont manifestement insuffisants par rapport à la réalité des besoins, un exemple : les crédits de frais de loyer manque à 30 millions d'euros seront en baisse de 10 pourcent par rapport à 2017 alors que les correctifs que vous souhaitez apporter à la sous-occupation chronique des centres de rétention administrative, les et et aussi le fait que les rétention peuvent désormais durer jusqu'à 45 jours vont automatiquement augmenter le nombre des candidats au retour. Une baisse des crédits à destination de CRA est en effet particulièrement dommageable dans un contexte de crise migratoire qui inévitablement conduire à une augmentation considérable des placements en rétention. Comme le dit fort justement François-Noël Buffet dans son rapport pour le seul 1er semestre de 2017 l'augmentation du taux d'occupation étaient déjà de plus 66 Actuellement le étrangers en situation irrégulière sur le sol français est certainement supérieur à 400000 personnes, il suffit de constater, on n'a pas les chiffres que le nombre des bénéficiaires de l'AME l'aide médicale d'État et de 311310 personnes à la fin de l'année 2016, soit plus 49 pourcent par rapport au 31 décembre 2011 pour pouvoir enfin imaginer leur nombre réel l'éloignement des étrangers en situation régulière, devrait donc être une vraie priorité si on veut trouver une vraie crédibilité dans toute une politique d'immigration. Faut-il seulement rappeler que 92000 mesures d'éloignement été prononcée en 2016 et seuls 18 pourcent d'entre elles ont réellement été exécutés, soit par un éloignement forcé aidés ou encore spontanée. Il faut donc se donner les moyens et renégocier avec les pays d'origine, en particulier le Maroc, la Tunisie ou le Pakistan, afin d'améliorer ses retours, la tâche s'annonce difficile, c'est vrai, mais les laissez-passer consulaires devrait aboutir à des résultats nettement supérieurs, voilà, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce qu'il faudrait faire, mais les chiffres annoncés dans cette émission démontre que votre gouvernement sera en 2017 dans l'incapacité de tenir ses engagements en matière d'éloignement forcé et nous sommes dans mon groupe pleinement d'accord avec l'avis défavorable de la commission des lois, face à l'adoption des crédits qui nous sont proposées aujourd'hui dans ce projet de loi des finances pour 2018. Merci, la parole est donc maintenant à Monsieur Bernard Fournier pour le groupe, les républicains pour 4 minutes. Monsieur président Monsieur le ministre d'État, mais chers collègues monsieur le ministre, le mot qui m'est venu à l'esprit après avoir examiné les crédits relatifs à cette mission et partagée, partagée parce qu'il est indéniable que les crédits de cette mission augmente fortement par rapport à 2017 on est fort et donc réalisé par le gouvernement, entre autres, pour accueillir dans de meilleures conditions, les demandeurs d'asile pour créer plus de places d'hébergement ou mener une politique d'intégration plus volontariste, je suis parfaitement d'accord avec l'intention du président de la République de réduire les délais de traitement des demandeurs d'asile de 12 à 6 mois mais partager aussi car la politique d'immigration n'est pas retrouve gouvernement reste assez fou et nous ne pouvons que constater un décalage entre discours et réalité l'immigration regroupe énormément de facteurs, dont tout le monde connaît la sensibilité dans notre pays et en Europe, rien n'est simple dans ce domaine et l'équilibre est souvent très fragile entre humanité et réalisme, les réponses apportées à ces questions qui concernent des femmes et des hommes qui fuient des situations humaines parfois extrêmement difficile dans leur pays d'origine sont complexes, nos politiques d'intégration depuis plus de 40 ans, ce sont souvent traduite par des échecs, et ça ne s'est pas amélioré ces dernières années, car la pression migratoire est extrêmement forte, certaines années, notamment en 2015, ce problème est en haut, de plus en plus aiguë, car nous devons intégrer des gens qui viennent de plus en plus loin et, pour certains qui ne partagent aucune de nos valeurs culturelles ainsi, je considère que ce budget pose de nombreuses questions auxquelles le gouvernement ne répond pas vraiment François-Noël Buffet a relevé dans son rapport que pour la seule année 2016 plus de 75000 personnes se sont maintenus sur le territoire français, malgré la mesure d'éloignement prononcées à l'heure, on en compte, seuls 18 pourcent des mesures d'éloignement sont exécutés, il est bien évidemment trop tôt pour juger certaines politiques du président, mais nous regardons avec attention ses engagements, notamment sur la mise en oeuvre d'une vraie politique de reconduite aux frontières. Sur laquelle il a beaucoup insisté, en août, je constate avec regret dans ce budget que les crédits consacrés à l'immigration irrégulière, baisse de 7 pourcent je déplore aussi la suppression de l'aide aux communes au-delà du territoire métropolitain, la Guyane et Mayotte sont confrontées à une explosion de l'immigration clandestine qu'il est bien difficile de juguler et qui pose de nombreuses difficultés d'énormes difficultés au plus populations locales au niveau européen certains pays comme l'Italie, la Grèce ou encore Chypre se sentent souvent bien seul face aux réfugiés arrivant sur leurs côtes, alors que de l'autre côté, le groupe de Visegrad refusent ouvertement les politiques migratoires de solidarité définie par Bruxelles, certains chiffres résument tout sur les difficultés d'avoir une politique efficace en matière d'immigration est asile lorsque vous apprenez que seuls 23 pourcent des franchissements irréguliers d'une frontière extérieure de l'Union, font l'objet d'un prélèvement d'empreintes digitales, que fera la France que fera l'Europe si demain l'accord qui a été conclu avec la Turquie, en mars 2016 et remis en question parce que Monsieur Erdogan décide de faire pression sur les pays de l'Union européenne, en conséquence, mes chers collègues, même si ce budget est en augmentation, je ne peux que trouver en décalage avec la réalité, je trouve que beaucoup de faits de chiffres sont sous-estimés, ou pas du tout pris en compte, ainsi, je doute de l'efficacité de ses politiques et c'est pourquoi monsieur le ministre, je voterai contre ce budget, je vous remercie. Eh bien maintenant la parole. Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur pour 10 minutes. Monsieur le président, monsieur le rapporteur spécial de la commission des finances, monsieur le rapporteur pour avis de la commission des lois, mesdames et messieurs les sénateurs,

leur occasion et surtout pour moi l'occasion de vous indiquer leur examen pardon et pour moi l'occasion de vous indiquer quelle est notre politique en ce domaine et comment nous entendons la mettre en oeuvre, je veux d'abord donner quelques chiffres parce que quelques fois des chiffres inexacts sont donnés comme vous le savez, l'Europe a été affronter depuis 2014 à une crise migratoire son précédent, c'est évidemment le fait de personnes fuyant le théâtre de guerre irako-syrien ou les pays où l'insécurité est forte, mais au-delà de ces réfugiés, on observe aussi à un flux grandissant de migrants à caractère économique venant de pays considérés comme sûrs, après avoir connu des plus hauts depuis 2014. Avec un 1000000 200 90 1000 demandes d'asile en 2016, 2017 a marqué une inflexion en Europe puisque, sur les 7 premières moi, nous sommes à 410000 personnes, la tendance n'est cependant pas la même en France en 2016 on avait enregistré 85726 demandes d'asile en 2017, sur les 6 premiers mois, nous en avons enregistré Swat cette hausse de la demande d'asile provient de plusieurs facteurs, comme vous le savez, l'Italie avait dû faire face à une arrivée croissante de migrants de Libye 180000 en 2016 encore 91000 2. Depuis le début de cette année, même si une rupture, a pu être constaté à partir de juillet : moins 56 pourcent mais surtout en août, moins 70 Mais on considère qu'aujourd'hui il y a en Italie à peu près 180000 personnes qui sont dans les différents sans beaucoup de ce. Qui sont arrivés dans ce pays cherche à passer la frontière française, c'est par exemple 1000 personnes qui sont interceptés chaque semaine à la frontière de Vintimille et une centaine dans Les Hautes-Alpes, d'autre part, une autoroute de migration est en train de s'ouvrir, passant par l'Espagne 25000 arrivées depuis le début de l'année, soit une hausse de plus de 150 le 3ème facteur est due à ce. Qui parmi les migrants ont été déboutés, les droits d'asile dans les autres pays européens pour ne prendre que l'exemple de l'Allemagne, vous savez qu'il y a eu 750000 demandeurs d'asile en 2015 475000 en 2016 mais aujourd'hui environ 300000 ont été déboutés et seulement 80000 ont été reconduits, si nous ne prenions pas un certain nombre de mesures, nous serions donc confrontés à une situation qui deviendrait insupportable face à ces défis, la position du gouvernement est clair : tous ceux qui sont réfugiés des théâtres de guerre ou victimes de persécutions politiques, religieuses, ethniques dans leur pays, ont droit à un droit imprescriptible à l'Asie, par contre évidemment la dynamique migratoire que l'on observe résulte de migration à caractère économique organisé, souvent par des réseaux de passeurs internationaux et à laquelle nous entendons mettre fin pour cela, le gouvernement veut agir dans. Plusieurs directions, vous savez que, par exemple, une proposition de loi relative à la procédure applicable au transfert du blanc sera examinée jeudi à l'Assemblée nationale, le gouvernement présentera par ailleurs. Un projet de loi qui visera à réduire les délais de l'examen de la demande d'asile à 6 mois, cela nous permettra de dire si effectivement a droit à l'asile et qu'il n'y a pas droit et doit être éloignée pour ce qui concerne ce que nous faisons aujourd'hui nous essayons de faire d'abord un accord avec les pays d'arriver, qui sont considérés comme sûrs, je me suis rendu avec le président de la République à Abidjan, et nous avons discuté avec l'ensemble des dirigeants de ces pays, de manière à pouvoir maîtriser une immigration économique irrégulière qui souvent les mais eux-mêmes en difficulté, cela ne premières direction d'actions pour cela, nous visons le renfort. Seulement les capacités des forces de sécurité local pour lutter contre les réseaux de passeurs et assurer le traitement judiciaire de cette. Criminalité, deuxièmement, nous visons la facilitation de la réadmission, c'est en effet en facilitant les réadmissions que l'on parviendra à dissuader un certain nombre de départs en 2016, 40 pourcent les mesures d'éloignement prononcées contre concernaient des nationalités couvertes par un accord de réadmission bilatéral ou européen avec nos partenaires européens, je souhaite donc que nous renforcions encore cette politique de réadmission en l'Alliance il besoin était à notre politique de visas enfin nous développons notre soutien à l'enrichissement de l'état civil par des éléments de biométrie, ce qui permettra notamment de disposer de manière certaine, d'informations sur la nationalité ou l'âge des migrants et donc de pouvoir obtenir des laissez-passer consulaires, la lutte contre l'immigration irrégulière efficace repose aussi sur une politique d'éloignement crédible et je voudrais souligner qu'en matière d'éloignement, nous enregistrons déjà les premiers résultats depuis le début de l'année 2017 l'ensemble des éloignements a augmenté de 8 pourcent 15098 à ce jour, et notamment les éloignements forcés

tout d'abord, qui a augmenté de près de 7 pourcent et enfin la mise en oeuvre des procédures de transfert prévu par le dispositif du blanc qui ont augmenté de 114 depuis le début de l'année, soit 2166 transfert en 2018, cette politique se poursuivra et je veux ici préciser que ce projet de budget comprend tous les moyens nécessaires à sa conduite, comme je l'ai déjà indiqué, nous créerons les places nécessaires en centre de rétention administrative, comme je l'ai déjà dit également, ce n'est qu'au petit comment que les crédits consacrés à cette politique sont affichés en diminution dans les bleus budgétaires, ils vous ont été communiqués en effet la fermeture, les camps de Calais de Grande-Synthe, qui étaient pris en charge par les crédits de cette mission entraîne de moindres dépenses à structure constante, les moyens de la lutte contre l'immigration irrégulière augmente donc de plus 4 millions d'euros dans ce projet de loi de finances, soit une hausse de plus de 5 enfin, et c'est là le dernier des aspects de notre politique parce que nous voulons une politique équilibrée, nous souhaitons renforcer notre politique d'intégration, car il s'agit d'un enjeu de 1er plan pour notre cohésion sociale que d'accompagner les étrangers à qui nous accordons le droit d'asile ou de séjour dans leurs apprentissages linguistiques leur formation civique et leur insertion professionnelle, nous nous appuierons dans ce domaine sur les conclusions des travaux, ils sont actuellement conduits par monsieur Aurélien taché, député du Val Oise comment cette politique est-elle traduite dans le projet de loi de finances, vous l'avez constaté parce que la dynamique constatée de flux migratoires demeure soutenue mécaniquement, cela conduit à une hausse des dépenses de la mission, comme vous le savez la philosophie du gouvernement et de présenter un budget sincère, c'est-à-dire un budget qui comprend des crédits à hauteur des dépenses qui sont attendus, nous avons donc souhaité budgétisé à leur juste niveau les dépenses qui concernent l'Asie nous avons donc financer la création pour 2018 de 4000 places pour l'hébergement des demandeurs d'asile, 1500 places en Cada, 2500 en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, le plan gouvernemental prévoit également de la refonte de nos politiques d'intégration, la création de 3000 places de centre provisoire des bergers voilà Mesdames et messieurs les sénateurs, nous voulons une politique équilibrée, où il y a effectivement à l'asile, non aux passeurs qui organisent les trafics et font mourir des dizaines de milliers de jeunes sur les routes du Sahel ou bien en traversant la Méditerranée. Merci, Monsieur le Ministre, nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Immigration, asile et intégration figurant à l'État B.. Et j'appelle pour son amendement 380. Monsieur à le présenter. Eh oui, la forme supporter encore quelques quelques instants encore 3 ans au moins, monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le présente en ordonnant vise à doubler les crédits consacrés à l'action 03 du programme 303 lutte contre l'immigration irrégulière, l'indicateur 3 1 de l'objectif numéro 3 du programme 303 montre en effet que le le taux des retours forcés exécuter stagne désespérément en-dessous de 50 en contrepartie les crédits destinés à l'action numéro 11 du programme CIV : accueil des étrangers primo-arrivants serait diminuer à due concurrence en effet une partie importante de ces crédits est consacrée au regroupement familial, je me demande ce qu'on peut encore regroupés parce que cela fait 30 ans quand même que ce regroupement a lieu, lequel a donc largement contribué à la déferlante migratoire et qui n'a plus sa raison d'être: le budget 2018 destiné aux expulsions ne permet de financer que 14500 l'éloignement, donc moins que sous François Hollande il fallait quand même le faire, qui lui a avait procédé à quelque 15000 en 2014, ce budget diminue, même de 3 1000000 300000 euros entre 2018 et 2017 quelle incohérence révélatrice, alors que vous même, Monsieur le Ministre vous draper de bonnes intentions, vous interpelliez il y a quelques jours, les services de l'État à travers ses préfets pour leur demander des résultats rapides et vous leur donnez moins de moyens pour ce par ce budget, vous n'êtes plus à une contradiction près, pour expliquer le faible nombre d'OQTF d'obligation de quitter le territoire français suivi d'effet, le rapport de notre commission avance que la réduction de 5 à 2 jours du délai de rétention avant l'intervention du juge des libertés a empêché l'administration de constituer des dossiers étayés, avec 19,3 pourcent des étrangers placés en rétention ont été libérés après 48 heures, contre 6,35 pourcent en 2016, d'autre part, les pays d'origine de ne délivre plus pas suffisamment de laissez-passer consulaire, seuls 46 pourcent ont été délivrés à temps, quand elles ne sont pas le clandestin et relâché, certains pays comme le Maroc, la Tunisie ou le Pakistan refuse l'éloignement groupés, nous sommes donc condamnée par les pays d'où sont originaires ces clandestins, une véritable double peine, il serait souhaitable, Monsieur le Ministre, que la France, un peu du poing sur la table et conditionne, par exemple, ces échanges commerciaux à l'acceptation des expulsions groupées, il y a la délivrance des laissez-passer consulaires en temps et en heure. L'avis de la commission. effectivement nécessaire d'avoir un véritable plan Marshall sur l'intégration et cet amendement vise à diminuer les mesures d'intégration pour les étrangers en situation régulière, donc la commission a donné un avis défavorable. Il y a un an, Monsieur le Ministre votre avis. Comme je l'indiquais, nous entendrons, avoir une politique équilibrée qui vise à faire en sorte que les étrangers en situation régulière, puissent s'insérer dans notre société et donc bénéficier de mesures nouvelles, c'est cela notre politique équilibrée : d'un côté, accueillir ceux qui ont droit à l'asile, de l'autre côté éloigner rapidement ceux qui n'y ont pas droit. nous allons donc passer au vote sur cet amendement avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, cet amendement est rejeté, nouvel amendement de monsieur 380. Merci monsieur le président, Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues par cet amendement, je voudrais revenir sur le scandale des centres de rétention administrative dans lesquels sont placés les étrangers qui n'ont donc pas le droit de séjourner en France, 44000 personnes y ont été placés en 2016 dont 22900 en métropole, plus de 50 pourcent d'entre elles ne sont pas expulsés, car le juge annule l'obligation de quitter le territoire où l'administration n'a pu organiser l'expulsion dans les délais, le taux d'occupation des CRA est de 60,9 pourcent en France depuis l'attentat de Marseille, le taux d'occupation des CRA approche les 100 pourcent rappelons ce drame de Marseille 7 attentats islamistes perpétrés par un clandestin un délinquant multirécidiviste pour lequel on n'a pas su trouver une place en CRA et qui a été relâché dans la nature, la vie de 2 jeunes filles a été volé fauchées sur l'autel de l'incurie des pouvoirs publics, comment se fait-il que dans ce contexte, l'accent ne soit pas mis sur la construction de nouvelles places de Serra, comment on peut imaginer que moins de 1800 places sont disponibles dans notre pays, comparé aux 100000 obligation de quitter le territoire français, c'est totalement dérisoire la réponse au drame de Marseille c'est une baisse de 7 millions du budget alloué à la Mission de lutte contre l'immigration clandestine, qui comprend le fonctionnement des CRA et les mesures d'éloignement des clandestins, les familles et les Français apprécieront. Alors, là encore, hein, je ne reviens pas ce que je dis sur l'ensemble de crédits de la mission, mais la commission a considéré que le taux d'occupation des des des CPH étaient déjà extrêmement élevé, donc on a, nous avons émis un avis défavorable, c'est sur cet amendement.

Qui est contre qui s'abstient l'amendement est rejeté, nouvel amendement 382 Monsieur Ravier, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le présent amendement vise à retrancher

intitulé : lutte contre l'immigration irrégulière à due concurrence en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, l'objectif de cet amendement et de voir et de revoir pardon à la baisse les montants alloués aux programmes d'alphabétisation et d'accès au droit à l'insertion professionnelle et à l'emploi des migrants pour renforcer le volume des dépenses relatives à l'éloignement des migrants en situation irrégulière, je vous remercie. Votre avis, monsieur le rapporteur. Là encore, ça concerne les biens intégration et les formations linguistiques, donc on peut pas souhaité diminuer les formations linguistiques et l'apprentissage de nos valeurs républicaines, donc, là encore, la commission a émis un avis défavorable. Votre avis, Monsieur le Ministre. Favorable 2 avis défavorables à qui est pour. Qui est contre qui s'abstient l'amendement est rejeté, nouvel amendement 382 Monsieur Ravier, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le présent amendement vise à retrancher 5 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 5 millions d'euros de crédits de paiement à l'action numéro 16 du programme 104 intitulée accompagnement du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants pour les affecter à l'action, numéro 3 du programme 303 intitulé : lutte contre l'immigration irrégulière, l'objectif est d'affecter 5 millions d'euros supplémentaires aux dépenses d'investissement immobiliers pour l'extension des centres de rétention administrative existants et la création de nouveaux centres de rétention administrative, dans le Calvados, dans le Pas-de-Calais et dans les Hautes-Alpes, merci. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur, alors ce n'est. Pas en dégradant, enfin en dégradant les conditions d'accueil des étrangers en situation régulière, qu'on va régler le problème des étrangers en situation irrégulière, donc la commission a émis un avis défavorable. Vide de du gouvernement. Oui, ces foyers, ces vieux travailleurs immigrés les chibanis, comme on les appelle, qui ont construit la France des 30 glorieuses, ne pas leur donner aujourd'hui un accueil digne serait totalement inhumain, le gouvernement est défavorable. 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient l'amendement est rejeté, 406 rectifier bis madame de La Gontrie, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre d'État, cet amendement a pour objet de renforcer les moyens des associations avec lesquelles l'État contractualisé pour intervenir dans les lieux de de rétention puisque vous le savez la loi ces à impose au gouvernement de contractualiser avec des structures qui apportent aux personnes retenues, la connaissance de leurs droits tout à l'heure, vous l'avez peu évoqué dans votre propos liminaire, mais je suis persuadé que quelle que soit la fermeté dont vous faites preuve ce point est important pour vous, vous avez pourtant prévu simplement 20000 euros de plus qu'au budget de l'an dernier 6 millions 30 30 l'an dernier 6 1000032 cette année, vous avez adressé à l'ensemble des préfets une circulaire le 20 novembre de 14 pages les enjoignant à la plus grande sévérité, vous avez annoncé l'ouverture de nouvelles places en centre de rétention, vous avez annoncé vouloir doubler la durée maximum de rétention possible pour un étranger, comment allez-vous, du coup, pouvoir permettre à ces personnes retenues l'accès à leurs droits et à l'information, avec 20000 euros de plus simplement que l'an dernier, donc cet amendement à cet objet de renforcer et j'apprécierais pour le coup que la commission des finances, et son rapporteur émettent un avis qui soit un avis sur le fond de l'amendement et pas seulement sur son gage, si ce n'est que, à défaut, je me permettrai d'y répondre. Merci l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Si le fond effectivement peut être positif, voilà, dans la forme, vous diminuez également les crédits destinés à la formation linguistique et civique des étrangers primo-arrivants, donc évidemment on peut pas, on considère que la formation linguistique et civique et XM, c'est absolument nécessaire, donc là, nous sommes effectivement aussi sur un un avis défavorable de la commission. Monsieur le ministre, votre avis. Défavorable, je rappelle, je n'ai pas pu le mentionner tout à l'heure que pour mener la politique que nous souhaitons 150 emplois seront créés dans les préfectures, au sein des services chargés des étrangers de l'asile que 15 TP seront créés à l'Ofpra et les moyens de cet opérateur renforcer le 5 millions d'euros, enfin pour l'ce sera une augmentation de 18 millions d'euros de ses moyens de fonctionnement et 35 ETP, nous nous donnons les moyens de mener la politique que nous souhaitons. Donc 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre.

avant l'expiration du délai limite je mets aux voix les crédits de la mission qui est pour. Qui est contre. C'est pas adopté les crédits sont rejetés, donc la mission. J'appelle en discussion : les articles 56. Et 57 et 57 bis et les amendements qui sont rattachés, article 56 amendements Monsieur Ravier 377.

ne règle rien à Mayotte, pardon, tant que les règles en matière migratoire ne changeront ne changeront pas radicalement pour rappel, le contrat d'intégration républicaine qui constitue le socle du dispositif d'intégration des étrangers primo-arrivants comprend notamment l'obligation pour tous les signataires de suivre une formation civique et pour ceux dont le niveau de langue est inférieur à 1 une formation en langue française, la belle affaire par cet amendement, nous ne nous ne signifie ont pas que les étrangers viendra Mayotte pour pour prendre des cours de français, nous voulons dire non à toutes ces dépenses endémique que nous consacrons et que nous sacrifions à une immigration incontrôlée, qui par sa proportions démesurées empêcher condamne même tout espoir d'intégration, bien évidemment, nous sommes favorables à l'intégration, mais pour que l'intégration est un avenir, il faut stopper Net cette politique de submersion migratoire dont Mayotte et l'emblème, nous devons totalement refondre notre code de la nationalité et rétablir le droit du sang, pour en finir avec l'acquisition automatique de la nationalité française à une personne parce que nés en France et qui permet aussi aux parents étrangers et même clandestins de demeurer sur notre sol je me permets de rappeler, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la lucidité qui avait frappé en 2005, alors le ministre français de l'outre-mer, un certain François Baroin et qui revenait de Mayotte, il avait appelé de ses voeux à des mesures radicales nécessaires selon lui pour lutter contre l'immigration illégale l'dans les îles françaises pour pour y parvenir, il se déclarait prêt lui François Baroin à remettre en cause le droit du sol depuis rien en changer, si ce n'est en pire, nous devons renvoyer chez eux les primo-arrivants et nous devons organiser le retour de de déprime riverains dans leur pays d'origine, organiser le retour des bateaux qui transportaient ces clandestins tout en les interceptant bien sûr et tous nos efforts doivent porter sur les filières des passeurs qui exploitent ces migrants. Monsieur le rapporteur, votre avis non il y a aussi une discussion commune, vous allez me donner votre avis non pas maintenant Monsieur après l'amendement 276 c'est votre amendement que vous présentez.

visait à soigner l'intégration en laissant le temps au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réellement matérialisait intégration et donner des cours d'intégration civique donc aux migrants et donc je vous propose d'être contre le 1er rapidement et pour bien sûr pour celui qui a défendu devant la commission. Donc Monsieur Mini sur les 2 amendements. Qui effectivement sont pas les mêmes. Alors le gouvernement sera défavorable aux 2 amendements donc le la, il devait y avoir donc une mise en oeuvre progressive du CIR à Mayotte, à compter du 1er janvier 2018, le gouvernement a souhaité reporter cette date au 1er janvier 2020, compte tenu des caractéristiques et contraintes particulières de Lille nous avons en effet un certain nombre de difficultés à pouvoir aujourd'hui ouvrir ses cendres. et vous donnez votre avis sur celui de Monsieur rend les 2 défavorable, donc. Sur l'amendement de Monsieur Ravier : avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

La commission est pour le gouvernement et compte qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il était adopté. Nous passons au vote de l'article 56 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il a été adopté.

Merci monsieur le président, Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le budget concernant l'allocation pour les demandeurs d'asile est extravagant désormais dans votre projet à 318 millions d'euros, cette aide dont bénéficient les demandeurs d'asile pendant toute la durée de la procédure d'instruction de leur demande varie autour de 350 euros mensuels si mais bénéficie pas d'une solution d'hébergement provisoire, c'est égal, voire supérieur à ce que gagnent nombres de nos agriculteurs ou éleveurs, pour ne citer qu'eux au 31 juillet 2017 ans, j'ai déjà pu l'exprimer 80000 ménages bénéficiaient de la notre politique d'asile coûte près de 2 milliards d'euros au budget de l'État, une somme aussi faramineuse démontre que l'asile a été complètement dévoyé et qui constitue désormais une filière de l'immigration clandestine,

je rappelle que l'instruction des demandes d'asile dure en moyenne entre 12 et 14 mois durant lesquels les 75 pourcent de déboutés du droit d'asile vont toucher leur leur allocation mensuelle, au total, le coût de l'asile atteint 13724 euros par demandeur, le budget de l'asile doit voir ses crédits réduits. Une telle dérapage n'est pas tolérable. Parmi toutes ces cette cohorte de migrants. En pleine forme physique. physique. Seul, sans enfant, et manifestement non accompagnés de leurs épouses combien fuient véritablement la guerre combien en réalité de migrants économiques qui souhaitent rejoindre l'eldorado français Dorado qui n'existe plus, si tant est qu'il est exister un jour, il y a 10 ans, les vérité, toute la vérité des attentats dramatiques de ces dernières années ont prouvé que des terroristes s'étaient infiltrés parmi ces réfugiés, cela veut-il dire que nous jetons l'amalgame sur toutes ces populations qui quittent leur pays bien évidemment que non, mais pour nous, mesdames et messieurs, mes chers collègues, hé bien, la sécurité des Français reste la priorité.

que la performance globale du système, ses doigts doit être prioritaire et là des réduire à 3 jours francs, ça paraît pas réaliste donc la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Monsieur le Ministre votre avis

Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté sur l'article 57 bis, il y a une demande de parole sur article de Monsieur Jean-Yves Leconte à vous la parole. le le le le président de de de sujets d'abord, je me permets d'intervenir parce que je, je vous avez demandé la parole pour explication de vote sur l'article précédent sur finalement la la manière dont la commission des finances à considérer qu'un certain nombre des amendements qui étaient déposées Teddy recevable, on constate que j'ai, j'avais déposé des amendements visant à rendre effectif le droit au travail pour les demandeurs d'asile qui n'ont pas vu leur demande encore complètement étudié après 9 mois, c'est totalement conforme à la directive européenne et nous sommes aujourd'hui hors des clous en ce qui concerne ce point donné droit au travail, c'est aussi permettre à la personne si elle travaille de ne pas percevoir les aides auxquelles elle a droit, dans le cas contraire, donc ça a un effet budgétaire et pourtant, la commission des finances, a considéré que mes articles mes à moment pas recevable alors que l'article 34 de la LOLF considère que on peut proposer des amendements qui comporte des dispositions affectant directement des dépenses budgétaires de l'année, je regrette donc cette interprétation excessive de la LOLF qui ne nous a pas permis de travail de, de, amendements alors maintenant sur l'article 57 bis je : je suis un peu inquiet de cet article et je voulais demander à monsieur le ministre, un certain nombre de précisions parce que je sais que les rédactions qui sont dans l'article 57 bis ont déjà plusieurs fois plus ou moins écrit de la même manière dans différents articles du ces aides à eau elle 300 213 toutefois, cet article stipule que lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé à compter de cette décision, jusqu'à la sortie de la zone d'attente, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ainsi que les frais de réacheminement incombe à l'entreprise de transport qu'il a débarqué en France il en est de même à compter de la décision de maintien en zone d'attente prises dans les cas prévus au 5ème alinéa de l'article L 221 et mes chers collègues, monsieur le ministre, je m'interroge sur la capacité des compagnies Air rien en particulier de bien évaluer le risque que comprendrait pour elle, ce type de disposition dans la loi, il ne faudrait pas qu'à titre préventif, elle se transforme en 2ème pas avant la PAF et refuse un certain nombre d'embarquement parce qu'elle supposerait que les personnes ne pourrait ne pas être acceptés sur le territoire, j'ai moi-même plusieurs fois vécu cette cette situation lorsque je me déplaçais vers les États-Unis et par conséquent, je voudrais Monsieur le Ministre, que vous nous précisiez si effectivement avec cet article-là, il y a un risque de voir finalement les compagnies aériennes se transformer en police de l'air et des frontières, de manière un peu discret. Donc dernière amendements à la discussion 395 rectifier Monsieur Bizet. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre d'État, Mécha collègue cet amendement vise tout simplement à supprimer l'article 57 bis article introduit par un amendement du gouvernement à l'Assemblée nationale cet article instaure une nouvelle redevance à la charge des compagnies aériennes visant à financer les frais de prise en charge des étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union auquel l'accès en France a été refusée, ainsi que les frais de réacheminement l'ensemble de ces frais est estimé par l'État à 7 millions d'euros par an, la création d'une redevance pour l'entrée, séjour des étrangers et du droit d'asile, telle que votée en première lecture à l'Assemblée nationale est une transposition du droit européen, il ne la remettrait donc pas en cause avant la mise en place de toute redevance, il serait souhaitable que soit proposée préciser 2 choses : tout d'abord une concertation avec les acteurs du transporteur du transport aérien, faire de du transporteur et du pavillon national un partenaire plutôt que contre chose vous le devinez tout simplement parce que les frais de transport vers les juridictions, les frais d'interprètes artistes d'interprétariat, l'entretien des bâtiments administratifs, voir les frais d'hébergement de demandeurs d'asile non présentait à l'avion, du fait du manque de diligence et de l'administration font partie des charges qui serait imputée au pavillon national et, deuxièmement, je crois qu'il faudra également des modalités de calculs, plus transparent, alors je sais que cela relève aussi d'une convention, la convention de Chicago à laquelle la France et est parti depuis un certain nombre d'années, je trouve qu'au travers de cet article 57 bis, la France s'était éloignés, voire affranchi de certaines règles de cette convention, c'est la raison pour laquelle j'estime que dans le cas du futur projet de loi asile et migration, il sera temps de revenir sur la participation de du transporteur national à ces opérations. Merci l'avis de la commission. Il s'agit là de de responsabilisé les acteurs des transports aériens, en l'occurrence, essentiellement et et là on peut pas être contre l'immigration et régulière et dédouaner la responsabilité, ce qui contribuerait la salle quoi concerne effectivement essentiellement les transporteurs aériens, mais d'une manière générale, ça vise à l'ensemble de la chaîne qui faciliterait l'immigration irrégulière et la responsabilité également pécuniaire, c'est pour ça que la commission, ce matin, a émis un avis défavorable sur cet amendement. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui défavorable, l'état de droit prévoit déjà à l'article L 213 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les entreprises de transport sont tenus d'assumer les frais de séjour des personnes étrangères qu'elles ont acheminé et qui font l'objet d'une décision de non-admission sur le territoire français, mais en raison d'une difficulté d'écriture, nous ne pouvons faire appliquer aujourd'hui cette nécessité, pour les compagnies de prendre en charge ces frais ainsi par exemple aujourd'hui à Roissy, c'est l'État qui est propriétaire des locaux héberge soigne nourris et assure la sécurité à ses frais des non-admis pour un coût total de 6,7 millions d'euros, donc nous voulons donc mettre fin à cette situation et donc avis défavorable à votre proposition.

Ne constitue pas une assurance de pouvoir entrer sur le territoire français et lorsque vous êtes ressortissant d'un pays qui est dispensé de cette obligation de VISA, ce n'est pas non plus l'assurance que vous pourrez rentrer sur le territoire et par conséquent, si on donne une responsabilité nouvelle aux compagnies aériennes. Alors qu'elles ont un pouvoir d'appréciation qui effectivement très large puisque le risque est énorme. Je crains tout simplement et je le dis, ça se voit déjà parce que les États-Unis pratiquent ce genre de choses, on risque d'avoir un certain nombre de refus d'embarquement arbitraire de la part d'un certain nombre de compagnies aériennes qui ne souhaiteront pas prendre le risque de transporter un certain nombre de personnes. Et, par conséquent, je pense que, en l'état actuel des choses, et compte tenu de l'absence de réponse concrète concrète de Monsieur le Ministre, nous dit : c'est dans ces États, mais aujourd'hui ce n'est pas applicable, donc il faut le rendre applicable, je comprends, ceci étant si effectivement c'est applicable telle qu'on le lit, je prends, je pense qu'on prend un risque trop important pour les, pour les compagnies aériennes et par conséquent, finalement on leur délègue la capacité d'estimer, au faciès, que la personne représente un risque ou non, pour elle, et il me semble que c'est abusif. Monsieur le ministre souhaite apporter aussi une réponse. Je rappelle que cette disposition est prévue dans la convention de Chicago, qui date de 1944 donc on voit que ce n'est pas quelque chose de nouveau, même si cela dans les dernières années n'étaient pas appliquées.

La séance est reprise. Donc, lors du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances adoptées par l'Assemblée nationale pour 2018 nous poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions : le Sénat va examiner maintenant les crédits de la mission, administration générale et territoriale de l'État et article 49 B.

j'ai le plaisir de vous présenter le budget d'administration générale et territoriale pour 1900 2018, qui s'élève à 2 milliards 700 57 une fois passées les rendez-vous électoraux, nous revenons à une situation correspondant au rythme de croisière d'une mission qui, c'est d'une évidence revendiquée comme telle n'est pas prioritaire, le projet de loi de programmation des finances publiques le confirme à retenir le simple maintien des dotations en valeur à l'horizon 2020, comme la mission a GTE, les moyens de l'administration générale de l'État dans les territoires qu'elles subissent une sourde réelégation budgétaire ne peut nous satisfaire, d'autant qu'elle subit des soupes juste budgétisation récurrente. Le programme 307 dans les crédits sont au niveau 2015 illustrent le manque d'attention portée à la mission, c'est-à-dire que rien ne s'est passé depuis, certes non, en application du plan préfecture nouvelle génération qui, avec la nouvelle directive nationale d'orientation des préfectures et sous-préfectures à ces dernières années, incarner les orientations de la gestion du ministère, les guichets du réseau préfectoral ont été fermés aux usagers. Dans la dernière décennie, le réseau des préfectures et les sous-préfectures, a perdu plus de 11 pourcent de ses moyens et la réforme des régions mais pour presque rien dans ce processus, ce sont les préfectures départementales et plus encore les sous-préfectures qui ont été touchés, la fin de l'accessibilité du réseau pour nos compatriotes, en particulier pour l'obtention des titres d'identité a pu être partiellement compensée par l'effort conséquent des mairies sélectionnés pour être les points d'entrée du système, mais dans le processus 2000 intériorisation qui presque achevée 33000 points d'entrée en mairie, ont dû être supprimés. Inutile de trop insister sur le fait que les emplois supprimés jusqu'à présent pas été raflés réaffecter au prix réel priorités fixées au réseau et qu'en particulier les moyens annoncés pour donner une nouvelle dynamique aux relations entre l'État et les collectivités territoriales, mais aussi pour améliorer l'animation des politiques publiques sur le terrain ne sont pas au rendez-vous, l'émission a été soit abandonné soit réduite dans leur ambition. Il serait utile que vous nous fassiez part de vos autres orientation stratégique pour le réseau, monsieur le Ministre, sans doute faut-il prendre en compte des événements et nécessité il y a l'accueil des étrangers ont mobilisé des moyens nouveaux, au demeurant très insuffisant compte tenu de l'augmentation des demandes adressées à la mi-station préfectorale et de la complexité de certaines situations, on peut en dire autant des besoins liés à la sécurité des Français, je relève que le projet de budget ne compte que 30 créations d'emplois sur c'était Matic, alors qu'il supprime 415 emplois temporaires temps complet dans le réseau des préfectures. Les créations d'emplois devraient être concentrés dans les services et devant les préfectures dans la tragique le tragique attentat de Marseille a pu illustrer certaines des incapacités. Progressivement privée de ses moyens, comme sont privés de leur les services de l'État et territoires de province en particulier territoires l'Euro, le réseau de l'administration générale de l'État a jusqu'à présent échappé à la fermeture, souvent redouté de trop de sous-préfecture néanmoins le 60 sous-préfecture soit doté de moins de 10 fonctionnaires en comprenant les contractuels temporaire de plus en plus nombreuses, constitue une évolution préoccupante. Quant au budget prévu pour informatiser ministère et pour pouvoir à l'entretien des bâtiments, il accuse une baisse importante, l'état des 1500 implantation du réseau et pourtant souvent mauvais et des collectivités territoriales qui en délègue utilisation mais aussi l'entretien à l'État en bien des motifs de s'inquiéter de son long de Bref, le projet de budget pour 2018 loin de dissiper le sentiment que l'État, c'est loin d'résolument hors du local, tant des usagers que des collectivités dans une ignorance totale des besoins mais aussi de l'intérêt que pourrait revêtir une politique d'aménagement du territoire abandonné au nom des prétendus plus- Value ajoutée par les grandes concentrations confirme des arbitrages à une métropolisation du pays la circonstance majeure pour le budget 2018, c'est la fin du cycle électoral de l'année en cours, elle entraîne la réduction des crédits du programme de 132 qui finance la vie politique, le financement de la vie politique de debout ne mobilisera qu'un peu moins de 100 millions d'euros l'an prochain, sur cette somme 68,7 millions d'euros iront formation politique en effet 26 virgule 3 millions serviront à combler le manque de crédit de 2017 cette enveloppe d'un pas été revalorisée depuis 2014, elle perd progressivement de sa consistance, c'est évidemment particulièrement vrai pour certaines parties du fait des résultats du scrutin 2017, par ailleurs, j'observe que l'extension de responsabilité conféré à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, par la loi, de confiance dans la vie politique ne trouvent aucune traduction budgétaire appréciable dans le projet de budget, enfin, je dirais, un dernier mot du budget en évoquant les frais qu'supportent au type d'administration centrale du ministère, c'est le programme de 116 j'observe qu'il va être lesté par la création de la commission du contentieux du stationnement payant mais que dans le même temps, le fonds interministériel de près leur sur la délinquance perd le quart de ces crédits le gouvernement explique qu'il doit mettre en oeuvre une nouvelle stratégie dans ce domaine, mais pour le moment, elle constitue surtout réaliser des économies sur les structures de réinsertion et de déradicalisation les dépenses de contentieux atteignent le sommaire 2017 à plus de 140 millions d'euros,

La parole est à monsieur Pierre-Yves Collombat, rapporteur pour avis de la commission des lois pour le programme administration territoriale. C'est le président ce nécessaire collègues je rappelle donc que la mission administration générale et territoriale de l'État rassemble donc les crédits de de 3 programmes scolaires vient des et de les énumérer l'administration territoriale qui regroupe les moyens des préfectures, sous-préfectures

vie politique culturelle et associative qui finance l'exercice des droits des citoyens dans le domaine des élections de la vie associative et de la liberté religieuse, comme ça a été dit, assez logiquement, on est plus en période électorale, il y a pas d'élections annoncées pour 2018, donc les crédits baissent n'a rien d'extraordinaire et le 3ème programme conduite et pilotage des politiques intérieure qui concerne le pilotage des fonctions dites supports en fait effectivement que le ministère dépense pour son fonctionnement, livrais mais je me limiterai à l'examen du programme le plus important administration territoriale si les crédits sont relativement stables par rapport à 2017 c'est la stabilisation d'une tendance longue à la restriction et surtout, surtout, la poursuite de la politique de réduction des effectifs de l'administration territoriale inlassablement conduite depuis plus de gouvernement en gouvernement moins 1300 postes ces 3 dernières années, et moins 4000 depuis 10 ans pour nos pas perdre cette mauvaise habitude, le ministre de l'Intérieur, ici présent, nous a annoncé un train de nouvelles réductions des effectifs de 350 emplois par an au cours des prochaines années, années, faut pas perdre de temps dans la version Bibliothèque rose du ministère de l'Intérieur, les réformes de l'administration territoriale qui suivent ces réductions d'effectifs depuis 10 ans, permettront de faire face et au-delà aux effets des hémorragies, dernière réforme en date, le plan préfecture nouvelle génération n'est pas arrivée à son terme que le 1er ministre vient d'annoncer la prochaine plus global action publique 2022 dont restent encore à définir les dispositions qui concernent l'administration territoriale, j'avoue que le la Story capacité d'adaptation des fonctionnaires, quel que soit leur statut fait mon admiration, reste à savoir jusqu'à quand cette situation pourra durer comme on le sait, des plans du plan préfecture nouvelle génération c'est la réorganisation complète de la délivrance des titres, cartes d'identité, passeport, permis de conduire, les cartes grises, la dématérialisation des procédures et des échanges entre les usagers entre les services entre les services préfectoraux et les collectivités territoriales, les gains de productivité ainsi dégagés sont donc censées compenser la baisse des effectifs : moderniser les procédures les sécuriser, faire en sorte que notre administration territoriale s'approprient l'outil informatique de plus quatre encourager, il serait stupide de se priver de tels instruments si c'est un moyen de renforcer la qualité de la présence de l'État républicain sur la totalité de notre territoire, pas si c'est un cache-misère pas si cela conduit à marginaliser un peu plus la population qui ne dispose pas d'un accès suffisant aux ou ou qui ne maîtrisent pas suffisamment l'outil informatique, constatant que, malgré les efforts, c'est encore trop souvent le cas surtout la présence de l'État, c'est d'abord celle de ses représentants, pas de la diffusion de leur image et et là, on est toujours loin du compte, quelles sont les raisons de fond pour lesquelles la commission des lois a émis un avis défavorable sur les crédits d'amis. et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de 10 minutes pour intervenir. Et je parole à Monsieur Hervé Marseille pour l'Union centriste 6 minutes. Monsieur le président, Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, avec 2 76 milliards d'euros de budget pour 2018, les crédits de la mission, administration générale et territoriale de l'État, recule de 11 pourcent par rapport à l'an passé, cette diminution, cela a déjà été dit et Prince il m'allemand imputables à l'évolution du programme 232 dans les dépenses sont liées à un cycle électoral qui, contrairement à 2017 sera a priori dépourvue d'échéances électorales majeures en 2018 la stabilité relative des crédits alloués à cette mission nous invite cependant Monsieur le ministre à la plus grande vigilance. Si, avec mes collègues du groupe Union centriste nous sommes favorables bien sûr à des mesures de redressement de nos finances publiques. Pour autant, nous demeurons attentifs à ce que cela se fasse pas trop au détriment du déploiement territorial de l'État au détriment de la complète information des Français en matière électorale, au détriment de l'accueil des usagers dans nos préfectures et sous-préfectures au détriment aussi et finalement de nos collectivités et de nos élus, le programme 307 relatif à l'administration territoriale est à cet égard révélateur, comme l'a fait remarquer, monsieur le rapporteur spécial des crédits restent au niveau de 2015, l'annonce du plan préfecture nouvelle génération et de la nouvelle directive nationale d'orientation des préfectures et sous-préfectures aura eu pour conséquence de supprimer 1300 emplois, soit 5 pourcent des effectifs de 2015, en disant : ce sont au total plus de 11 pourcent des employes du réseau d'administration générale de l'État qui ont été amputé la réduction des effectifs laissé près de 60 sous-préfecture doté de moins de 10 fonctionnaires, prenons l'exemple de l'accueil des étrangers, les dossiers afférents sont bien sûr toujours plus nombreux et plus complexe : la baisse des effectifs et des moyens ne contribue donc ainsi ainsi pas à garantir l'efficacité d'une mission pourtant étroitement lié aux conditions de sécurité du pays, autre exemple, celui de la lutte contre la fraude documentaire érigée en priorité par le ministère de l'Intérieur, je ne peux que rejoint des préoccupations de mes collègues de la commission des lois même interrogé sur les failles existantes dans la prévention de la fraude et la gestion parfois hasardeuse de fichiers qui ne sont d'ailleurs par ailleurs multiplié le programme 232 portant sur la vie politique, culturelle et associative voit ses crédits réduits de 344 millions d'euros, en raison de la fin du cycle électoral depuis 2014 l'enveloppe dédiée au financement des partis restée constante avec 68,7 milliards d'euros de crédit, nous avons tous pu constater la longueur des délais tenant au traitement des comptes et au remboursement des frais de campagne conviendrait à l'avenir, de permettre à la commission des comptes de disposer de crédits suffisants afin d'organiser une formation approfondie des personnels qui la rejoignent en année électorale, l'extension des responsabilités conféré à la Commission des comptes de campagne par la loi, de confiance dans la vie politique ne s'est malheureusement pas traduite par une augmentation de ses moyens, j'aimerais enfin Monsieur le Ministre, prendre quelques instants pour parler de la propagande électorale dans le projet de loi ne propose pas la dématérialisation mais dont on sait que la mesure deviendra très très prochainement à l'ordre du jour, vous connaissez l'attachement de la haute assemblée à la propagande papier et celle aussi de l'Assemblée nationale par ailleurs sur tous les bancs, nous saluons les avancées apportées par la modernité, bien sûr, mais encore faut-il respecter le principe d'égalité, il y a encore trop de zones blanches sur notre territoire entre population non reliés pour que la démocratie face économie de cette propagande papier il y a certes monde hyper-connectés, mais n'oublions pas une partie de nos concitoyens dans les zones rurales, alors que les dernières élections ont témoigné d'une abstention record, faudrait-il en effet accélérer le mouvement en cessant d'adresser aux électeurs les listes et professions de foi des candidats, c'est par souci démocratique Monsieur le Ministre, que nous saisissons cet instant pour vous demander d'être vigilants sur ce point nous indiquer et vous indiquer notre enfin le programme 216 sur la conduite et le pilotage des politiques de l'Intérieur appelle 3 remarques : d'abord, et malgré les rapports successifs, nous constatons que les dépenses contentieuse reste sous-budgétisé, ce qui provoque de nombreux dommages, il faut parfois attendre plusieurs mois pour qu'une décision de justice soit exécuté, ce qui n'est plus acceptable, enfin, la Cour des comptes a sévèrement critiqué l'action sociale au sein du ministère de l'Intérieur en pointant du doigt des situations inégalitaires préoccupante. Je voudrais vous manifestez enfin Monsieur le Ministre, notre inquiétude pour la révision à la baisse des crédits prévus au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance au moment même où le gouvernement entend développer une nouvelle stratégie ambitieuse de prévention de la radicalisation et de la délinquance, il est bien sûr dans notre groupe, coutume de voter cette mission et GTE et notre groupe le fera encore cette année, cependant nous souhaitons Monsieur le ministre est entendu et entendent de votre par les arguments du gouvernement sur l'essentiel des observations que je viens de vous exprimer, je vous remercie. Monsieur Marseille. La parole est à monsieur Éric Kerrouche pour le groupe socialiste et républicain pour 7 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à travers la mission administration générale et territoriale de l'État, le ministère de l'Intérieur, je cite, met en oeuvre 3 de ses responsabilités fondamentales garantir l'exercice des droits des citoyens dans le domaine des grandes libertés publiques : assurer la présence et la continuité de l'État sur l'ensemble du territoire de la République et mettre en oeuvre au plan local, les politiques publiques nationales : c'est en ces termes que l'annexe budgétaire introduit la présentation de la mission stratégique de la mission du PLF en débat à cet instant. Au-delà des 3 programmes qui constituent cette mission et sur lesquelles je vais revenir l'énonciation de ces trois responsabilité amène donc à questionner tout simplement l'les émission exercées par la puissance publique dans nos territoires et donc la place de l'État sur ceux-ci, ainsi que son articulation avec les acteurs locaux, alors certes, cette réflexion est censé être engagée dans le cadre d'un nouveau programme Action publique 2022, qui vient d'être lancé par le 1er ministre. Mais si une telle réflexion est loin d'être nouvelle, elle n'a trouvé jusqu'à présent comme réponse principale qu'une succession de réformes sans que l'on s'interroge réellement sur la mission et l'implantation de l'État dans les territoires et donc sur le rôle du réseau des préfectures et des sous-préfectures, ce sont bien les missions qui doivent déterminer les moyens et non pas l'averse en visant un égal accès à un service public de qualité, notamment pour les territoires les plus éloignées permettez donc que je développe 3 pour le 1er. S'adresse au programme 307 un état de proximité dématérialisé Métropolis et. S'agissant des moyens, des efforts importants ont été consentis en matière de rationalisation et de mutualisation, d'une part, mais également d'adaptation des préfectures et de leur personnel à la nouvelle carte des régions, d'autre part, au-delà des effets économiques de la reconfiguration géographique du réseau, il en ressort néanmoins souvent un sentiment d'éloignement, voire d'abandon des territoires de la part des usagers et des élus locaux qui voient une forme de démantèlement de l'État de proximité, à ce titre-si le plan préfecture nouvelle génération a permis ou devrait permette de moderniser l'administration et de simplifier la complète l'accomplissement pardon de démarches administratives pour les usagers, avec il est vrai, le concours non négligeable des mairies en ce qui concerne les cartes d'identité, il y a quand même lieu de s'interroger sur l'accès équitable de tous les usagers au service désormais dématérialisé. Je vous rappelle que la fracture numérique continue d'être une réalité pour plus de 3 millions de personnes et que tous nos concitoyens ne maîtrise pas de façon uniforme, les nouvelles technologies cette fracture numérique nécessite des moyens d'accompagnement dans les démarches de télé-procédure difficile à envisager dans le cadre de la réduction d'émissions de guichet ainsi la simplification et le progrès pour les uns, deviennent l'exclusion pour les autres, que ce soit pour des raisons géographiques socio-économiques ou générationnel dans cette perspective, il apparaît est essentiel de déployer des moyens pour le renforcement du dispositif des poids numérique permettant à tous les usagers de réaliser l'été, les procédures, l'objectif de 100 pourcent de services dématérialisés, d'ici 2022 fixé par le président de la République appelle une action budgétaires plus volontaristes, à la fois en matière de développement des services dématérialisés existant, mais également en investiguant de nouveaux champs pour cette dématérialisation étonnamment la mission administration générale et territoriale de l'État dans son programme 307 ne fait pas apparaître untel volontarisme en la matière, mais plutôt une curieuse contradiction lorsqu'il réduit les crédits alloués au fonctionnement et à la maintenance des matériels informatiques et des systèmes d'information, nous serons donc plus qu'attentif aux moyens qui seront mis en place pour qu'aucun usager ne soit exclu exclu, pardon, du service public dont l'État a l'obligation de garantir un égal accès à chacun d'entre nous. 2ème point des moyens limités pour exercer les missions des préfectures auprès des collectivités locales sur un autre plan, le P. PNG devait également permettre à l'État de se recentrer et de renforcer ses missions prioritaires dans l'expertise juridique, le contrôle de l'égalité et la coordination territoriale des politiques publiques, cela nous amène tout simplement à nous interroger sur le rapport de l'État aux collectivités territoriales et à sa mission de conseil inhérente à celle du contrôle de légalité pour que l'État soit ce qui est sans c'est être un co-constructeur est un facilitateur du développement des territoires cette réflexion apparaît d'autant plus importante suite à l'annonce du renforcement de l'ingénierie territoriale par le président de la République, d'une part et du dialogue de gestion par les préfectures, avec les collectivités locales dans le cadre des fameux contrats d'objectifs, d'autre part. En matière de contrôle de légalité, le PSG a permis la montée en puissance du pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité et le renforcement de la capacité d'expertise juridique par la création de 4 pôles et 2 à venir toutefois et dans le même temps on constate parallèlement un resserrement du nombre d'actes à transmettre au contrôle de légalité et une priorisation des actes à contrôler qui est inégal entre la préfecture, le rapport de la Cour des comptes de 2016 relève comme un facteur explicatif : le manque de temps de capacité d'expertise des agents et efficience de la procédure de transmission des actes dans cette perspective, la soutenabilité démission du réseau des préfectures pose question, tout comme la place des sous-préfectures dans l'architecture du réseau malgré une augmentation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement de 2,4 pourcent les moyens octroyés nous semble sous-estimer point 3, une limitation des moyens du Fonds amis interministériel de prévention de la délinquance. Bon dernier point porte sur la réduction sensible et moyens consacrés au fond à midi au fonds interministériel de prévention de la délinquance dans le cas du programme 216 de de 27 millions d'euros, cette baisse s'explique par la réduction du format des centres de réinsertion et de prévention de la délinquance dans le contexte de la mise en place d'une nouvelle stratégie pour autant ce fonds étant destinés à la à l'accompagnement des jeunes en voie de radicalisation et à leur insertion sociale l'actualisation de la stratégie interministérielle ne devrait pas se limiter à réaliser des Scud, des économies sur les structures de de réinsertion et de déradicalisation, dans le contexte que nous connaissons, ainsi pour les raisons évoquées précédemment qui relèvent principalement de la présence de l'État et de la perception de cette présence dans les territoires, nous ne sommes pas favorables au vote des crédits de la mission, administration générale et territoriale de l'État, je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, doté de 2,757 milliards d'euros en crédit de paiement, la mission administration générale et territoriale de l'État comprend 3 programmes poursuivant les objectifs diversifier et d'ampleur inégale, le programme 300 cette administration territoriale qui concerne principalement les moyens du réseau préfectoral 1 virgule 690 milliards d'euros, le programme 232 vie politique culturelle et associative finance essentiellement certaines expressions de la vie politique du pays 125 il y a 6 millions d'euros, le programme 216 conduite et pilotage des politiques de l'Intérieur est un programme réservoir qui moyens généraux du ministère de l'Intérieur et certaines interventions de ce dernier, c'est tout ceci pour un montant de 941 millions d'euros les dotations de la mission s'inscrivent en nette diminution, moins 349,6 millions d'euros, cette évolution en traduisant essentiellement la fin du cycle électoral chargé de l'année en cours, le projet de budget pour 2018 présente ainsi une très forte réduction des crédits qui recule de plus de 11 pourcent cette évolution est due au programme 232 dont les dotations diminuer de 344 millions d'euros, soit une baisse de 73 ainsi les économies de la mission, son toit attribuables au programme 232 dont les dépenses sont déterminées par le cycle électoral lourd d'événements 2017 et dénuée de rendez-vous significatif d'un point de vue budgétaire en 2018 je souhaiterais m'attacher au programme 307 qui rassemble les moyens des préfectures au commissariat, sous préfecture de métropole et d'outre-mer, ce programme avec le plan PPM j'ai voit ses crédits diminuer de 607309 euros en 2018 3 ans liée au plan préfecture nouvelle génération, il s'agit d'un recul, excusez-moi des services publics 415 emplois seront encore supprimés en 2018, portant à 1300 en 3 ans liée au plan préfecture nouvelle génération, les citoyens perçoivent une nette perte de qualité et de proximité du service rendu en préfecture et tout préfecture certains territoires très ruraux ne sont pas équipés d'infrastructure, ni d'internet toujours pénalisés car éloigné les sous-préfectures et dénuée de réseaux de connexions de qualité pour procéder aux démarches en ligne étaient les procédures en milieu rural, c'est généralement l'exclusion totale, l'État n'est plus un partenaire des collectivités locales et des prestations sont délégué souvent à des services extérieurs, heureusement que les collectivités sont là, malgré les promesses, l'État se désengage pour preuve dans le budget de cette mission après 2 années de baisse, moins 550 emplois en 2 ans et détective repartent à la baisse avec moins de 187 emplois en 2018 dans ce contexte budgétaire, les préfectures et sous préfecture peuvent-elles maintenir des équipes polyvalentes et capable d'assister les petites collectivités territoriales en matière d'engineering aussi, même si ce budget reste stable, je regrette que l'État ne fasse pas preuve d'une vraie volonté d'aller jusqu'aux confins de ces territoires oubliés aussi le groupe des indépendants s'abstiendra lors du vote sur les crédits de la mission, administration générale et territoriale de l'État, du projet de loi de finances pour 2018, je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Maryse Carrère pour le groupe RDSE pour une durée de 6 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre d'État, messieurs les rapporteurs, chers collègues, les grands chiffres relatifs à cette mission sont connus et en été rappelés, elle prévoit près de 2 8 milliards d'euros de crédits de paiement en baisse de plus tout d'abord le programme de 132 vie politique cultuelle et associative qui traite notamment l'organisation des élections et du financement des partis retranscrit le creux d'une année post-électorales sans scrutin je relève d'ailleurs à cet égard l'insuffisance de la subvention versée par l'État aux communes pour commencer pour compenser les frais engendrés par l'organisation des élections. à cette occasion je tiens également à rappeler l'opposition des membres du RDS au au projet maintes fois repoussé, Marietta dématérialisation de la propagande électorale une nouvelle tentative devrait être intégrées au projet de loi pour un État au service d'une société de confiance si nous mesurons l'intérêt d'une telle mesure durant en matière de maîtrise des coûts et à une pacte environnemental, elle ne permet pas un égal accès à tout ça, c'est information capitale. Le programme conduite et pilotage des politiques de l'Intérieur connaît quant à lui un léger fléchissement de ses crédits à 125,6 millions d'euros, parmi les mesures notables je peux relever la création de 119 TP pour traiter l'important contentieux du stationnement au sein d'une nouvelle commission dédiée induite par la décentralisation du stationnement payant prévue par la loi mais apte à monsieur le rapporteur spécial et monsieur rapporteur pour avis ont surtout relevé quelques étrange dans ce programme, notamment, des diminutions de crédits dans le cadre du plan de la lutte antiterroriste et du plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme ou encore une réduction des crédits affectés au fonds interministériel de lutte encore note Jean-Pierre au crédit du programme administration territoriale, le plus important, globalement stable à une virgule 7 milliards d'euros, il cache cependant d'importantes mutations à l'oeuvre depuis depuis plusieurs années, sur lesquelles je reviendrai l'actualité récente vient nous rappeler les implications dans le quotidien de nos concitoyens de cette mission, en effet, depuis le 1er décembre dans les préfectures et sous-préfectures les guichets pour la délivrance des cartes grises et des permis de conduire ont définitivement baissé le rideau, ils sont désormais remplacés par des procédures indignes, cet événement est une des dernières étapes de la mise en oeuvre du plan préfecture nouvelle génération lancée en 2015, il vise à recentrer les missions des préfectures autour de 4 priorités la sécurité et l'ordre public, le contrôle de légalité des collectivités, la lutte contre la fraude et la coordination territoriale des politiques publiques, une telle évolution rend également le lien qui unissait les citoyens à leur préfecture ou à leurs sous-préfecture, on peut se réjouir de la généralisation des télé-procédure car elles constituent des outils privilégiés de simplification des démarches pour la majorité des usagers et d'optimisation des moyens publics mais on peut également s'inquiéter de l'accès équitable des citoyens au service du réseau préfectoral, même si Madame la ministre pourra objecter que des points de contact numériques sont prévus dans chaque préfecture et sous-préfecture nous élus de proximité, comme vous d'ailleurs Monsieur ministre sont d'ailleurs sensibles à ces problématiques, d'autant que nous assistons sur le terrain aux conséquences des différents plans, dit de modernisation de la préfectorale, s'agissant des implantations que de la qualité de l'action de l'État, ces plans s'appelle aujourd'hui peine j'ai actualisé par la directive nationale d'orientation hier en les nommer RGPP ou réforme de l'administration territoriale de l'État demain leur succès de rang, le programme Action publique 2022 lancé par le 1er ministre le 13 octobre dernier il devrait se selon toute vraisemblance, poursuivre ce mouvement. Dans le présenter à la fin 415 au ETP sont supprimés au titre du PNG, principalement dans l'échelon départemental et infra-départemental, c'est ainsi que nous avons de plus en plus de sous-préfecture dans lesquelles travaillent une dizaine d'un tout au plus, même si la situation est contrastée selon les territoires, si jusqu'à présent, il n'y a eu que peu de fermeture, cette évolution s'apparente à une lente dévitalisation, à l'issue de ce plan : 1300 ATP auront été supprimés et dans le même temps, les crédits de personnel du programme 307 auront connu une légère augmentation, comme le souligne le rapporteur spécial, cette hausse ne peut être seulement expliqué par le protocole de parcours professionnel Carrière et formation dans l'application, a été reporté, ni totalement par la revalorisation du poignet à ce à ce stade, alors que le plan des peines Jesse achève, on peut s'interroger sur l'atteinte des objectifs qui lui était assigné si la diminution des effectifs qu'il prévoyait semble avoir été accompli, il n'est pas certaine que l'amélioration du service rendu aux particuliers, aux collectivités soient au rendez-vous, je pourrais par exemple évoquer les missions de contrôle de l'égalité et le conseil aux collectivités locales le présenter prévoit une enveloppe en hausse de 2 3 pourcent succédant à plusieurs exercices de baisse tendancielle, or et même si le périmètre du contrôle de légalité ont été réduit les moyens aujourd'hui affecté apparaissent clairement insuffisant pour l'accomplissement de ses missions, je pourrais tout aussi bien mentionné la délivrance des titres sécurisés leur gestion de plus en plus dématérialisés, a-t-elle permis de diminuer la fraude documentaire de réduire les délais et les coûts de fabrication à ce stade, la réalité semble bien plus grande contrastée qu'attendu, j'en profite pour relever que le montant de la dotation pour les titres sécurisés, bien que réévalué à l'article 62 du PNF demeure loin de compenser les dépenses engagées par les communes, au final, cependant, et malgré les réserves que je viens de présenter les membres du groupe RDSE voteront les crédits de la mission, administration générale et territoriale de l'État. La La parole est maintenant à monsieur Pierre Yves Collombat pour le groupe communiste, républicain, citoyen écologiste pour 5 minutes. minutes. Il a un minute chers collègues monsieur le président, mettant, vous l'avez vu par nécessité sur le côté strictement budgétaires de la mission et la poursuite des réductions d'effectifs qui il implique, je reviendrai maintenant sur quelques-uns des aspects qualitatifs de cette évolution réorganisation de la vie France des titres 1er point la mise en place, DC ERT que les demandes de titres faites par les administrés dans le département ne sont désormais plus traités par les services de la préfecture de ce département, selon le titre concerné, la demande est transmise à un CRT Centre chaque centre étant spécialisée sur un type de titres chaque département dépendant de plusieurs CRT 58 CRT délivrent désormais les cartes d'identité, les passeports, les permis de conduire et les cartes grises, les compétences des objectifs de production, les départements servi les moyens dont dispose chaque CRT dépendent largement de l'importance des effectifs à réaffecter concurremment à d'autres options promotions internes : départs à la retraite, mise en place de pôles départementaux, spécialisée dans la sous-préfecture importante, félicitons-nous que le volontariat des éventuelles migrations géographiques aient été et heureusement prévalu pour donner un exemple de cette organisation, le C. que nous avons visités à Châlon-sur-Saône en Champagne traite avec un effectif de 20 équivalents temps plein, les demandes de permis de conduire de 5 département la Meurthe-et-Moselle, les Deux-Sèvres, la Haute-Marne, le Lot, Hautes-Alpes. 2ème point les problèmes liés à la dématérialisation obligatoires, des demandes cette modernisation de la délivrance des titres par ailleurs souhaitables représente comme on l'a dit et en même temps un nouvel éloignement des services de l'État, c'est aussi une nouvelle charge pour les collectivités territoriales s'agissant des nouvelles modalités de demande de carte d'identité, ce sont désormais 2300 communes qui assume la resp la réception des demandes au lieu de 35000 ce qui ne satisfait ni les usagers des zones éloignées de ces points de contact ni les maires qui doivent assumer la tâche : l'augmentation de la compensation de 3500 euros par dispositif avec un supplément pour les plus actifs, soit un impact budgétaire de 17 millions devrait répondre en partie à leur attente, j'ai déjà évoqué le pour les problèmes techniques, une qualité insuffisante du réseau et psychologique, une maîtrise minimale de l'outil informatique, mais force est de constater que même là où les réseaux sont suffisants ou les points d'accès supplémentaires sont accompagnés, où le personnel est ouvert à la nouvelle approche des problèmes embarrassants continue de se poser ainsi à la préfecture de la Marne, par ailleurs, les choses se sont globalement bien passé, nous a-t-il été rapporté qu'une partie non négligeable des usagers vivait comme une discrimination à leur endroit, le fait qu'il ne puisse bénéficier d'un accueil par un agent alors que ce n'est pas le cas, écoutez bien, pour les titres de séjour des étrangers. Réaction évidemment non mais qui en l'espèce, en dit long sur le sentiment d'abandon par l'état des administrés, comme quoi les réformes apparemment les plus rationnels que avoir des coups politiques à soupçonner le fichier TER, cette réforme a aussi justifié la création du fichier TER, ce qui a entraîné de nombreuses réactions, l'audit de ce fichier, que le ministre de l'Intérieur avait demandé à la suite des réactions des parlementaires, on se rappelle l'audition du ministre de l'intérieur par la commission des lois du Sénat, a conclu que la sécurité du système n'était pas parfaite et que celui-ci pouvait être détournée à d'autres, à des fins d'identification, le ministère nous a dit avoir Dupouy pris en compte les recommandations du rapport si on a vu, on est si on n'a aucune raison de ne pas le croire, il n'en demeure pas moins que ce fichier n'est pas le plus sûr possible en l'état des technologies, les sous-préfectures, la réforme des ce profile de leur implantation, attendue depuis longtemps, a finalement été très limité finalement le plus important, c'est ce qui a été fait c'est finalement faire coïncider les ressouder les limites des arrondissements avec avec les intercommunalités qui ont beaucoup bougé, comme vous le savez, mais au-delà de la carte des sous-préfectures. Il conviendrait de redéfinir et d'adapter les moyens pour leur permettent de remplir comprennent concrètement leur rôle de proximité. Vie politique culturelle et associative, je terminerai par là principal chantier la réforme des modalités d'inscription sur les listes électorales à la mise en place prochaine du répète dupés répertoire électoral unique les 2 opérations sont en bonne voie, quoi qu'il ne serait pas inutile de rappeler aux communes arrive une réforme va prochainement modifier l'inscription sur les listes électorales, s'agissant de la dématérialisation de la propagande électorale gouvernants qui semblent décidés à contourner le Parlement, une 4ème fois par le biais d'une demande d'habilitation à légiférer par ordonnances dans la future loi pour un État au service d'une société de confiance et bien finalement il y a renoncé, reste à savoir pendant combien de temps comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pensant pas que l'on puisse se satisfaire de cette politique récurrente de retraite, l'état des territoires, suivant l'avis de la commission des lois, notre groupe ne votera pas les crédits de la commission de la mission acte. La parole est à monsieur Marc Laménie pour le groupe, les républicains pour une durée de 8 minutes maximum. Monsieur le président, Monsieur le ministre d'État, mais sur rapporteur rapporteur spécial, rapporteur pour avis Monsieur le président de la commission des finances, chers collègues, je voudrais bien entendu lui donc le travail de nos reporteurs partager avec l'ensemble des personnels des commissions et de notre institution, dans le cadre de la loi de finances pour 2018, les crédits de la mission, administration générale territoriale de l'État s'élève à 2 7 milliards d'euros, qui regroupe 3 programmes, comme cela a été rappelé, alors je reviens sur quelques chiffres tout d'abord le programme 307 l'administration territoriale 1,69 milliard d'euros avec une stabilité des montants financiers et sur lequel je reviendrai plus on détaille le programme 232 dit quelques mots : vie politique que cultuelle et associative qui regroupe tout ce qui est lié principalement aux organisations des élections en 2017 il y avait quand même 4 dimanche concernés, donc d'où l'importance du montant financier en 2017 et c'est sûr qu'en 2018 ce montant baisse à hauteur de ici élève à 125 millions d'euros, soit moins 73 pourcent donc avec différents engagements aussi pour la vie politique, commission des comptes de campagne notamment, en particulier le programme de son 16 941 millions d'euros, a aussi une certaine stabilité donc principalement l'administration centrale, sous votre autorité, le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre d'État État-Major et services sont trop qui est-ce élèves 373 millions d'euros, mais globalement, cette mission a GTE et surtout une mission d'effectifs, d'où le rôle important des moyens humains en soulignant naturellement le dévouement de l'ensemble des personnels qui oeuvre aussi avec dévouement ce agissons du projet de budget de l'administration territoriale, les crédits de paiement sont inégalement répartis réglementations générales, garantie de l'identité et de la ne nationalités, il y a aussi l'automatisation avec la numérisation du processus de délivrance des titres sécurisés ou si un un sujet important au niveau de la délivrance D D des titres et le montant pour cette partie, c'est quand même 688 millions d'euros, le pilotage des politiques gouvernementales à hauteur de 514 millions d'euros, la coordination de la sécurité des personnes et des biens, 172 millions d'euros de la légalité, notamment j'en dirai aussi quelques mots à hauteur de 153 millions d'euros, sans oublier l'animation et le soutien des réseaux nous assistons depuis plusieurs années à une baisse des effectifs re re, réduction des effectifs de 2007, 2017 avec moins de 3357 équivalent temps plein 11 pourcent des effectifs en moins et les effectifs s'élèvent un peu près 26000 emplois pour 2018 on assiste malheureusement aussi à une baisse dès ses effectifs et ces réductions d'emploi toucheront principalement le Chlons départementale, nous restons très attachés à l'administration préfectorale, les préfets, sous-préfets et leurs services leurs services joint rôle important dans l'eau, territoire les représentants de l'île étant sur les Terres aussi pour beaucoup de nos collègues sont les interlocuteurs des élus locaux, interlocuteur du monde économique, sociale, de l'éducation nationale, de la santé, également en liaison avec les agences régionales de son service public de proximité aussi Roland portant en liaison avec nos 3 fonctions publiques : État, territoriale et hospitalière, des sous-préfectures, a évolué dans beaucoup de de départements comme la carte aussi des intercommunalités, celle de nos départements respectif, ce n'est pas simple dans le département des Ardennes que je représente une préfecture Charleville-Mézières reste 3 sous-préfectures, ce nom, Rethel et vous y donc avec aussi des des moyens humains très variables d'une sous-préfecture à l'autre, je tiens aussi à le dire, mais c'est vrai qu'en terme de de points de contact de proximité, nous y sommes attachés et aussi avec l'évolution à la mise en place d'une maison de l'État et des maisons de service au public, ces réductions d'effectifs, moins de moyens humains, malheureusement nous inquiète beaucoup, ça l'était, il vous crier aussi avec le regroupement ou des régions, réduction des effectifs au niveau des des égards s'agissant du contrôle de la légalité du conseil aux collectivités territoriales qui c'est action est réellement historiquement le coeur des métiers, on a vu aussi malheureusement une très forte baisse des moyens humains jusqu'en 2016 la semaine dernière dans cette hémicycle lors de l'examen de la mission, relations avec les collectivités territoriales depuis représente 3,6 milliards d'euros, nous avons largement évoqué les Liens de confiance entre les élus locaux, départementaux également régionaux, l'ensemble des des élus avec les représentants de l'État comme ancien maire d'une petite commune 170 habitants jusqu'au mois de juin dernier, je peux modestement témoigner, c'est vrai que les services de la préfecture et sous-préfecture pour l'établissement des déclarations de récupération de TVA ADF, c'était je pense est exemplaire : le financement des investissements pour le soutien à l'investissement, anciennement le DGE la des aujourd'hui le fil également aujourd'hui les représentants de l'État suivent également naturellement suivez la gestion de la réserve parlementaire dont nous regrettons beaucoup ici la disparition puisque la dotation d'action parlementaire était parfaitement en encadré, vous nous avez nous, les dernières notifications nous on nous vous en remercions monsieur le ministre d'État pour la réserve parlementaire et localement, c'était quand même suivi par les services préfectures et sous-préfectures, nous restons très attachés à cette présence de l'État, rôle déterminant pour la sécurité, un, c'était un peu dans l'émission précédente la mission sécurité police nationale Gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers, la mise en place de la police de sécurité du quotidien, c'est aussi un enjeu important au niveau des représentants de l'État et puis j'aime oublie pas non plus de citer le rôle important des représentants de l'État, dont les actions dans le cas du devoir de mémoire cérémonies patriotiques nationales et locales, soutien aux associations patriotiques et de mémoire, au vu je dirais de ces différentes observations que je partage naturellement avec les différents collègues qui se sont exprimés sur cette mission réellement important de la présence de l'État sur notre territoire respectif soutiendra suivra la vie de notre commission des finances et adoptera les crédits de cette mission, je vous remercie. La parole est à monsieur Julia, un Bargeton pour le groupe, la République en marche pour 6 minutes. Oui. Chers collègues, je remplace au pied levé Alain Richard tire c'est user je voudrais essayer de faire passer les messages qu'il aurait sans doute voulu vous faire passer d'abord derrière intitulé technique cette mission cache 3 missions extrêmement importante, l'exercice de des droits des citoyens, la continuité de l'État sur le territoire et la déclinaison sur le plan local des politiques publiques, c'est ça, cette mission d'administration générale et territoriale de l'État, elle est marquée, cela a été souligné par notamment le plan préfecture nouvelle génération qui est l'élément le plus important, c'est une réforme qui répond aux enjeux d'accessibilité et de modernisation de des usagers enfin attendue par les usagers et qui s'appuie sur 2 piliers essentiels d'abord dématérialisé, ça c'est le premier et puis mettre en place un réseau de centre d'expertise et de ressources Titre qui permettra d'accélérer la délivrance d'un certain nombres de titres si le programme 307 qui traduit en quelque sorte ce plan préfecture nouvelle génération et dont on peut relever d'ailleurs que certaines des actions progressent certes certains orateurs ont ont souligné évidemment les économies, c'est vrai que ce plan se traduit par une des volontés de réaliser des économies sur les fonctions support du pays du territoriale par la mutualisation c'est le principe d'une modernisation et ça c'est plutôt souhaitable mais les actions, les actions 3 progresse et d'ailleurs l'action 3 qui correspond au contrôle de légalité est évidemment extrêmement importante et aller en progression, le 2ème sujet c'est les conduites et la pilotage des des politiques de de l'intérieur, c'est évidemment ce programme qui porte les les fonctions d'État-Major un de ce type de cette mission, c'est-à-dire les fonctions centrales là aussi avec une volonté d'en renforcer la cohérence à à travers plusieurs sujets bien sûr notamment en en mettant en oeuvre un certain nombre de, de, de projets, comme sur la la les la prévention de la délinquance ou encore l'amélioration de l'efficience des fonctions support voilà donc un certain nombre d'éléments et puis bien sûr, le programme de 16 est aussi celui, je terminerai par là, qui porte la la stratégie immobilière de l'État, monsieur le président, on a vu déjà dans l'immeuble Garance dans le 20ème arrondissement qui a permis d'accueillir un certain nombre de de services et cette stratégie immobilière se poursuit, s'est poursuivie sur plusieurs îlots bien sûr l'îlot au bout l'îlot Beauvau et se traduit par un schéma pluriannuel de travaux 2016 fin de de du 16 2018 et qui permettra de de compléter des éléments aussi de mutualisation via les stratégies immobilière qu'il faut soutenir donc pour ces 3 raisons, la modernisation, la stratégie immobilière et le le renforcement d'un certain nombre de de mesures, le groupe la République en marche votera les crédits de cette mission, je vous remercie. Merci, parole est maintenant à monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur pour une durée de 10 minutes. Monsieur le président, monsieur le rapporteur spécial, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames et messieurs les sénateurs, la mission administration générale et territoire de l'État. Qui comprend en particulier le budget, les préfectures et celui de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Présente pour 2018 des crédits consolider et préserver, si l'on met à part le budget consacré à l'organisation. Selon les élections qui ont évidemment été nombreux en 2017 avec 2,1 milliards de crédits, le budget et la mission que je présente aujourd'hui devant vous est stable, cela a eu évidemment pas toujours été le cas dans le passé un certain nombre d'entre vous ont fait allusion prend Real et puis aux suppressions de postes qui avait pu être réalisé et c'est vrai qu'entre 2010 et 2017 il y a eu des suppressions de postes extrêmement nombreux, nous avons voulu stabiliser les choses car les missions accomplies par le réseau préfectoral sont à mes yeux, extrêmement important, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que le budget des préfectures soient préservés avec 1,22 milliards de d'euros de crédit ce budget. Prévoit certes certaines réductions d'emplois, mais elles sont largement permise par la mise en place du plan préfecture nouvelle génération décidée en décembre 2015, cette réforme repose, comme vous le savez, sur la numérisation des procédures de délivrance de titres et sur leur simplification, elle a permis de réinjecter 1000 agents sur les missions prioritaires des préfectures, la mise en oeuvre de cette réforme est d'une grande actualité puisque de nouvelles télé-procédures concernant les demandes de carte grise et le permis de conduire, viennent d'être déployés, je dois dire que je m'interrogeais un peu sur la façon dont les choses se passeraient parce qu'évidemment des réformes nouvelles comme celle-ci sont toujours un peu délicat, or le nouveau système, même si, ici ou là, il y a pu avoir quelques grippage semble fonctionner en novembre 2007 885198 cartes grises ont été édités, et 2000 286255 nouvelles immatriculations ont été comptabilisés, soit 3 pourcent de plus qu'novembre 2016 nous avions un certain nombre de problèmes avec donc les importateurs de voitures étrangères avec certains professionnels de l'automobile, nous venons de les régler, je crois que cet après-midi même, nous avons signé un protocole d'accord avec eux ainsi les problématiques semblent se régler, donc nous avons également dans ce plan, une nouvelle génération, la nouvelle organisation de l'instruction des demandes de titres qui se fera donc dans les centres d'expertise et de ressources tit dit compteront 15, sans emploi, 27 pour laisser passeport 21 pour les permis de conduire, dont 2, spécialisé dans l'échange de permis 6 pour les cartes grises et enfin 3 CRT polyvalent outre-mer je rappelle à ce sujet qu'en ce qui concerne les cartes nationales d'identité 22 millions d'euros oui était dégagée dans le PLF pour accompagner les communes dans la mise en place de la réforme au travers de la dotation titre sécurisé sur les moyens technologiques, nous, on nous avait dit mais ce qu'il y a véritablement une sécurisation comme vous le savez, des demandes sont maintenant traitée avec le fichier texte ce qui a pu susciter des inquiétudes, mais nous y avons répondu en particulier à toutes les observations, il y a une vérité faite par là même si, en renforçant la cryptographie et la protection contre les risques d'intrusion par exemple dans le cadre du nouveau plan que souhaite le 1er ministre action publique. 2022, nous voulons lancer une réflexion plus globale sur l'administration territoriale de l'État, il s'agit pour nous d'abord de mutualiser un certain nombre de fonctions supports de se poser la question de la fusion de certains programmes budgétaires, voire de la réforme de l'échelon départemental de l'administration territoriale de l'État, de manière à ce que les préfets disposent de leviers plus efficace pour assurer la gestion de l'administration, je recevais hier les préfets et les sous-préfets et on leur a indiqué. C'est ce que devait être le coeur de leur mission animée effectivement avec les collectivités locales, l'ensemble des territoires qu'il soit urbain ou qu'il soit ruraux, effectivement cela, monsieur le rapporteur ah. Toute son importance : bah, par ailleurs, au-delà des missions prioritaires du plan préfecture nouvelle génération, ce budget permettra de renforcer les services des étrangers de la ville, comme je l'ai indiqué tout à l'heure avec 150 recrutements de personnels titulaires pour ce qui concerne les crédits de l'administration centrale 795 millions d'euros sont prévus, c'est-à-dire un budget stable avec une réduction de 35 emplois par rapport à 2017, car évidemment l'administration centrale doit elle aussi participer aux efforts d'économie 4 faits sont cependant à signaler d'abord des crédits qui sont inscrits pour l'installation et la sécurisation d'un 3ème site pour la DGSI à Neuilly, en attendant la réalisation d'un site unique sur lequel nous sommes en train de réfléchir ensuite le budget comprend une forte augmentation des crédits de contentieux en effet par le passé, ces crédits se sont trouvés notablement insuffisants, ce qui a conduit les parlementaires, a qualifié les Budgets d'insincère nous passons donc de 55 millions d'euros en 2017 à 80 millions d'euros en 2018, ce qui reflète davantage la réalité des besoins, vous savez que c'est là le souhait du gouvernement d'avoir dans tous les domaines, une plus grande sincérité budgétaire enfin pour ce qui concerne la stratégie de prévention et de radicalisation, la baisse des crédits, comme vous le savez, est due à la fermeture du centre de pont qui, qui, comme vous le savez, avait été un échec. Que parce que nous n'avions pas pu réaliser ce qui avait été initialement prévu et donc nous avons fermé se sentent nous réfléchissons également en ce moment sur la répartition des crédits à certain nombre de crédits ayant été donnée par le passé à un certain nombre de d'associations un peu auto-proclamé donc leader dans le domaine de la. Des radicalisation et nous souhaitons davantage travailler sur le terrain, nous aurons donc l'occasion de vous faire de nouvelles propositions, enfin les crédits de cette mission permettront de financer la mise en place de la juridiction spéciale chargée du contentieux des forfaits du stationnement payant qui accompagnera l'entrée en vigueur au 1er janvier prochain de la réforme de la décentralisation du stationnement payant 119 ETP, 8 millions d'euros de budget sont ainsi prévus pour armer cette juridiction qui sera établi comme vous le savez, à Limoges, c'est un acte de décentralisation qui avait voulu le précédent gouvernement, voilà, Mesdames et messieurs, pour ce qui concerne l'ensemble des crédits de cette mission. Merci monsieur le ministre, nous allons donc procéder au vote des crédits de la mission, administration générale et territoriale de l'État figurant à l'État, mais je n'ai été saisi d'aucune demande explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets donc on voit les crédits de la mission qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Les crédits sont eux adopté. J'appelle en discussion à l'article 49 B, qui est rattachée, pour son examen au crédit de la mission, administration générale territoriale de l'État, je mets au voilà 49 B qui est pour. Qui est con. Qui s'abstient l'article est adopté. J'appelle en discussion maintenant l'amendement tendant à insérer un article additionnel, qui est rattachée, pour son examen au crédit de la mission, administration générale était de l'État, monsieur Dominati votre amendement 393 vous le défendez. Oui, monsieur le président, Monsieur le président, Monsieur le Ministre d'État avant dimanche le présenté il y a déjà j'ai eu l'occasion de l'Euro défendre au cours de la loi de moralisation de la vie politique et comme il, il, il concerne la liberté de tous les parlementaires et notamment parce que la France a choisi le système de financement de la vie publique par le financement public, vous savez que nos partis politiques bénéficient essentiellement de la manne de l'État pour développer leur vider leurs actions, leur programme, leur projet et tous les parlementaires doivent faire le mois de novembre, ça s'est produit il y a quelques jours, choisir sur une liste 11 partis politiques, ceux qui ont présenté des candidats dans un certain nombre de départements en France pour bénéficier de la manne publique, il y a une sorte de monopole des grands partis qui peuvent se partager cette dotation financière l'année 2017 a été veut paradoxal sur ce plan puisque nous avons vu d'une part un candidat non issu des partis politiques, devenir président de la République et puis je dirais les partis traditionnels du gouvernement malgré le financement public ne pas gagner les élections législatives et un parti au contraire devenir majoritaire à l'Assemblée nationale et surgir somme aucune aide publique le président abonnement a pour but de laisser d'abord la liberté de choix des parlementaires s'ils sont par exemple l'indépendant divers droite ou divers gauche de ne pas choisir, parce que c'est un parlementaire ne choisit pas sa dotation pour autant est partagée par les 11 formations qui peuvent du coup se partager cette dotation, et il est tout à fait naturel à mes yeux qu'un parlementaire puisse dire le plus naturellement du monde qui leur reverse sa dotation au budget général, ce qui permettra de contribuer à amoindrir le déficit public, c'est l'objet, monsieur le président, Monsieur le Ministre d'État de cet amendement et j'espère que malgré la technicité qui on n'arrive pas toujours nécessairement à comprendre, il sera adopté après un long cheminement.

tout d'abord je voudrais quand même féliciter aussi Hervé Marseille, ancien rapporteur pour son rapport qui m'a bien aidé dans le travail, dans cette mission, alors au sujet de l'amendement de monsieur Dominati, qui a déjà été voté par le Sénat, la commission des finances, a donné un avis de Serge très favorable et antipersonnel je voterais pour.

dans ce gouvernement, hé bien pour lui démontrer qu'il y en a, puisqu'il avait présenté 3 fois cet amendement, cette fois-ci le gouvernement sera favorable. Donc, je fais le point, je ne connais pas la vie sagesse très favorable, donc c'est sagesse, pour la Commission. Sagesse. Le gouvernement est favorable, qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, cet amendement est adopté, nous avons fini la discussion des crédits de cette mission je vais suspend la séance, elle sera reprise.